La parole est à monsieur Damien Régnard pour une mise au point, au sujet d'un vote. Oui bonjour. Merci Monsieur le Président, je souhaite faire une mise au point, au sujet d'un vote lors du scrutin, numéro 125 du 7 février 2023. J'ai été considérée comme votant pour le texte, je souhaitais en réalité voter contre ce texte. Je vous remercie de prendre en compte cette modification. Merci cher collègue. Et la parole est à monsieur Olivier Henno également pour une mise au point, au sujet d'un autre. adoptée à l'Assemblée nationale visant à réhabiliter les militaires fusillés pour l'exemple. Durant la première guerre mondiale et monsieur Jean à voter contre. Ils souhaitaient voter pour. Je vous remercie. Merci, cher collègue, acte et donner de ces mises au point figureront dans l'analyse politique des scrutins concernés. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. Dans la discussion générale la parole et sans tarder à Madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. On compte aujourd'hui près de 1000 centres dentaires sur le territoire français. Leur nombre a progressé de 60% en l'espace de 5 ans. La tendance est similaire pour les centres de soins ophtalmologiques de 88 en 2015, la Caisse nationale d'assurance maladie en recensait 157 en 2020. Le développement rapide et soutenue des Centres de santé à travers notre pays nous impose une double exigence. D'une part car je suis une optimiste, je les vois, je vois les opportunités à saisir. Nous devons soutenir ce modèle d'exercice collectif, de la médecine qui est de nature à améliorer l'accès aux soins pour nombre de nos concitoyens. D'autre part avec réalisme. Il nous faut lutter avec intransigeant intransigeance contre les dérives gouvernement et législateur, il est de notre responsabilité de créer le cadre légal permettant un développement éthique et encadrer des centres de santé au service de la santé des Français. C'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Je tiens à avoir un mot pour Madame la députée Fadila Khattabi, présidente de la commission des affaires sociales qui est à l'origine de cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Je salue également monsieur le rapporteur Jean Sol et les commissaires aux affaires sociales du Sénat pour leur travail en commission. Du fait de leur important écho médiatique et de l'émoi légitime qu'ils ont suscitée dans la société, nous avons tous été marqués par les scandales impliquant les centres de santé Dentexia et proxy dentaires. Il y a eu des manquements évidents et répété à la qualité et à la sécurité des soins. Il y a eu aussi certes plus rarement des choses assez grave pour conduire à des chefs d'accusation de violences volontaires de mutilations volontaires et qui ont entraîné chez les victimes des infirmités permanentes. Je pense également au fléau de la fraude des surfacturations des sur traitement et multi-facturation. Le 23 janvier dernier encore de centres de santé dentaires et ophtalmologiques dans les Yvelines et en Seine Saint-Denis, ont été déconventionnés par la sécurité sociale. Le préjudice pour l'assurance maladie s'élève à 1,5 millions d'euros. C'est un coût important pour nos finances sociales mais surtout un autre coup pour les usagers qui sont aussi les victimes de ces pratiques tarifaires frauduleuse. Ce que je vous décris est d'autant plus choquant que ces centres de santé ont généralement abusé de la confiance de patients précaires qui voyait en ces structures une solution à leurs difficultés d'accès aux soins. Je pense aussi au témoignage d'un retraité qui n'y ont pas eu les moyens de payer les 3400 euros qu'un centre-dentaire lui. Pour remplacer ces six Sidan arrachées sans nécessité a perdu la capacité de s'alimenter normalement et une partie de sa dignité. On m'a volé une partie de moi. Ces mots nous oblige. Face à l'ampleur de la situation, le gouvernement a rapidement réagi l'ordonnance du 12 janvier 2018 a permis sans attendre la mise en oeuvre de premières avancées concrètes pour contrôler davantage les conditions d'ouverture et de fonctionnement de ces centres. Nous avons également consolider l'arsenal de notre système de santé en matière de lutte contre la fraude sociale. Ce qui nous a, ce qui nous permet notamment en cas d'infraction grave de déconventionner ces Centre beaucoup plus rapidement. Pour ancrer et renforcer cet encadrement nécessaire des mesures avaient été travailler dans le cadre du budget de la Sécurité sociale pour 2022, avec notamment la création d'amendes administratives. C'est l'Union des différentes forces de contrôle qui nous permettra d'être efficace. Ainsi en oeuvrant vos derniers 10 centres de santé dentaires dans 10 régions ont fait l'objet d'une inspection de contrôle par les agences régionales de santé conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie, les services d'inspection du travail et les services fiscaux. Cette inspection de contrôle a également bénéficié du soutien de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude. Cette proposition de loi nous donne aujourd'hui l'occasion de concrétiser ses mesures pour toujours mieux sécuriser les prises en charge et assurer la qualité des soins à tous nos concitoyens. Mesdames, et messieurs les sénateurs et sénatrices notre objecter premier avec François Braun et de lutter contre les inégalités d'accès à la santé. L'accès à la santé est une préoccupation majeure qui est au coeur de notre action. Je le dis ici devant vous, car c'est un objectif que je sais partagée par votre hémicycle et parce que c'est aussi de cela dont il est question aujourd'hui. En effet dans un contexte de tensions sur l'offre de soins. Les difficultés d'accès à la santé, touche l'ensemble du pays et un pacte en 1er lieu les plus fragiles. Pour beaucoup de nos concitoyens, les centres de santé qu'il soit urbains ruraux ou dans les quartiers prioritaires de villes sont reconnues comme des lieux qui leur permettent d'accéder facilement et rapidement à des soins. Avec 2400 structures à travers le pays, qui rassemble 38.000 professionnels, leur présence au coeur des territoires répond à cet objectif de responsabilité populationnelle qui nous est cher. Ce sont également des structures collectives. Répondant à l'aspiration des professionnels en particulier des jeunes permettant de rompre avec l'exercice isolé et que le gouvernement soutient et encourage pleinement. Si les dérives sont graves est toujours inacceptable. J'ai pu le décrire. Elles sont fort heureusement minoritaires et je ne veux pas jeter l'opprobre sur ce modèle. La multiplication des centres dentaires et ophtalmologiques permet avant tout de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens au plus près de ses besoins. Aussi j'envisage le fait de lutter avec fermeté contre les deux rives et de créer un cadre législatif adapté comme le meilleur moyen de soutenir le développement de ces structures d'accès à la santé. Car réguler c'est redonner confiance aux Français dans les centres de santé car encadré c'est assurer des opérateurs fiable pour garantir la qualité des soins. Mesdames et messieurs dans la poursuite de cet objectif. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui prévoit des dispositions légitime et équilibrée. La logique d'agrément sur laquelle nous avançons permet de renforcer la démarche du projet de santé autour de laquelle doivent être construits les centres de santé dentaires et ophtalmologiques. L'agrément envisagé au niveau régional, permet également d'inscrire les structures dans un projet territorial plus large définies localement par les ARS. La qualité des soins sera garanti grâce à la transmission et à la vérification des Duplo mes contrats de travail des chirurgiens dentistes. Assistant dentaire ophtalmologistes et orthoptistes dans le dossier de demande d'agrément. Comme à chaque nouvelle embauche. Nous ne transigerons pas avec la sincérité de la gestion financière en actant l'obligation de certification des comptes par un commissaire et leur transmission aux ARS. Nous nous donnerons les moyens de procéder plus largement à des contrôles et vérifications notamment durant la première année puisque l'agrément délivré ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période de 12 mois. Les sanctions seront parallèlement renforcées avec des amendes pouvant aller jusqu'à 500.000 euros en complément d'éventuelles sanctions pénales pour les cas les plus graves. Sur proposition du rapporteur votre commission des affaires sociales a d'ailleurs souhaité durcir ce dispositif issu des travaux de l'Assemblée nationale afin de le rendre plus dissuasif. Nous y souscrivons pleinement. Mesdames et messieurs régulée, encadrée légiférer, c'est créer les conditions du développement des centres de santé de qualité pour nos concitoyens. Le gouvernement soutient ainsi pleinement les mesures de la présente, proposition de loi dont les dispositions nécessaires répondent à ses exigences. Elles nous permettront d'assurer un développement éthique des centres de santé au service d'un accès à des soins adaptés et de qualité pour chacun de nos concitoyens. Je vous remercie. merci madame la ministre et je vais. Tout de suite donner la parole à notre collègue Jean-Sol, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission. Mes chers collègues. En 2015, 3 ans seulement après son ouverture, les centres de santé Dentexia. Fermé après avoir mutilé. De nombreux patients. En septembre 2020, les centres dentaires l'Access fermé à leur tour. Créé en 2015 dans les Alpes Maritimes, ils avaient fait l'objet de nombreux signalements et de plusieurs inspections de l'Agence Régionale de Santé. À partir de 2016 et en mars 2018, une patiente de 75 ans était même décédés pendant une intervention. En 2021, éclater le scandale proxy dentaire du nom de cette chaîne bourguignonne de centres exploitant les mêmes recettes avec les mêmes résultats. Des patients attirés par la promesse de soins à bas coût des soignants sommé de faire du chiffre des soins superflus facturée en quantité excessive des victimes parfois édenté à vie. À chaque fois la même indifférence à la raison d'être de ces structures, de la part de ce qu'il faut bien appeler des aigrefins. Les profils des gérants mise en cause dans ce scandales était effet aussi éloigné qu'il est possible du monde sanitaire. De telles dérives ont été rendues possibles par un assouplissement du cadre juridique de ces centres qui a sans doute mal anticipé les failles dans lesquelles ne tarderaient pas à s'engouffrer des gérants peu scrupuleux. Afin de favoriser leur développement. La loi hôpital, patients, santé et territoires de 2009 avait ainsi notamment substituer au régime d'agrément. Un régime de simple déclaration de conformité à la réglementation. Une telle souplesse caractérisait également la nature juridique des centres la forme associative est assez recherché. Ainsi que les activités qu'ils peuvent entreprendre. Après le scandale Dentexia. L'ordonnance du 22 janvier 2018 avait cherché à mettre de l'ordre. Elle a interdit notamment dans ces centres et la distribution des bénéfices issus de leur exploitation. La publicité est rendue plus explicite le principe d'une ouverture à tous les patients et de la dispensation à titre principal. De De prestations remboursables. Ces mesures n'ont à l'évidence pas suffi. Certes la CNAM peut déjà que déconventionner. Les acteurs malhonnête, comme elle l'a fait opportunément le 22 janvier dernier de de centres francilien et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, a également mis fin au conventionnement d'office des centres de santé, mais cela ne résout pas le problème posé plus largement par segments de l'offre qui semble échapper en partie aux efforts de maîtrise. Le nombre de centres a bondi de 50% entre 2017 et 2021. Cette proportion. 124% pour les centres ophtalmologiques conduisant à une significative augmentation des remboursements liés à des consultations d'orthoptiste et le secteur se financiarisé, à l'instar du secteur des maisons de retraite. C'est assez dire si cette proposition de loi déposée par la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Fadila Khattabi et bienvenue. Il ne s'agit bien sûr pas de jeter l'opprobre sur tout le secteur car bien heureusement l'écrasante majorité des centres de santé fournit des soins de qualité mais de prévenir de prochains scandales rendue possible par les lacunes du quad résistant. Son article 1er rétabli un agrément pour les centres de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés. Il ne concernerait cependant que les seules activités dentaires et ophtalmologiques. Les autres activités des centres de santé demeure soumise au seul engagement de conformité dont le récépissé vaut autorisation de dispenser des soins. La demande d'agrément était d'examiner sur le fondement d'un dossier comprenant nécessairement les déclarations d'intérêts des membres de l'instance dirigeante. Ou encore les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces l'agrément pourra être refusée en cas d'insuffisance du dossier ou de manquements aux exigences du projet régional de santé. Un agrément provisoire délivrée pour une durée d'un an, pourra être remise en cause, suivant les résultats d'une éventuelle visite de conformité organisée par l'ARS. Enfin, comme souhaité par le rapporteur de l'Assemblée nationale l'agrément est délivré définitivement et maintenu sous réserve d'une transmission sans délai aux ARS et aux ordres concernés des contrats et diplôme des professionnels. La commission a clarifié la formulation de cet article, et notamment préciser les dispositions relatives au retrait de l'agrément provisoire comme définitif d'ailleurs particulièrement en cas de manquement aux règles applicables au Centre de santé ou relatives à la qualité et à la sécurité des soins. La commission a également souhaité renforcer les moyens d'information des ARS. Postérieurement en l'envoi de la demande d'agrément sur les Liens d'intérêts. Comme les contrats liant l'organisme gestionnaire. L'article 1er quater prévoit un mécanisme transitoire de gestion de stocks. Afin de faire entrer les centres de santé existant dans le nouveau régime d'autorisation. La commission a clarifié le dispositif transitoire car il est indispensable de contrôler aussi les centres existants. Elle a un outre aménager le délai prévu afin de mieux prendre en compte la charge de certaines ARS. L'Arctique le 1er bis prévoient l'exclusion du dirigeant d'un centre de santé de toute fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire si celui-ci a des Liens d'intérêt avec une entreprise délivrant des prestations à la structure. Il s'agit de prévenir certains montages complexes que l'IGAS avait identifié l'article 1er terre introduit une obligation d'information des ARS, des CPAM et ordres en cas de fermeture d'un centre de santé cet article répond là aussi à des dérives constatées d'utilisation frauduleuse de carte CPS et de facturation réalisé posteriori demain à des fermetures. La commission a approuvé ces 2 articles sous réserve de clarifications nécessaires. À ce 1er bloc d'articles relatifs à l'autorisation des activités de centres de santé et à la prévention de certaines dérives. La commission à outre adopté 2 articles additionnels. L'article 1er bis visant à assurer la continuité de la prise en charge des patients de centres de santé après une fermeture, il entend répondre aux situations constatées de passants mutilés dont les soins ne pouvait pas être repris par d'autres praticiens faute de dossiers médicaux suffisamment documenté. L'article 1er qu'Quiès renforce l'interdiction de publicité des centres de santé. L'article 2 obligent les centres à se doter d'un comité dentaires ou ophtalmologiques. Pour ceux qui exerce ses activités. Un tel comité qui sera chargé de contribuer à la politique d'amélioration de la qualité des soins et à la formation continue des salariés formera un utile contrepoids au pouvoir du gestionnaire. Il serait composé des seuls médecins du Centre. Mais pour être invités à ses réunions des représentants des usagers. L'article 2 propose. Également de faciliter l'identification par les patients. Des professionnels qui les prennent en charge. Les amendements adoptés par la commission à cet article vise à clarifier la rédaction de la loi et a renvoyé le détail au décret. L'article 2 bis. Dispose que les salariés des centres sont identifiés par un numéro personnel distincte de celui de la structure dans laquelle ils exercent. La commission a étendu cette mesure à tous les praticiens et non aux seuls salariés car les centres peuvent également faire appel à des bénévoles. L'article 4 vise à préciser les conséquences d'un constat de manquement à un centre de santé à ses obligations légales et réglementaires. Il garantit d'abord que les décisions de suspension et de fermeture prise par le directeur de l'ARS sont transmises sans délai à la CNAM et aux instances ordinales compétente il prévoit qu'une décision de suspension encore en vigueur ou une décision de fermeture peu pendant 8 ans, justifier le refus de délivrance du récépissé d'engagement de conformité. Ou de l'agrément demandé par le même organisme gestionnaire le même représentant légal ou un membre de son instance dirigeante. Il facilite en fait le recensement des mesures de suspension et de fermeture prise dans toute la France à l'attention des services de l'État et de l'assurance maladie. La commission a en outre rendu obligatoire la publication de telles mesures sur le site internet de l'ARS à l'initiative du groupe écologiste. L'article 5, dispose que les gestionnaires des centres de santé vont certifier leurs comptes et les transmettent annuellement au directeur général de l'Agence Régionale de Santé lorsqu'ils remplissent certains qui quittèrent qui seront fixées par voie réglementaire.

Enfin, complète et les dispositions relatives aux sanctions financières à la main du directeur général de l'ARS en élargissant les hypothèses dans lesquelles il peut les prononcer. En prévoyant un barème graduée qui serait précisé par voie réglementaire et en relevant la valeur de l'amende maximale et de l'astreinte journalière que la commission a de nouveau augmenté pour les porter respectivement à 500.000 et 5000 euros afin de rendre ce pouvoir de sanction plus dissuasif. Mes chers collègues, cette proposition de loi ne porte pas de vision nouvelle d'organisation de l'offre de soins de ville et nous pouvons le regretter. Elle est cependant indispensable. Nul n'en doute La commission sous réserve des derniers ajustements souhaitables espère que ce texte se trouvera au Sénat une rédaction permettant au bénéfice d'une navette constructive. Son adoption définitive au Palais Bourbon. Je vous remercie. Merci, merci monsieur le rapporteur. Et dans la suite de la discussion générale. La parole est maintenant à notre. Collègue Joël Guerriau pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre. Madame la présidente de la commission. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Une recherche rapide Internet sur le scandale Dentexia m'a conduit à avoir quelques photos choquantes. Témoignant du traumatisme qu'ont subis les victimes. En 2016, ce scandale explosa dans les médias et sera le début d'une longue série proxy dentaires dont excellence ou dans. Derrière ces noms se cacher en fait problème d'hygiène surfacturations et escroqueries mutilation. Ce sont ainsi plusieurs milliers de victimes qui ont malheureusement fait les frais. De ce centre dentaire dit low cost. Se soigner bien sûr pour moins cher. Pourquoi pas. Mais avec quelles conséquences. En 2009, le développement des centres de santé a été favorisée avec la suppression de l'obligation d'agréments nécessaires à leur ouverture par la loi du 21 juillet 2009. Remplacé par une simple déclaration de conformité. Cela répondait aux problèmes observés selon lequel beaucoup de Français, soit se rendaient à l'étranger pour payer moins cher leurs soins dentaires avec les risques que cela comportait soit il renonce hein tout simplement quelques années et de nombreuses victimes plus tard. Nous devons aujourd'hui revenir sur la législation applicable à ces centres d'autant plus que les dérives constatées ne concerne évidemment pas tous les centres, les 100 de santé présente l'Avantage de pouvoir délivrer des soins médicaux ou paramédicaux, ils peuvent regrouper des médecins généralistes, des spécialistes des kinésithérapeutes et caetera. Il permet ainsi aux patients l'accès à plusieurs professionnels de santé au même endroit et ce à des conditions tarifaires abordables. Du côté des professionnels de santé qui exercent les centres de santé leur offrent des conditions d'exercice intéressante avec la possibilité du salariat. L'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les congés payés, le bénéfice de l'interdisciplinarité la mutualisation d'investissement et de tâches administratives, de quoi finalement, satisfaire des aspirations nouvelles de et tout à fait. Compréhensible. Les dérives de quelques-uns ne doivent pas entacher l'exemplarité des autres au delà d'une réponse uniquement judiciaire une prise en compte. Législatives s'impose. La PPL illustre justement cette prise en compte et a pour objet de renforcer davantage les conditions d'ouverture et les contrôles internes des centres de santé exerçant une activité dentaires ou ophtalmologiques. Non seulement elle vise à rétablir l'obligation d'agrément supprimé en 2009 mais en plus elle propose de ne délivrer qu'un agrément provisoire soumis à une visite de conformité dont on peut néanmoins regretter le caractère facultatif et à la transmission de diverses pièces telles que les contrats de travail et les diplômes professionnels. Elle vise également à prévenir les conflits d'intérêts, mieux encadrer les situations de fermeture des centres instaurer un comité médical chargé de l'amélioration continue de la qualité de la sécurité des soins imposé la transmission des comptes annuels à l'ARS. Autant de mesures qui viendront assurément encadrer plus strictement l'activité de ces centres et surtout sécuriser la prise en charge des patients afin qu'a lieu de soin de devienne jamais à un endroit dans lequel on se fait voler ou mutilés. Toutefois, afin que l'objectif visé par cette PPL soit atteint. Il faudra que les ARS dispose des moyens nécessaires pour effectuer les contrôles Haddock. Sans cette capacité la portée de ce texte ne sera malheureusement que symbolique. Au delà de ce qu'elle propose cette PPL nous rappelle qu'en toute situation, le manque de contrôle favorise des dérives. Elle nous rappelle aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'à vouloir parfois trop simplifier la réglementation pour fluidifier d'accès aux soins des patients, on les expose en réalité à d'autres risques. Enfin elle nous invite tous à toujours mesurer l'impact des décisions que nous prenons afin que les patients ne soit jamais victime ni de charlatan, ni de mauvaises décisions politiques, et bien sûr pour toutes ces raisons le groupe les indépendants votera en faveur de ce texte. Merci de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Raymonde Poncet moche pour le groupe écologiste pour cinq minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues. Pratique commerciale trompeuse surfacturation manquent pas hein l'hygiène opacité concernant les employés dilution des responsabilités. Après l'affaire des Ehpad Orpea ce terrible. Constat vice-donc des centres dentaires. Ces dernières années des scandales sanitaires ont mis en lumière des pratiques de sur prescription de soins et de. Fraude à la sécurité sociale dans le but là aussi de réaliser d'énormes bénéfices ceci est de nouveau l'histoire de la rencontre entre la lucrative IT et la santé. Rencontre qui impacte plus durement les plus pauvres. Rappelons l'existence d'une prévalence entre la gravité des pathologies bucco-dentaire et le statut socio-économique et la persistance hein. Si de fortes inégalités de santé bucco-dentaire. D'après une enquête en 2000 Ducret DES selon la catégorie socio-professionnelle, le pourcentage d'adultes ayant des dents manquantes non remplacés varie du simple au double, 45% des ouvriers non qualifiés sont concernés, parmi les causes. Parmi les causes. Une des causes et le coût des soins dentaires pour des personnes aux revenus modestes et ou qui ne possèdent pas de complémentaire santé. Les études dont une de lire d'sur le renoncement aux soins démontre. Que pour des raisons financières. Les soins dentaires sont sacrifiés en 1er suivi des soins ophtalmologiques, c'est pourquoi l'offre de soins de certains centres de santé dits à bas prix est devenue attractive pour ces publics. Pourtant la lucrative IT est antinomique avec le modèle des centres de santé. Qui s'inscrit dans un projet collectif dont une des prairies des priorités justement de favoriser l'accessibilité financière aux soins de santé primaires et souvent aux spécialistes, limitant ainsi le renoncement aux soins. Les centres de santé demeurent des piliers de l'accès aux soins et de la lutte contre les déserts médicaux. Il n'est donc pas question de les amalgamer avec ces pratiques délétères. La majorité notamment les Centres mutualistes ou gérés par les caisses d'assurance maladie ou par les collectivités territoriales. Joue un rôle médico-social essentiel en France. D'autant que des surfaces surfacturation peuvent aussi exister dans le cadre d'une pratique libérale. Il s'agit donc, comme l'indiquait le rapport de l'IGAS de 2017 de mettre en place des garde-fous législatifs et réglementaires pour prévenir une gestion à but lucratif des centres de santé. Cependant, certaines mesures. Comprises dans le texte sans doublonner des dispositions légales et conventionnelles existants. De plus c'est prévu bien le rétablissement d'un agrément par l'ARS qui avait été supprimé, faute de moyens humains à l'ARS et en raison du frein, qu'il a constituée au développement des centres de santé. Dans le rapport précité. L'IGAS estime qu'il vaut mieux mobiliser les ressources humaines, des pouvoirs publics sur des contrôles ciblés. Car cet agrément coûteux en moyens n'aurait, je cite toujours l'IGAS. Qu'un impact limité sur l'ouverture de centres s'inscrivant dans une logique lucrative. Les moyens humains d'inspection, contrôle de l'État ainsi que ceux des organismes d'assurance maladie se sont raréfiés au fil des années. Nous appelons certes. À leur augmentation mais partageons l'appréciation qui sont plutôt dévolu et efficace au contrôle notamment inopiné. Nous regrettons que les maisons de santé pluridisciplinaires d'ailleurs soient exemptées des dispositions du texte créant une inégalité entre structures de soins coordonnés. Malgré tout, nous notons que cette proposition de loi contient des mesures importantes. Elle permet une meilleure traçabilité des actes un renforcement des sanctions financières. La création d'un répertoire national des mesures de suspension et de fermeture. Ainsi que la facilitation de l'identification des professionnels. Le texte prévoit également un renforcement du suivi des comptes de gestionnaires et des pratiques de facturation et entendu tu es contre les conflits d'intérêts. À l'origine des montages financiers. Nous saluons l'adoption en commission de notre amendement qui, par souci de transparence rend obligatoire la publication de la sanction financière prononcée à l'encontre d'un centre frauduleux sur le site de l'ARS. In. Nous soutenons le modèle des centres de santé dont la forme associative a été dans le passé. Parfois détournés dans un but lucratif afin de contrer ces pratiques frauduleuses et malgré les réserves que j'ai formulé le groupe écologiste solidarité et territoires votera pour cette proposition de loi, je vous remercie.

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi présentée aujourd'hui dans notre hémicycle est particulièrement attendue et nécessaire. Elle est attendue par nos concitoyens qui souhaitent accéder à des soins de qualité, abordable et pratiqué dans de bonnes conditions. Elle est aussi largement soutenu par les acteurs de la santé, je pense aux ARS à la CNAM à la Fédération nationale des centres de santé aux ordres et syndicats des professionnels de santé et bien évidemment aux associations de victimes. Elle est enfin nécessaire car 13 ans après le vote de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Nous avons constaté que le cadre juridique des centres de santé existants n'avait pas empêché de nombreux scandales sanitaires au sein de ces derniers. En remplaçant le régime d'agrément par un gym de sample déclaration de conformité à la réglementation. Certains centres de santé se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont profité de la souplesse, permise par la forme associative des centres de santé pour en faire des entreprises purement lucratives. En 2015, le scandale dans Dexia et en 2021, le scandale proxy dentaires ont révélé les pratiques d'une extrême gravité pour de nombreux patients. Je parlais précédemment des dérives lucrative auxquelles j'ajouterai des escroqueries aux patients et les fraudes à l'assurance maladie. Mais il faut souligner, mes chers collègues, la question des soins de leur pertinence de leur qualité et les conditions dans lesquelles ils sont exercées, à titre d'exemple, le scandale dans Dexia ce n'est pas moins de 2400 victimes et 350 plaintes. Qui ont été réalisées avec toujours la même méthode des tarifs au départ très attractif des soignants à qui l'on demande de faire du chiffre des soins réalisés à la va-vite et dangereux et au final des victimes trop nombreuses qui souvent se sont endettés pour des traitements dentaires marraine mal réalisé est pas terminé. Ces dérives ne sont évidemment pas la norme et une majorité des centres de santé, je pense notamment au centre mutualiste ou encore au centres municipaux continuent de jouer un rôle majeur et et remplissent parfaitement leur mission. Pour autant ces cas nous oblige, pour la sécurité des patients et pour ne pas jeter l'opprobe sur tout le secteur qui protège qui soigne et qui est au coeur de notre système de santé. Il nous faut donc pallier les limites. Dont. Ces quelques acteurs profitent attirés par l'intérêt lucratif. Il existait un réel besoin de légiférer sur le sujet. Je me félicite que nous puissions débattre aujourd'hui de ce texte et de ces avancées majeures. Je tiens d'ailleurs à saluer les parlementaires à l'initiative de cette proposition de loi et tout particulièrement la présidente Khattabi pour son travail et son agacement sur le sujet, je profite d'ailleurs de cette occasion pour lui donner au nom de notre groupe toute notre solidarité concernant les attaques qu'elle a été dont elle a été victime. Il s'agit ici d'aller donc, plus loin dans le contrôle des comptes des centres de santé. Je tiens également à souligner le travail de le rapporteur qui a renforcé avec justesse plusieurs dispositions de ce texte. Il était indispensable de durcir les conditions d'ouverture des centres de santé notamment rétablissement l'agrément préalable nécessaire et valant autorisation à dispenser des soins au même titre que le renforcement de refus et le retrait de l'agrément. D'autre part, le renforcement des mesures de contrôle et les moyens donnés aux ARS doivent être conséquent. Il s'agit de pour vous de pouvoir contrôler en amont de l'ouverture du Centre d'éventuels contrevenants s'à une gestion saine de ces centres. Par ailleurs, comme indiqué dans le rapport de la commission, je me félicite que l'agrément comme son maintien sont conditionnés soit conditionné à la transmission des diplômes et contrat de travail. Quant aux ARS qu'aux heures d'autres compétent. C'est une avancée en la matière comme d'autres moyens de contrôle présenté dans ce texte qui vont dans le bon sens.

Trop de victimes qui Dark qui garderont des séquelles trop de patients arnaquer. Pour éviter les dérives pour assurer des soins de qualité. Il nous faut donc mes chers collègues, revenir à un encadrement plus strict réguler mais aussi mieux contrôler l'accès égal à des soins de qualité n'est pas négociable. C'est pourquoi, chers collègues, le groupe RDPI soutient avec force cette proposition de loi. Ce texte est l'aboutissement d'un travail collectif pour répondre aux attentes des Françaises et des Français en la matière de santé. Je vous remercie. merci, cher collègue. Et puis je passe maintenant la parole à d'autres collègues Anne Le Huérou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues l'émergence et le développement des centres de santé a considérablement modifié l'accès aux soins et la pratique de la médecine de ville dans notre pays. Ces structures sanitaires, publiques et privées dispense des soins de 1er et second recours. Ils sont indispensables pour répondre à l'organisation au besoin de soins dans notre territoire. Toutefois différents scandales tels que celui de de Dentexia et plus récemment celui de proxy dentaires ont révélé les dérives d'ampleur de certains de ces centres. Nous ne pouvons tolérer que des patients ne soit pas correctement pris en charge, soient mutilés encore escroqués par des charlatans qui n'ont pas d'autres objectifs que le profit et qui n'ont rien à faire dans notre système de santé. La proposition de loi visant à encadrer les centres de santé que nous examinons aujourd'hui était nécessaire, il n'est pas acceptable que dans, dans notre pays au regard du système de soins qui est le nôtre de telles dérives puisse encore avoir lieu. Il en va de la sécurité sanitaire et de la garantie de pérennité de notre système de sécurité sociale. Il s'agit d'éviter les abus et fraudes recensées par l'assurance maladie en luttant plus sévèrement contre l'exercice illégal de la profession les surfacturations et autres sur traitement. Cette proposition de loi s'ajoute à une succession de proposition de loi visant à mettre un bout de sparadrap sur un système de santé à bout de souffle dont une remise à plat globale est aujourd'hui nécessaire. Les soins ne sont pas des produits de consommation. Le service public doit garantir la pertinence des soins et la qualité des soins à tout citoyen de notre pays. Les centres de santé sans médecin physiquement présents se multiplient dans mon département des Côtes d'Armor, un centre ophtalmo a ouvert ses portes en 2021. Sur place aucun ophtalmologue présent des assistants réalise des examens Post de diagnostic à distance sans entrer en contact avec le patient. Ces pratiques profite de la situation de pénurie des professionnels de santé elle déshumanise progressivement notre système de santé. La confiance entre le personnel médical et les patients se détériore. Face à ces dérives un encadrement s'impose. Le texte vient renforcer les contrôles de ce centre en rétablissant l'agrément délivré par l'autorité administrative autorisant l'exercice de l'activité dentaires et ophtalmologiques. D'autre part afin d'éviter que les gestionnaires sanctionné sur le plan ordinale ou pénale puisse pratiquer du nomadisme en passant d'une région à une autre. Le texte propose également la création d'un répertoire national des gestionnaires sanctionné. L'article 3 de la proposition de loi instaure l'obligation pour le gestionnaire de transmettre à l'ARS. Les copies des contrats de travail et les diplômes des chirurgiens dentistes. Enfin, le texte prévoit la possibilité pour le directeur général de l'ARS de refuser un gestionnaire, l'ouverture d'un nouveau centre lorsque l'un de ces centres fait déjà l'objet d'une procédure de suspension de fermeture, le renforcement des contrôles permettra de lutter contre les dérives et garantira à nos concitoyens la qualité des soins dispensés pour être efficace, ce renforcement doit être accompagnée d'une augmentation des moyens attribués aux ARS pour mener à bien leur mission de contrôle et d'instruction des dossiers à l'heure actuelle, elle ne dispose pas des moyens humains ni matériels nécessaires pour le faire. Se pose également la question du caractère lucratif de ces centres en 2018 le gouvernement a par ordonnances permis aux personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé à but lucratif de créer et de gérer les centres de santé, ce n'est pas notre conception de l'organisation des soins jusqu'alors uniquement réservé aux organismes à but non lucratif, aux collectivités territoriales aux établissements publics et encore aux établissements publics de santé dénaturant ainsi des centres de santé cette mesure sert la marchandisation de la santé et organise la concurrence entre des grands groupes privés et d'autres acteurs dans le domaine de l'offre dense Nous nous opposons à la financiarisation de la santé le 1er recours et les structures commerciales, à but lucratif. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la le choix d'appliquer de nouvelles mesures d'encadrement aux seuls centres dentaires et ophtalmologiques ça sent qu'il y a d'autres centres de en psychiatrie ou gynécologie par exemple qui se développe contre cette dégradation de l'offre de soins, nous avons proposé un amendement fixant un ratio d'assistants dentaires ou médicaux par rapport au dentiste ou after ou ophtalmologiste présents dans un centre. Ce ratio a pour objectif de garantir les conditions d'une prise en charge adéquate des patients et la qualité des soins. Ce texte encadre les dérives trop souvent constaté et comme en commission. Notre groupe socialiste, écologiste et républicain soutiendra cette proposition de loi et nous nous interrogeons néanmoins sur. La question des moyens nécessaires à l'ARS pour mener à bien sa mission et le contrôle de ces centres de santé. Merci. Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord remercier le rapporteur Jean-Sol pour la qualité de son travail. Vous connaissez l'attachement de mon groupe au centre de santé pour nous ces structures constituent une réponse essentielle dans l'accès aux soins, établissements de proximité implantés historiquement dans des villes et quartiers populaires qui se sont développées ces 10 dernières années dans des zones rurales dispensant des soins de qualité sans dépassement d'honoraires avec une pratique généralisée du tiers payant, et surtout structures collectives permettant un exercice médical et paramédical salariés plus attractif pour les jeunes professionnels aujourd'hui nous en sommes profondément les défenseurs à l'heure où la santé et de plus en plus considérée comme une marchandise, ouvrant des perspectives de profits juteux certains centres de santé sont pourtant ébranlé depuis quelques années par des scandales sanitaires et il me paraît ici essentiel de préciser d'emblée qu'il y a en réalité 2 catégories bien distinctes de centres de santé d'un côté les centres de santé publics municipaux mutualiste, associatif, à but non lucratif où le patient est réellement au coeur de la prise en charge et de l'eau, des structures qui ont de centres de santé que le nom à vocation lucrative financière ou le ce qu'on est en réalité loin des préoccupations cette seconde catégorie que l'on pourrait renommer les marchands d'actes ont pu s'implanter ces dernières années du fait de la loi HPST et de la suppression du régime d'agréments préalables pour ouvrir de telles structures, contre l'avis des organisations syndicales, professionnelles, ces centres locaux spécifiquement dentaires et ophtalmologiques détenus par des holdings faisant remonter leurs bénéfices dans des structures commerciales à but lucratif se sont multipliées fortement selon la CNAM, la patiente elle de ces centres a doublé de 2015 à 2019 passant de 400.000 à 800.000 patients. En 4 ans alors que le coût des remboursements pour leurs actes a bondi de 245% pour atteindre 69 millions d'euros parallèlement à cet assouplissement et cette croissance exponentielle ne le nombre de contrôles, faute de moyens de des ARS a diminué, ce qui était malheureusement prévisible arriva avec les affaires donc en 2015 et proxy dentaire en 2021. Comment ne pas être en colère et profondément choqué de voir des patients mutilés de trop nombreuses victimes de ces sentent low cost ne peuvent même pas recourir à des soins de qualité réparateur faute de reconnaissance réelle et d'indemnisation de la part des autorités. À quand un procès pénal pour dénoncer ces escroqueries qui ont ruiné la vie de ces hommes et de ces femmes. Comment ne pas être en colère alors que malgré les recommandations de l'IGAS en 2016 et 2017. Rien n'a été fait et que les dérives ont pu continuer cette PPL et donc la bienvenue, mais sera-t-elle suffisante et efficace. Nous avons quelques doutes rétablir un agrément pour les centres ayant une activité dentaires ou ophtalmologiques activités pour lesquelles les dérives sont les plus fréquentes, est une bonne chose. De même, la transmission des copies des diplômes et contrats de travail des chirurgiens dentistes assistant ophtalmologistes et orthoptistes peut contribuer à plus de transparence et d'exigence. Mais nous sommes très perplexe sur l'efficacité de ces contrôles et de cet encadrement par les directeurs des ARS puisqu'aucun moyen supplémentaire ne va leur être accordé pour ses nouvelles missions. De même, nous regrettons que la rédaction laisse la possibilité pour les centres d'Évian de poursuivent leurs activités, même en cas de manquement à la qualité ou à la sécurité des soins. Il aurait fallu adopter un caractère automatique à la fermeture comme d'ailleurs aux sanctions financières infligées même si nous saluons leur réévaluation par notre rapporteur le directeur d'une ARS sera toujours la possibilité de ne pas. Prononcer d'amende. Nous aurions souhaité plus d'exigence et de fermeté à tous ces niveaux pour rendre le dispositif réellement dissuasif. Soyons lucides, mes chers collègues, nous sommes face ici à des prédateurs qui ont une grosse capacité de contourner la loi si celle-ci n'est pas suffisamment encadrante nous leur laisserons les mains quasi libre nous aurions même mais que cette PPL aille plus loin et supprime la possibilité d'ouvrir des centres de santé pour des gestionnaires à but lucratif je sera d'ailleurs l'objet d'un de nos amendements. Il faut en finir avec les structures privées lucratives, qui voit la carte vitale comme une carte bleue, cela étant nous prenons cette PPL comme une petite avancée, une première étape nous la voterons donc en souhaitant qu'il y a une prochaine loi plus général sur les centres de santé afin d'encourager le développement des centres vertueux et des bien davantage les collectivités qui souhaitent avoir recours à ces structures n'oublions pas mes chers collègues et Madame la Ministre que c'est un des moyens de faire reculer les déserts médicaux. Je vous remercie. Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à Olivier Henno. Pour le groupe Union centriste pour huit minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Je souhaite d'abord saluer votre excellent travail. Monsieur le rapporteur sénateur Jean-Sol qui aura permis de soulever les grandes problématiques de notre système d'encadrement de centres de santé. La révélation de scandales, ça a été dit comme Orpea où certains centres dentaires ou ophtalmologiques a confirmé nos inquiétudes aujourd'hui le constat est simple, il y a urgence à renforcer l'encadrement de nos centres de santé pour lutter contre ces carences et ses abus, c'est d'ailleurs un constat partagé par tous les acteurs auditionnés ces dernières semaines en en commission en 2009 la suppression de l'agrément préalable et la souplesse du cadre juridique permise par la forme associative pour détourner le modèle de santé sont à l'origine de ces dérives. Le résultat est accablant, ça a été dit patients mutilés de multiples fraudes à l'assurance maladie. Je n'ai donc aucun doute sur le bien-fondé de cette PPL mais mes chers collègues. Madame la Ministre je veux profiter de cette discussion parlementaire pour aborder d'autant plus que j'ai 8 minutes, une question qui me tient à coeur, la perte de sens de légiférer à tour de bras sur le système de santé. Un petit bout par ci, un petit bout par là. Pour preuve, nous débattrons tout à l'heure d'une autre PPL et pas des moindres. La PPL Rist. Mes chers collègues, je vous faire partager une citation d'Euripide. Les amateurs de théâtre se reconnaîtront. Ce n'est pas l'abondance. Mais l'excellence qui est richesse Ma conviction c'est que la multiplication des initiatives législatives gouvernementale souvent parlementaires parfois participent davantage à stresser le système de santé qu'à l'améliorer. C'est d'une grande loi santé dont nous avons besoin, ni plus ni moins. Pour faire écho à l'exaspération, légitime d'ailleurs on le voit aujourd'hui des soignants et des médecins. Je veux faire mienne la citation du président Pompidou arrêtons dans ce pays d'emmerder les soignants et les médecins. Une autre priorité doit être de former plus de médecins car tous ces problèmes résultent en bonne partie de la pénurie. Or, monsieur le ministre de la Santé sur ces bancs ici même lors des discussions sur le PLFSS du mois de novembre avait reconnu que malgré le déblocage du numerus clausus nous ne formions quand en France que 10 pour 7% de plus de médecin parce que pas assez de locaux, pas assez de professeur de médecine autant de mauvaises raisons, autant de blocages et de freins malheureusement spécifique à notre pays la France. Résultat, beaucoup de Français, de jeunes Français se forme en Roumanie ou ailleurs absurde ubuesque. J'en viens au fond de cette. Proposition de loi. Je dois reconnaître ma satisfaction de sa d'Arte sur un fléau qui touche concrètement le quotidien de plusieurs de nos concitoyens car l'ordonnance du 22 janvier 2018 prise après le Skandia le. Dentexia a certes précisé un peu le droit mais cela n'a visiblement pas été suffisant. Ce texte contient de réelles avancées. Le rétablissement de l'agrément délivré par le directeur de l'ARS, l'obligation pour le gestionnaire de transmettre les contrats de travail des praticiens de l'ARS, l'obligation pour l'ARS de communiquer ces contrats de travail aux ordres. L'article 2 obligent les centres à se doter d'un comité dentaires ou ophtalmologiques pour ceux qui exerce ses activités un tel comité serait chargé de contribuer à la politique d'amélioration de la qualité des soins et à la formation continue des salariés, c'est une bonne mesure attendue des patients qui ont vécu de vrais traumatismes des chirurgiens dentistes, pour qui les excès de certains cabinets dentaires ont tâché l'image d'une profession qui ne le méritait pas attendu au également par l'assurance maladie, victime de nombreuses fraudes. Cette proposition de loi doit être appliquée, rapidement. Mais rappelons-le, ça a été dit, mes chers collègues, dans leur grande majorité, les centres de santé, qu'ils soient communaux mutualiste ou associatif à but non lucratif effectue un travail de qualité. Les brebis galeuses n'attachent pas la probité de la totalité du troupeau. Parlons des brebis galeuses de Dentexia de proxy dentaire qui a mis en lumière le fonctionnement de certains centres de santé dentaires ou la qualité et la sécurité n'était clairement pas une priorité. Preuve que la lutte contre ces centres de santé dit low cost est indispensable. Voyez ce débat me rappelle le cours d'économie sur les effets de la surconcentration en effet nous sommes soumis dans le domaine de la santé des soins des difficultés autrefois inconnus cette surconcentration se caractérise par la parution d'acteurs financiers en recherche de rentabilité record qui ne sert ni les patients ni les soignants ni l'aménagement du territoire. C'est vrai pour les maisons de retraite, c'est vrai pour les soins dentaires, ophtalmologiques pour les laboratoires, voire même sur un autre sujet pour les biotechs. C'est le mérite de cette PPL de s'attaquer à cette surconcentration je tiens de. Je tiens à saluer de mesures dans son texte. Premièrement, l'introduction d'une obligation pour le représentant légal de l'organisme gestionnaire d'informer dans les 7 jours, le directeur général de l'ARS, le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental de l'Ordre compétent en cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ces centaines, une telle faire mesure viendra apporter une réponse à la problématique des cartes de professionnels de santé qui continue à circuler sans contrôle alors que les centres de santé dans lesquels exercer les professionnels de santé avait fermé. Deuxièmement, l'obligation pour les professionnels de santé, salariés d'un centre de santé d'être identifié par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure de leur activité. Une telle traçabilité est une exigence morale. Au delà des scandales médiatiques, le développement de ces centres à bas prix a largement participé aux abus et fraudes recensées recensées par l'assurance maladie. Il s'agit donc aujourd'hui de lutter plus sévèrement contre cette forme d'exercice illégal de la médecine. J'ajoute. Un autre effet pervers de cette. Sur-concentration. La fermeture de certains laboratoires qui transforme encore un peu plus la ruralité en désert médical. Cette question est d'autant plus préoccupante que les centres de santé. Ça a été dit, je ne sont souvent fréquenté par des publics vulnérables disposant de de peu de moyens. Voilà, mes chers collègues. Parce que la qualité des soins n'est pas négociable. Parce que toute fraude doit être lourdement. Notre groupe votera en faveur de cette PPL je vous remercie. Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à Véronique Guillotin pour le groupe RDSE. Pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de commission. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il n'est effectivement pas possible de transiger avec la qualité des soins et la sécurité des patients. Si en 2009, le législateur a considérablement assoupli la procédure préalable à l'ouverture des centres de santé c'était avant tout ça a été dit pour améliorer l'accès à des soins de meilleure qualité aux plus démunis en particulier dans les zones sous-dotées. Ces centres présenter une alternative à l'offre libérale dans un contexte de fortes inégalités dans l'accès aux soins dentaires, avec des prestations principalement remboursé par l'assurance maladie. Le tiers payant et l'absence de dépassement d'honoraires aussi face à des devis de libéraux qui dépassait les capacités financières de certains patients. Ils se sont tournés vers des centres de santé dentaires d'un nouveau genre plutôt que de renoncer aux soins ou partir se faire soigner à l'étranger, ils l'ont fait en toute confiance. Mais alors que l'ouverture de ces centres étaient limité à une déclaration avec dépôt d'un projet de santé d'un règlement intérieur les pouvoirs publics n'ont pas renforcé leurs systèmes de vigilance ni les contrôles pour s'assurer que la sécurité et la qualité des soins, été garantie comme le relève le rapport de l'IGAS de janvier 2017. Il n'en fallait pas plus pour que des gestionnaires peu scrupule et sont peu scrupuleux s'engouffre dans la brèche, faisant des milliers de victimes mutilées et endetté actes de soins fictifs ou inappropriés infection due à un manque d'hygiène surfacturation des infractions multiples qui ont laissé des patients désemparés, confronté à des abandons de soins et dans l'impossibilité financière de les poursuivre pour que des scandales tels que Dentexia et proxy dentaires ne puisse plus se reproduire. Il est indispensable de renforcer les règles et les procédures de contrôle. Les associations de victimes attendent cela depuis longtemps. Mettre un terme aux dérives sans entraver le développement et le fonctionnement des centres de santé vertueux, telle est l'objectif de cette proposition de loi à laquelle le groupe RDSE souscrit pleinement je salue bien sûr le rétablissement de l'agrément préalable, les travaux de réécriture de l'article premier tant au niveau de l'Assemblée nationale que de notre commission ont amélioré le dispositif et renforcer le pouvoir des ARS. C'est une très bonne chose, je me félicite notamment de la transmission de la déclaration des Liens et des conflits d'intérêts, ce qui évitera que des sociétés privées en lien avec les centres dentaires serve de canaux pour faire sortir l'argent de l'association à but non lucratif. Mais cela nécessitera certainement, d'augmenter significativement les moyens alloués aux ARS pour leur permettre d'affecter du personnel à la surveillance de ces centres de santé. Nous saluons également l'interdiction faite à toute personne de diriger un centre de santé dès lors qu'elle a des Liens d'Inde serré avec une entreprise délivrant des prestations à la structure gestionnaire jusqu'à présent le président d'une association pouvait par exemple exercer cette fonction à titre bénévole et être en même temps rémunéré par une société dont l'association était la seule cliente donc de fait par l'argent provenant de l'association dont il était président. J'espère que vous m'avez suivie. 5 des 7 centres dentaires associative visé par la mission de l'IGAS en 2017. Fonctionner de la sorte, c'était un moyen de contourner la gestion désintéressée et l'obligation de n'avoir aucun intérêt direct dans les résultats de l'exploitation. L'article 1er bis permet notamment de mieux cibler les dérives observées et de les contrer. De la même façon interdire le paiement anticipé intégrale des soins qui n'ont pas encore été dispensé est une très bonne chose, cette pratique qui a pu être observée s'accompagnait, parfois même d'offres de crédit avec de terribles conséquences sur ce que les soins était de mauvaise qualité ou qu'il n'est pas qu'il n'était pas tout simplement effectué enfin ce texte renforce le pouvoir de sanction des ARS et empêchera ainsi qu'un gestionnaire fautif contourne les sanctions et puis s'ouvrir une nouvelle structure de soins Madame la Ministre vous l'aurez compris, le groupe RDSE soutiendra cette proposition de loi. Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à notre collègue Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. J'attends donc aujourd'hui l'examen en séance publique de la proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé ce texte résulte d'un double constat l'augmentation exponentielle et rapide du nombre de centres de santé et malheureusement l'augmentation du nombre de dérives constatées. Alors je tiens à le rappeler. Ne s'agit pas là d'un procès intenté à l'encontre des centres de santé le modèle des centres de santé a permis de résoudre un certain nombre de difficultés en matière d'accès aux soins et de façon qualitative. Même si on ne peut que regretter leur forte concentration dans l'écran 100 turbin. Mais les pratiques frauduleuses. Même si elle ne concerne qu'une minorité de ces structures sont intolérables. Et inacceptables. Ce texte se focalise sur les activités dentaires et ophtalmologiques qui demeure majoritaire comme cela a été rappelé le scandale Dentexia a permis de mettre en lumière des pratiques frauduleuses et dangereuses qui nuisent à l'image de ce type de structure. Les dérives constatées et cela a été dit se situe à différents niveaux. Non respect du code de travail fraude à l'assurance maladie, fraude fiscale ou encore et surtout, mise en danger de la sécurité du patient. Ces dérives sont inacceptables et intolérables au regard de la gravité des faits et de l'éthique qui doit normalement prévaloir dans l'univers de la santé ainsi elle fragilise la confiance des patients qui deviennent des victimes et sont une entorse au pacte républicain. La majorité sénatoriale intervient régulièrement sur les questions de fraude à l'assurance maladie et réalisé par des patients, nous devons également être intransigeant lorsque les auteurs sont des professionnels de santé. Les professionnels de santé auditionné dans le cas de cette proposition de loi sont favorables aux mesures contenues dans ce texte en effet ces scandales à répétition ont un impact désastreux sur la confiance accordée à certaines professions à une époque, je le rappelle ou le fait scientifique est régulièrement remise en cause. C'est également à saluer la réintroduction bienvenue d'un agrément nécessaire avant d'ouvrir un centre de santé, cette disposition avait été supprimé par la loi de 2009, afin d'éviter aux professionnels de santé le capharnaüm administratif trop souvent présents dans notre pays. 14 ans plus tard, nous pouvons constater que cette mesure de bon sens et de simplification administrative a eu des effets désastreux pour certains patients à cause de personnes mal intentionnées qui ont vu dans les centres de santé, une manne financière sponsorisés par les Français. C'est pourquoi je souhaiterais que, dans les textes à venir nous soyons particulièrement vigilants sur les questions de simplification afin de ne pas ouvrir une nouvelle boîte de Pandore aux escrocs en tout genre. Afin de compléter ce texte déjà bien aboutie après son passage en commission et j'en profite pour saluer l'excellent travail du rapporteur Jean Sol. J'ai déposé un amendement visant à introduire un ratio de 1 pour 1 dans les centres de santé ophtalmologique ratio entre le nombre d'assistants médicaux, et le nombre de médecins. Ainsi cette limitation serait un garde-fou utile pour éviter des dérives dans des centres de santé peu scrupuleux cet encadrement étaient présents dans la proposition de loi sur l'amélioration de l'accès aux soins dont nous débattrons en fin d'après-midi il me semble plus cohérent de le réintroduire dans cette proposition de loi. Vous l'aurez compris, mes chers collègues. Ce texte est relativement consensuel et ne devrait pas rencontrer d'opposition frontale dans cet hémicycle. Notre rôle au Sénat sera de veiller à la bonne application de ces dispositions et de pouvoir prochainement en mesurer les effets. Notre système de santé en sera grandit pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi nécessaire et bienvenu. Je vous remercie. Merci cher collègue et la parole est maintenant à notre collègue Jean-Luc Fichet, du groupe socialiste. Pour 4 minutes. Monsieur le président. Madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Nous siégeons aujourd'hui pour examiner la proposition de loi d'encadrement de centres de santé dentaires et ophtalmique suite à une multiplication de scandales affectant très douloureusement les patients concernés. Ces scandales illustre parfaitement certaines dérives qui affectent notre système de santé. Force est de constater que les centres de santé non pas essaimé sur l'ensemble du territoire mais se sont concentrés dans des zones urbaines déjà surdotées. C'est particulièrement le cas pour les centres de santé visés par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui.

Se sentent ne participe clairement pas au rééquilibrage de l'offre de soins. Qu'une non prise en compte des besoins des populations en fonction des territoires. C'est pourquoi le groupe des sénateurs socialistes, écologistes et républicain proposera un amendement à cette PPL tendant à remédier à cet état de fait il faut clairement ne plus autoriser l'implantation de nouveau Centre dans des zones géographiques où ceux-ci se concentre déjà. Notre groupe entend ainsi lutter contre les dérives nées de la recherche de la maximisation des profits. Cette proposition de loi d'encadrement des Centres de santé propose certaines dispositions qui vont dans le bon sens comme l'agrément nécessaire et autorisation pour les centres de santé et dispenser des soins cet agrément qui est délivré par le directeur général de l'ARS avait été supprimé par la loi hôpital, patients, santé et territoires de 2009 dans l'espoir de multiplier les installations sur l'ensemble du territoire français comme moyen de lutte contre la désertification médicale. Notre groupe entend faire des propositions. Pour améliorer le dispositif. De l'agrément telle que prévue par la proposition de loi en effet. Le contrôle sur pièces est insuffisant pour se prémunir des dérives et scandales sanitaires des centres de santé hein, structure commerciale utilisés comme des machines à profit. Nous proposerons donc l'agrément définitif soit soumis à une visite de conformité par l'ARS. Cette disposition permettrait à la fois de tirer les leçons de scandales dentaire et de se prémunir d'un futur scandale de type Orpea dans le secteur des soins des premiers secours comme je le disais, cette proposition de loi contient certaines dispositions bienvenue mais elle ne lutte absolument pas contre la véritables fléaux de la financiarisation de notre système. Malheureusement, la politique de santé menée depuis 2017 accroît un con c'est incontestablement cette financiarisation. Pour tenter d'y mettre un coup d'arrêt, nous proposerons par voie d'amendement. De soumettre tous les centres de santé agrément. La réintroduction de cet agrément a fortiori. Pour tous les centres de santé avec visite de conformité comme nous le proposons nécessite une augmentation des moyens des agences régionales de santé pour rendre effectif ce que la représentation nationale vote. C'est là votre responsabilité politique, Monsieur le Ministre. Il en va de la sécurité et de la santé de nos concitoyens. Je me réjouis des dispositions prévues à l'article 4 de la proposition de loi et nous proposerons, par amendement d'accentuer encore l'interdiction de Nouma 10 des fraudeurs et des structures commerciales déviantes. Les centres de santé ont suscité beaucoup d'espoir, avant l'apparition de scandaleuse dérive. C'est pourquoi notre groupe propose dans le cas de l'examen de cette PPL de fixer un ratio d'emploi d'assistants par rapport au dentiste il aux ophtalmologiste. Les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain vont voter cette proposition de loi parcellaires mais utile mais soulignent l'absence de volonté politique de s'attaquer à la financiarisation du système de santé. Il est urgent de réécrire une nouvelle loi de santé qui structure l'offre de soins sur l'ensemble du territoire au service des Français. Et dans le respect des professionnels de santé. Merci cher collègue. Et je vais maintenant passer la parole à la présidente. Pascale Gruny pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Comme beaucoup de Français, j'ai été révolté par les récents scandales survenus dans certains centres de santé particulièrement dans des centres dentaires et ophtalmologiques dans certains cas, ils ont causé des dégâts irréversibles sur la santé des patients dans d'autres, ils les ont conduits à contracter des emprunts pour financer leurs soins avec pour conséquence des dettes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comme à chaque fois ce sont principal ne constituent principalement nos concitoyens les plus fragiles qui en ont été victimes au delà des scandales médiatiques de nombreux abus et fraudes recensées par l'assurance maladie ont malheureusement accompagner le développement de ces centres entorse aux règles déontologiques exercice illégal de la profession. Surfacturation soins non pertinents inachevé ou de mauvaise qualité. Dans un esprit de rentabilité financière certains gestionnaires mal intentionnés se sont installés dans de grandes villes. Au lieu de s'implanter dans des territoires ruraux et moins dotés dévoyant ainsi la vocation. Première de ces centres. Il est inacceptable que l'on puisse jouer ainsi avec la santé des Français. Il y a donc urgence à renforcer notre arsenal pour lutter contre ces abus, mais que de temps n'avons-nous pas perdu il y a 3 ans et demi le gouvernement a refusé de soutenir une proposition de loi du groupe Les Républicains visant à réinstaurer un agrément. Tout comme il a systématiquement rejeté les nombreux amendements au texte législatif sanitaire objectant qu'un tel problème n'existait pas. Cela étant dit, je me réjouis de l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Parlement, ce texte contient en effet de réelles avancées. Le rétablissement de l'agrément délivré par le directeur de l'ARS, l'obligation pour le gestionnaire de transmettre les contrats de travail des praticiens à l'ARS. L'obligation pour l'ARS de communiquer ces contrats de travail aux ordres ou encore l'introduction d'un numéro personnel obligatoire pour chaque praticien d'un centre de santé pour mieux lutter contre les fraudes à l'assurance maladie et réduire le risque de pratique illégale de la médecine. Je veux saluer le travail de la commission des affaires sociales et de son rapporteur Jean Sol qui ont eu à coeur de renforcer l'efficacité pratique de cette proposition de loi en précisant certaines de ses modalités opérationnelles et en veillant à la coordination d'ensemble de ces dispositions. Je suis très notamment le renforcement des pouvoirs d'information des ARS après la délivrance de l'agrément afin de faciliter les contrôles sur les Liens d'intérêts ou les contrats liant les organismes gestionnaires à des sociétés tierces ou encore le retrait possible en cas de manquement aux règles applicables, centres de santé ou relatifs à la qualité et à la sécurité des soins. L'alourdissement des sanctions applicables en cas de manquement des centres de santé à leur engagement de conformité va également dans le bon sens en portant les valeurs de l'astreinte journalière à 5000 euros au lieu de 2000 et de l'amende administrative maximale à 500.000 euros au lieu de 300.000. La Commission donne ainsi la possibilité au directeur de l'ARS de prononcer des sanctions réellement dissuasives. Enfin, je veux saluer la volonté du rapporteur de permettre aux ordres du consulter le projet de santé du centre afin d'apprécier les contrats et diplôme qui lui sont soumis en vue de la remise de son avis motivé, répondant ainsi à une demande légitime de l'Ordre des médecins. Pour toutes ces raisons je soutiendrai cette proposition de loi parce que la régulation de l'installation des centres de santé trop souvent synonyme d'entorses aux règles déontologiques de fraude à la sécurité sociale et de soins non pertinent est un combat, que notre groupe les républicains mènent depuis longtemps, nous attendons bien entendu ce texte avec beaucoup de de vigilance. Merci beaucoup pour votre attention. Merci cher collègue. Et enfin pour clore la discussion générale, je vais passer la parole à Édouard Courtial du groupe les républicains pour 4 minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur madame la présidente. Monsieur le rapporteur. Chers collègues jamais hein. Nous ne le dirons suffisamment l'accès aux soins proximité est un enjeu fondamental pour notre pays car la désertification médicale qui s'accroît encore malgré des propositions faites dans cet hémicycle et l'engagement de nombreux élus sur le terrain remet en cause une liberté fondamentale, celle de choisir d'habiter à la ville ou à la campagne. je suis convaincu qu'en participant à vider nos campagnes de leurs habitants elle fragilise notre identité nationale. Mais le combat qu'il doit être menée à tous les étages ne doit pas nous conduire à accepter les pires ZAFR de l'appât du gain d'un petit nombre d'un libéralisme débridé sans foi ni loi du l'exception de d'une exception praticiens au mépris de la santé de nos compatriotes. Ainsi, la proposition de loi visant à améliorer l'encadrement de santé, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale fait trop rare pour ne pas de souligner est indispensable à double titre, d'une part, car le nombre de cabinets dépasse aujourd'hui les 2500 se sont pour moitié des centres exclusivement dentaire et l'on compte plus d'une centaine de centres uniquement ophtalmologique ce chiffre continue d'augmenter, a bondi de 50% entre 2017 et 2021. Cet opportuniste doit donc être aujourd'hui davantage réguler car elle conduit parfois à des drames. Ainsi, d'autre part cette régulation est rendue nécessaire après les scandales que nous avons encore tous en mémoire et qui nous oblige à l'action en 2015 3 ans seulement après son ouverture d'un Dexia fermé après avoir mutilé escroqué de nombreux patients auxquels étaient proposés toujours plus date afin de maintenir des flux de trésorerie élevée en 2021 éclatait celui de proxy dentaire du nom de cette chute bourguignonne de centres exploitant les mêmes recettes avec les mêmes résultats des patients attirés par la promesse de soins à bas coût des soignants sommé de faire du chiffre des soins superflus facturée en quantité excessive des victimes parfois édenté à vie. La liste ne s'arrête pas là et d'autres affaires apparaissent au gré des signalements et des inspections. Or de telles dérives ont été rendues possibles par un assouplissement du cadre juridique applicable à ces centres afin de favoriser leur développement. La loi de 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé aux territoires avait notamment substituer au régime d'agrément, un régime de simple déclaration de conformité à la réglementation. L'ordonnance du 22 janvier 2018 avait vocation à mettre de l'ordre, notamment en interdisant à assez sans que la distribution des bénéfices issus de leur exploitation en promis bon la publicité on explique citant le principe d'une ouverture à tous les patients. Force donc est de constater que ce que la loi a défait, il nous appartient de le refaire en mieux, c'est ce qui a été entrepris et je tiens à su saluer le travail de grande qualité du rapporteur. Je salue donc son travail de grande qualité au rapporteur mais aussi celui réalisé par nos collègues au Palais Bourbon effectué dans un peu plus de Concorde semble-t-il que ces derniers jours ainsi au-delà du rétablissement de l'agrément pour ces 2 types de santé certaines avancées sont à noter comme par exemple la création d'un comité médical ou dentaire en guise de contrepoids au pouvoir du gestionnaire ou le renforcement du pouvoir de sanction de l'ARS pour plus de réactivité et de contrôle. Nécessité faisant loi j'appelle à l'adoption de ce texte afin de circonscrire une dérive et de mettre réellement fin à des pratiques inacceptables mais Madame la Ministre nous serons particulièrement vigilants quant à la mise en oeuvre de ce texte au terme de son parcours législatif afin de nous assurer de son effectivité. Pour permettent de redonner confiance aux patients envers une immense majorité de centre de soins effectuant un travail sérieux et qui pâtissent grandement de cette mauvaise presse. Je vous remercie. merci chers collègue la discussion générale est Close, nous allons passer à l'examen du texte de la commission. Et nous démarrons avec un amendement avant l'article 1er. c'est l'amendement 12. Si la présente, proposition de loi vise à lutter contre les dérives et scandales. Elle ne prend pas en compte le phénomène de multiplication de centres de santé spécialisés en psychiatrie et en gynécologie par exemple ou le lien que médecin spécialiste fait uniquement avec Telecom L'objectif des gestionnaires de ces centres et de faire de l'argent au détriment du juste soin cette dérive est actuellement à l'oeuvre, favorisée par la politique du gouvernement pour lutter contre cette financiarisation en marche. Il convient de soumettre tous les centres de santé agrément afin de limiter la multiplication de structures purement commerciale et l'emprise de la concentration capitalistique dans ce secteur. Sinon l'avis sera défavorable. Alors je rappelle, chers collègues, que la loi HPST avait supprimé l'agrément. Auxquels été jusqu'en 2009, soumis les centres de santé. Pourquoi d'une part car il fallait soutenir le développement des centres de santé, d'autre part, car l'agrément était une procédure jugée bien trop lourdes pour les autorités administratives. Alors que la charge pour les seuls centres dentaires et ophtalmologiques et déjà estimé particulièrement lourde pour les agences régionales de santé. Il me paraît tiré dit ça à ce stade de rétablir l'agrément pour tous les centres de santé, cela représenterait, vous en conviendrez non seulement un travail substantiel pour le flux de nouveaux centres mais cela aurait en outre colossal pour gérer les centres existants. Concentrons-nous à ce stade sur les activités qui ont manifestement été concerné par les dérives. Ce sera donc un avis défavorable. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Le gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement, vous souhaitiez comme l'a dit monsieur le rapporteur. Mettre un agrément. Pour l'ensemble des centres de santé, je tiens à rappeler tout d'abord l'importance des centres de santé comme ça a été rappelé par plusieurs. Sénateurs dans la réponse aux besoins de santé notamment auprès des patients les plus fragiles et pour faire une tournée actuellement des différents modes d'exercice de centres de santé je peux en témoigner. De plus les dérives observées en centre concernent des centres ayant une activité dentaires ou ophtalmologiques. Si d'autres moments venait à constater les ARS peuvent diligenter des inspections de contrôle et mettre en oeuvre une palette de réponses en cas de dérive qui vont de l'amende administrative à la fermeture du centre, l'assurance maladie peut elle aussi déconventionner les centres d'Évian. Enfin les dérives que vous mentionnez ne sont pas spécifiques au Centre de santé notamment en gynécologie cette activité, il est très rarement présente. L'article 53 de la loi de finances de Sécurité sociale a justement prévu en agrément pour les sociétés de téléconsultation qui est adapté aux exemples que vous donnez dans la présentation de votre amendement pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable à votre amendement. merci madame la Ministre, donc un double avis défavorable, madame Pumerole. Oui, merci Monsieur le Président, je voulais revenir un petit peu sur l'intérêt du Centre santé du contrôle contrôle de ses cendres santé puisque le premier de février 2022, j'avais interpellé Monsieur le Ministre de la Santé qui était alors. Olivier Véran sur le projet de vente de centre de santé appartenant à la Croix-Rouge au groupe Ramsey. Je l'avais alors interrogé sur la volonté du gouvernement de protéger notre système de santé face à cette marchandisation puisqu'il faut l'appeler comme ça. Afin de défendre en elle un égal accès à tous nos concitoyens à des soins de qualité. La réponse du ministre avait été clair, l'État n'a pas à intervenir dans le cadre d'un rachat de acteur privé par un autre et nous avaient confortés fait part de sa volonté de conserver déséquilibre que soit disant entre tous les acteurs publics, privés à but lucratif et l'associatif privé non lucratif il faut laisser agir le marché cette vision a d'ailleurs été rappelée par le chef de l'État lors de ses voeux aux soignants au début du mois de janvier. Donc après la biologie de vide, la gestion des agendas médicaux et on verra les inconvénients que cela peut avoir le rachat des cliniques par des fonds d'investissement la financiarisation de touche désormais les soins primaires, les chaînes de cliniques commerciales créent descendre santé de premier recours et plusieurs centres ont déjà ouvert leurs portes dans le cadre d'expérimentation autorisée au titre de l'article 51 de la loi de finance de sécurité sociale de 2018. Ainsi les Centres de santé de Ramsey expérimente aussi un nouveau mode de tarification la tarification à la une capitation c'est-à-dire que plutôt qu'une tarification à l'acte. Cette tarification prose sur forfait versé aux établissements en fonction du nombre et la typo tout logis des patients qu'elles accueillent l'axe le sexe et. Ce mode de tes tarification incite au tri des patients en fonction de leur rentabilité des en sélectionnant des patients les moins coûteux, les autres. Dans le monde. La prise en charge dépasseraient le montant du forfait sont dirigés vers l'hôpital public parce que ne l'oublions pas, la rentabilité reste le maître mot de ces organisations pas les besoins en santé de la population pas le service public pas l'intérêt du patient et à force. Que les pouvoirs publics doivent avoir un rôle pilote dans la gouvernance de la politique de santé la santé ne doit pas devenir une marchandise comme une autre. Merci cher collègue. Donc nous allons passer au vote sur le premier amendement. Avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté. Ensuite, nous passons aux amendements sur le, l'article 1 avec un amendement numéro 6 présentée par Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, nous proposons avec cet amendement, d'éviter de faire des amalgames avec tous les centres de santé, je l'ai dit lors de mon intervention générale les scandales sanitaires telles que ont émaillé l'image de tous les centres de santé cette PPL souhaite encadrer les dérives et c'est une très bonne chose mais la rédaction actuelle sur l'agrément risque en réalité de pénaliser tous les centres de santé même les centres de santé médicaux ou polyvalents vertueux. C'est pourquoi nous proposons d'opérer une distinction et de soutenir le principe de l'agrément pour les structures mono-professionnelles dentaires ou ophtalmologiques et pour les pseudo polyvalent dont l'activité principale et dentaires ou ophtalmologiques, ce sont ceux-là qui doivent être visés au risque sinon de jeter l'opprobre sur tous les sur toutes ces structures de stigmatiser ce modèle d'accès aux soins et donc par là même de freiner leur développement cette distinction. Nous sommes fondamental pour ne pas se tromper de cible. Nous proposons donc plus concrètement de considérer qu'au-delà d'une part principal d'activité supérieur à 50% du chiffre d'affaires l'agrément est obligatoire. L'objectif de cette PPL et je crois qu'on en est tous d'accord avec les interventions général est clairement la lutte contre les centres d'Évian et locaux aussi les moyens pour y parvenir doivent être clairement et et uniquement identifié et les cibler tel est le sens de notre amendement, je vous remercie. Merci madame Cohen. Monsieur le rapporteur. Bien chers collègues l'avis sera défavorable, alors je comprends que si le centre et pluridisciplinaire l'agrément puissent apparaître lourd pour une activité minuit minoritaire ou potentiellement limité à un ou 2 fauteuils cependant pour les nouveaux centres. Comment savoir a priori que l'activité est minoritaire sur tout cela me semble poser un problème au regard du principe d'égalité, il conduirait à traiter différemment le régime d'autorisation d'une même activité. Je le rappelle l'agrément est une procédure préalable. C'est pourquoi l'amendement ne me semblent pas opérants, ce sera donc un avis défavorable. Madame la Ministre. Vous souhaitez mettre en place une procédure d'agrément pour les seuls centres de santé une activité dentaires ou ophtalmologiques principal en vous appuyant sur leur chiffre d'affaires. Or l'activité majoritaire dans le centre de santé ne peut se caractériser avant sa création. Lors du dépôt du dossier ainsi la procédure d'agrément. A priori, serait alors inopérante. De plus, cette proposition pourrait entraîner des comportements opportunistes dans l'application de la procédure a posteriori les centres d'Évian risquant de licencier les personnels ayant pas d'activité dentaires ou ophtalmologiques dès lors que la procédure d'agrément ne leur est pas plus applicable pour ces raisons le gouvernement mais un avis défavorable à votre amendement. Bien double avis défavorable. Pas de demande d'explications de vote, je le soumets aux voix qui est pour. Qui est qui et contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté l'amendement numéro 13 madame Le Houerou. L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à lutter contre les dérives de centres de santé dentaires ou ophtalmologiques au rabais véritable structures commerciales parfois sans spécialiste physiquement presse présent, notamment pour les ophtalmos leur objectif 1er est la rentabilité au détriment et aux dépens de la qualité des soins. C'est une mesure de bon sens que nous vous proposons, nous déplorons la déshumanisation en marche notre système de santé où seule la stabilité compte ainsi pour éviter la multiplication des centres où le lien avec le médecin spécialiste se fait uniquement par consultation, nous proposons d'instaurer une obligation de présence physique d'un dentiste pour les centres dentaires en général, c'est le cas ou d'un ophtalmologue pour les centres ophtalmologiques, ça n'est pas le cas. Merci. Avis de la commission sur le rapporteur. Ce sera un avis défavorable. Chers collègues, je comprends l'intention de l'amendement mais je doute fortement de sa portée. En effet, concrètement, de telles situations sont-elles susceptibles de se produire sans que cela ne constitue déjà une fraude. Les actes ses prestations délivrées sont des actes médicaux. Il faut donc bien a priori la présence du dentiste ou de l'ophtalmologue dans le centre, l'avis est donc défavorable. Madame la Ministre. Même avis que que le rapporteur donc satisfait sinon rejet. Merci. Donc, je le soumets aux voix avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement numéro 14 monsieur. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Comme l'indique le rapporteur de la commission des affaires sociales, les centres de santé visés par la proposition de loi sont principalement implantées dans les zones urbaines. Centre, le l'ensemble des centres ophtalmologiste et pour 91% des centres dentaires. Ils sont surtout implantés dans des zones où la densité de professionnels de santé et déjà la plus dense. Ces centres de santé ne viennent pas compléter une offre de soins dégradé en Île-de-France, le nombre de centres de santé ont augmenté de 160%. Entre 2016 et 2022. Cette croissance est pour l'essentiel, tirée par les activités dentaires et ophtalmologiques la première représentent 58% du total des centres de santé franciliens contre 49% en 2017. Ces chiffres sont certainement sous-évaluée. Certains gestionnaires préférant déclaré dans le centre en médical ou polyvalents afin de ne pas attirer l'attention. Ne plus autoriser l'implantation de nouveau chantre dans les zones géographiques où ceux-ci se concentre déjà participe de la lutte contre les dérives inhérentes à la logique de leurs profits. Telle est l'objet de ces amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain. dans les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins et particulièrement élevé mais il conduirait aussi dans les 2 ans à la fermeture des centres de santé ophtalmologiques et dentaires existant dans ces territoires puisque ceux-ci ne pourrait accéder à l'agrément devenu obligatoire. Je comprends l'enjeu de cet amendement que vous portez qui est d'éviter que les centres de santé s'implante dans des territoires où le besoin n'est pas établie au détriment d'une bonne répartition géographique de l'offre de soins. Cependant, il me paraît disproportionnée dans son dispositif. J'indique par ailleurs que l'agrément pour être refusée en cas d'incompatibilité avec le projet régional de santé. Comme je l'avais expliqué en commission. Cette disposition discrète est un outil de régulation des implantations. Pouvant limiter les installations dans des zones déjà très doté l'avis est donc défavorable. Madame la Ministre. À travers cet amendement ou souhaitait interdire la délivrance d'un agrément dans les zones où le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé. Je partage totalement votre souhait de lutter contres les dérives des centres de santé d'Évian. C'est d'ailleurs l'objet de cette proposition de loi portée par la présidente Khatami cependant ne pas autoriser les seuls centres de santé créerait une rupture d'égalité avec les autres professionnels de santé, cela serait d'ailleurs préjudiciable au Centre vertueux et in fine et aux patients, notamment car elles ont une offre à tarif opposable enfin l'article 1 de cette proposition de loi répond partiellement à votre amendement car il prévoit à la ligne à sept que l'agrément peut être refusé en cas d'incompatibilité avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé pour cette toutes ces raisons je suis défavorable à votre amendement. un double avis défavorable Madame Cohen. même si le le but c'est effectivement d'éviter. L'installation de centres d'Évian et ça on le partage mais en même temps un amendement rédigé telle qu'il est rédigé et discriminatoire de mon point de vue parce que, effectivement, par exemple, il ne se concentre que sur les centres de santé n'est pas du tout sur les pratiques libérales que ce soit en individuel ou en maison de santé pluri-professionnelles. Donc en fait pour moi c'est une fausse bonne idée et pour l'ensemble de mon groupe également. merci. Donc je vais soumettre l'amendement voit avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Et l'amendement numéro 20 madame c'est mon Merci monsieur. Le Président à heure l'article 1er rétabli l'agrément des agences régionales de santé. Et aussi. D'agrément deviendrait pour se pour les Centres de santé déjà existant ne deviendraient définitifs qu'au bout d'un an à compter de l'ouverture du Centre sous réserve des résultats d'une visite de conformité notre amendement a pour objet de supprimer justement le caractère provisoire de l'agrément prévues par cet article, en effet, la mise en oeuvre de ce dispositif semble complexe pour les ARS et une incertitude plane quant à leur capacité à instruire correctement les contrôles nécessaires. Rappelons-le, un agrément préalable de l'ARS avait été supprimé en 2009, faute de moyens humains dévolus à l'ARS et en raison aussi du frein qui constituait au développement des centres de santé. Si nous saluons l'intégration par la commission sociale d'une visite inopinée dans les 12. Premiers mois suivant la délivrance de l'agrément que nous avions également d'ailleurs proposé sous forme d'amendement. Nous jugeons que cette visite inopinée et inopinés se suffit à elle-même le caractère provisoire pendant un an de l'agrément risque en effet de freiner le développement des centres de santé y compris polyvalent. La priorité devrait davantage consister en partant de l'existant à renforcer les moyens de contrôle des ARS et de et de la CPAM en conséquence. Cet amendement a donc pour objet de supprimer le caractère provisoire de l'agrément prévues par cet article, tout en maintenant. La visite inopinée dans les 12 premiers mois. Ajouté par le rapporteur au stade de la commission, je vous remercie. Chers collègues, l'avis sera défavorable cet amendement et que au contraire à la position de la de la commission qui avait adhéré au schéma proposé par le texte, adopté à l'Assemblée nationale qui prévoyait prévoyait notamment un argument de temps avec une période an durant laquelle l'agrément délivré n'être que provisoire. Cet agrément provisoire a du sens avec un retrait facilité durant l'emmener au regard de la visite de conformité. Le régime de retrait de l'agrément définitif et beaucoup plus contraignant. Il convient de maintenir cette souplesse et ce retrait rapide en cas de manquement constaté dans les mois qui suivent l'autorisation pour répondre aux contraintes et les agences régionales de santé dans leur contrôle mais aussi et surtout pour agir vite en cas de dérive. Madame la Ministre. Pas mieux que le rapporteur avis défavorable. Il y a donc un double avis défavorable je soumets l'amendement voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté, je vais soumettre aux voix l'article 1er qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er bis à même vote. Ensuite, on passe un amendement. Après l'article 1er bis. Donc il y a trois amendements identiques, le 1er présentée par Madame Cohen. Oui, merci monsieur le président. Nous sommes ici donc pour débattent d'une proposition de loi dont l'objectif est la lutte contre des structures de santé déviantes celles qui n'ont pour seule obsession, que la rentabilité financière et le profit. Il paraît donc pour le moins, totalement incompatible de laisser s'implanter dans nos territoires des des structures qui utilise le nom de Centre de santé qui sont gérés par des organismes dont la vocation est avant tout lucrative pour nous c'est antagonistes. Un bel exemple d'oxymore, la santé ne peut être considéré comme une marchandise. Ce n'est pas un slogan si des scandales comme nous les avons dénoncé dans nos différentes interventions générales ont pu éclater ont pu exister, c'est précisément parce que ce sont des structures lucrative qui était derrière et on ne parle pas ici de petites erreurs de diagnostic, on parle d'un véritable système qui s'est créé sur les failles de notre législation pour abuser des centaines de patientes et de patients dans Dexia mais Orpea aussi on ne connaît que trop les dérives d'une gestion privée lucrative. Il est temps, je crois, mes chers collègues. Madame la Ministre d'y mettre fin et nous proposons donc ici de modifier l'article L 63 23 tirer un tiré 3 du code de la santé publique pour que les personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé à buts lucratifs soient exclus de la possibilité de créer et de gérer des centres de santé, je vous remercie. Nous proposons d'interdire également la gestion des centres de santé pour les groupes de santé privées à but lucratif. Cette proposition de loi ne met pas suffisamment en cause des dérives de certains centres de santé, à savoir le caractère lucratif de certains de ces centres qui permet d'en faire des machines à profit en exploitation de la tarification et en exploitation aussi de personnes vulnérables. Donc en 2018 le gouvernement a lui-même permis aux personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé à but lucratif de créer et de gérer des centres de santé, ça ne mesure contribue à la marchandisation de la santé et organise la concurrence entre les grands groupes privés privés et d'autres acteurs dans le domaine de l'offre de soins. Nous nous opposons donc à cette marchandisation de la santé, c'est l'objet de notre amendement. Merci Monsieur le Président. Alors je peux pas être redondantes. Mais je voudrais dire que c'est pour pousser jusqu'au bout quand même. L'alerte de l'IGAS. Sur le développement série des dysfonctionnements qui a pointé la nécessité de mettre en place des garde-fous législatifs et réglementaires pour prévenir une gestion à but lucratif des centres de santé dentaires. Parce que la maximisation du profit ne peut guider, cela a été dit. La gestion des centres de santé le présent amendement entend mettre fin tout simplement à la possibilité d'ouvrir des centres de santé administrés par des gestionnaires d'établissements privés de santé à but lucratif. Pourquoi parce que le lucratif tu ouvres trouvera toujours les moyens de contourner les tentatives de régulation et nous aurons comme ça peut être une nouvelle PPL. Sur ces nouvelles façons de de de contourner. Les ces garde-fous législatifs et réglementaires. tout simplement pour mettre fin à cela, nous proposons de réserver dans le code de la santé publique, la possibilité d'ouvrir des centres de santé aux seuls organismes publics ou de l'économie sociale et solidaire, mutualiste, associatif, coopératif. Merci donc trois amendements identiques avis du rapporteur pour la commission. Avis défavorable. Nous avons vu le débat la semaine passée, l'exclusion des cliniques ne semble pas pertinent à ce stade, la commission a d'. Différentes reprises exposé de vives inquiétudes quant à la place prépondérant que tant à occuper les acteurs privés lucratifs dans la gestion de l'offre de soins sur le territoire. Nous avons considéré que ce n'était pas l'objet de ce texte, même si une vigilance nous semble particulièrement nécessaire sur ce point, il ne faut pas être naïf et sur les intentions qui sont celles de certains acteurs sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je rappelle que les dérives constatées sur les centres de santé ne viennent pas de cliniques privées gestionnaires pas d'acteurs déjà positionnés et connaisseur du système de santé. Ces dérives ont été le fait de groupes privés utilisant des associations comme paravent et avec des gestionnaires déconnectés du monde de la santé. Je pense en outre que les groupes de santé gérants des établissements de santé ont un enjeu réputationnel les invitant à être exemplaire. Un scandale pouvant atteindre toute leur activité, l'avis est donc défavorable. Merci à vide, madame la Ministre. Vous souhaitez interdire aux établissements de santé lucratif de créer et de gérer des centres de santé, si un établissement de santé lucratif peut actuellement créer et gérer un centre de santé cette possibilité, nous, on met toutefois pas en cause l'obligation de gestion non lucratif du dudit centre ainsi une clinique gestionnaire a interdiction de redistribuer les bénéfices issus de l'exploitation de son centre de plus les dérives qui ont été observées concernent exclusivement des centres de santé, géré par des associations à but non lucratif qui détourne ce statut pour frauder votre proposition n'aurait donc pas d'effet sur les déviances contre lesquels la proposition de loi entend lutter pour l'ensemble de ces raisons je suis défavorable à votre amendement. un double avis défavorable sur ces trois amendements que je vais soumettre aux voix l'amendement cinq amendement 17 rectifier l'amendement 21 rectifié. Qui est favorable à ces amendements. Qui est contre. Qui s'abstient et ne sont pas adoptés. Ensuite, nous passons à l'article 1er bis. L'amendement 24. Sur le rapporteur. Monsieur le président. Cet amendement a pour objet une coordination rédactionnelle. Madame la ministre, avis favorable. Favorable. Donc amendement rédactionnel avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient est adopté l'amendement 22. Madame Poncet Monge. Merci monsieur le président. Alors l'article 1 bis a été introduit. Par un amendement du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, donc nous nous en félicitons. En effet, il prévoit l'impossibilité de cumuler la direction d'un centre de santé avec une fonction dirigeante de la structure gestionnaire et se fondent sur les conclusions du rapport de l'IGAS sur les centres de santé dentaires. Ce rapport met en lumière des montages juridiques opaques dans le, dans le cas de plusieurs centres de santé dentaires visités par la mission qui aboutissait à remettre en cause le principe de non-lucrative IT des associations gestionnaires des centres de santé. Je cite le rapport, au-delà de ses limites par une société dont l'association est la seule cliente donc de fait par l'argent provenant de l'association dont il est président. Pour contrer ces pratiques l'IGAS recommandait de systématiser la déclaration des Liens et conflits d'intérêts des dirigeants des associations gestionnaires cite d'exclure la poursuite des fonctions au sein de la structure gestionnaire lorsqu'ils ont un intérêt Direct ou indirect avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. En conclusion n'autrement notre amendement vise à préciser la rédaction de l'article 1er bis afin que cette piste de régulation n'emporte pas d'effets disproportionnés sur les structures mutualistes coopératives lorsque leur organisation est réalisé dans le cadre de groupement d'achat au statut de groupement d'intérêt économique. Merci. Monsieur le Président c'est un avis défavorable. Je tiens à souligner que le caractère lucratif ne se postule il conviendrait de parler de but lucratif sur le fond, je considère qu'il conviendrait de mieux expertisée par ailleurs les cas réel ou la disposition serait bloquant en matière de gestion. Quelle situation concrète d'incompatibilité de gestion. Les mutuelles qui ont suggéré cet amendement n'anticipe-t-elle. La vie est donc défavorable. Le. Merci madame la ministre. Avis du gouvernement. Un avis défavorable. Vous souhaitez que l'interdiction d'exercice d'une fonction dirigeante lorsqu'il y a des Liens d'intérêts avec des entreprises privées, soit restreinte à des entreprises uniquement lucrative. Or dans le cas de la gestion des viandes de ces centres de santé, il a été fréquemment constaté le détournement du caractère non lucratif de ces structures aussi il apparaît nécessaire de contrôler l'ensemble des Liens financiers du gestionnaire, y compris avec des prestataires non lucratif l'interdiction d'exercice étant contrôlé par l'Agence Régionale de Santé, le directeur général appréciera la nature et les risques des Liens d'intérêts. Afin d'éviter un usage disproportionné de cette interdiction, en particulier auprès de structures vertueuse pour ces raisons je suis défavorable à votre amendement. Il y a donc un double avis défavorable, je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je soumets aux voix l'article 1er bis qui est pour.

La mise en place d'un comité médical au niveau de chaque centre pose des difficultés pratiques d'abord quand il s'agit de petits Centre puisque s'il y a qu'un seul cabinet, voire de praticiens dans un cabinet c'est pas ça pose une difficulté particulière et puis aussi lorsqu'il s'agit de centres pluridisciplinaires dans lesquelles retrouvera une, voir plusieurs. Voire plusieurs comités médicaux pour ces raisons, il est donc proposé que le comité médical soit mis en place au niveau de l'organisme gestionnaire. Et non pas dans chacun des centres et dans quel gestionnaire une activité nationale pluri-régional le comité pourrait être mis en place au niveau régional sur le parrain périmètre de l'ARS. Par ailleurs, il est essentiel pour que le comité joue un rôle sur les modalités de gestion du Centre que le représentant de l'organisme gestionnaire puissent y participer, comme dans le cas des comités médicaux mis en place dans les hôpitaux.

il nous a été. Transmis par les organismes gestionnaires de centres de santé en effet selon le Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé qui regroupe la Fédération de l'aide à domicile. La Fédération des Mutuelles de France, la FEHAP, la Croix-Rouge et l'Uniopss, l'article 2 propose une double difficulté, d'une part, la rédaction ne tient pas compte des difficultés de la création d'un comité ophtalmologique ou dentaires pour les centres de santé. De faible taille, d'autre part et c'est le principal grief de l'article de ce comité de près de professionnel de santé ne prévoit pas la présence de l'organisme gestionnaire. Dès lors, cette instance qui va doublonner l'instance de dialogue social sans représentants des salariés du centre de santé ne pourra jouer le rôle d'un dialogue social ou même d'organisation du Centre de tant que le représentant. De l'organisme gestionnaire en ect exclus, ça va de soi. Cette exclusion est d'autant plus préjudiciable que seul le représentant légal de l'organisme gestionnaire, assume la responsabilité pénale en cas de non respect des règles de sécurité, d'hygiène et de comptabilité vis-à-vis de l'assurance maladie alors même que ce texte vise à lutter contre les centres de santé déviant, il apparaît que la présence de l'organisme gestionnaire. Est indispensable dans ce comité. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président oui cet amendement est identique à celui qui vient d'être défendu par mes collègues, mes collègues, je voudrais néanmoins. Dire que il me semble quand même préférable aujourd'hui de renforcer plutôt le contrôle de la bonne application des dispositifs de droit commun pour garantir le respect des bonnes pratiques. Je pense en particulier aux obligations ordinale conventionnelle au contrôle de l'assurance maladie obligatoire pour autant à partir du moment où où un comité médical ou dentaire et créer. C'est le sens de cet amendement il me semblait important que ce soit mis en place au niveau d'un organisme gestionnaire et non pas au niveau de chaque centre. Merci donc 6 amendements identiques, enfin 5 il reste 5 mai. Monsieur le rapporteur. Madame Poncet Monge. Peut être ajouté que dans de petits centres, notamment dans le secteur dentaire n'exerce qu'un ou 2 par praticien de plus dans les centres pluridisciplinaires. Il y aurait un voire 2 comités médicaux pour les activités visées par la proposition de loi alors que ce dispositif n'existera pas pour les autres disciplines. fait effectivement. L'objet de l'amendement est le même, c'est bien effectivement suggéré par la Mutualité française de proposer que le comité médical soit mis en place au niveau de l'organisme gestionnaire et non pas au niveau de chaque centre. Merci donc monsieur le rapporteur. très intéressantes mais totalement contreproductive et certainement contraire à l'esprit de la loi. Le comité médical, ophtalmologique, a vocation à faire contrepoids au pouvoir de gestionnaire pour contrebalancer la logique de gestion efficace par une logique prenant mieux en compte l'amélioration de la qualité de la sécurité des soins. C'est bien de ça dont il s'agit. Associer le gestionnaire à s'est réunis à ces réunions pardon risquerait donc d'en saper le principe même, il semble par ailleurs plus efficace de le positionner le comité à l'échelle des centres plutôt que des organismes gestionnaires afin de faire remonter rapidement les risques de dérive compromettant la qualité des soins. Le décret pourra parfaitement adapté les modalités de fonctionnement des comités à la taille et descendre ce que vous venez d'exprimer avis défavorable. Madame la Ministre. Monsieur le Président. Donc vous souhaitez à travers cet amendement que le comité médical soit installé non pas au niveau de chaque centre mais au niveau de l'organisme gestionnaire du Centre de santé. Vous proposez aussi de permettre à l'organisme gestionnaire d'être membre de ce comité. Au vu des enjeux de qualité et de sécurité des soins, il est nécessaire que le comité soit situé au sein de chaque centre afin d'être plus proche des pratiques de terrain et de pouvoir en signaler les éventuels dysfonctionnements. De même, il est nécessaire de permettre à l'ensemble des salariés concernés, d'être présente à l'échelle de leur lieu de travail. Il convient également que le gestionnaire en soit exclu afin d'offrir une instance dépendante favorisant le dialogue et les Brawn pratiques en matière de soins, nous avons vu trop dérive en la matière. Il me semble que cet amendement va à l'encontre de la proposition de loi sur laquelle nous sommes en en train de discuter, donc je suis défavorable à votre amendement.

Oui moi je voulais dire que sur ces amendements en effet je je conçois qu'ils aient été proposé à nos collègues par des. Que ce soit la Mutualité française par en effet des des organismes qui ont des centres. Tout à fait classique classique et qui ne rentre pas dans les dérives. Mais l'objectif du comité médical c'est justement d'éloigner le gestionnaire et si on met le gestionnaire à l'intérieur du comité médical on perd tout le bénéfice du texte.

que vous soutenez de bonnes intentions mais qui peuvent avoir des conséquences à l'encontre du texte et je porte je rappelle de plus que Jean Sol va proposer pour les petits centres, là où il y avait des médecins que ce soit plutôt un comité élargi aux professionnels de santé du centre donc. On sera sur un nombre plus important mais attention au risque que cet amendement fait courir à la proposition de loi. Madame Cohen. C'est juste pour dire qu'effectivement. On le retire.

Vous mettez votre amendement. Le groupe les indépendants, vous maintenez votre amendement pardon. Il est routier, il Excusez-moi, je suis un peu souvent. Alors donc. Les amendements sont retirés donc. Nous passons au suivant l'amendement. Présenté par le rapporteur Monsieur Alors cet amendement dis ça permettre d'intégrer au comité des professionnels paramédicaux dans le cas des comités ophtalmologique, il serait par exemple pertinent. De permettre aux orthoptistes de prendre part aux travaux d'amélioration de la qualité et de la sécurité de soins dans le comité et de garant. Madame la Ministre. Les professionnels de santé non médicaux tels que les assistants dentaires ou les orthoptistes interviennent à part entière dans l'activité dentaires ou ophtalmologiques du centre. De plus les dérives observées dans certains centres sont souvent très à des glissements de tâches. La politique d'amélioration de la qualité de la pertinence et de la sécurité des soins, ainsi que la formation continue de salariés concerne bien l'ensemble des professionnels de santé dédiée aux activités pour cette raison, je suis favorable à votre amendement. Donc un amendement de la commission du rapporteur avec avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Amendements suivant le 26 Monsieur également. Cet amendement vise à renforcer les obligations d'identification des professionnels réalisant les soins des patients pris en charge en centre de santé en prévoyant une information sur les praticiens dès la prise de rendez-vous. Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Vous proposer à travers votre amendement, de renforcer les l'homme les obligations d'identification des professionnels de santé en prévoyant une information du patient, dès la prise de rendez-vous cette obligation va dans le sens d'une meilleure information des patients et d'un meilleur contrôle des éventuelles dérives aussi, je suis favorable à votre amendement. un amendement du rapporteur avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Ensuite de. Deux amendements en discussion commune le 11 rectifié madame Le Houerou. c'est un amendement qui vise à instaurer un ratio d'emploi d'assistants dentaire par rapport au dentiste et d'assistants médicaux par rapport aux ophtalmologistes. Il s'agit ainsi de garantir des conditions d'une prise en charge adéquate des patients et la qualité des soins. Cet amendement reprend d'ailleurs une disposition qui étaient inscrites dans la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé qui a été supprimée par la rapporteure de la commission des affaires sociales, madame la sénatrice Imbert au motif qu'elle trouverait davantage sa place dans la proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé et nous trouvons que c'est une bonne proposition. Merci. Merci et donc l'amendement 3 rectifier Madame Imbert. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues. Oui en effet ben comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, cet amendement propose d'introduire un ratio de 1 pour 1 dans les centres de santé ophtalmologique entre le nombre d'assistants médicaux, et le nombre de médecins cette limitation serait un garde-fou utile pour éviter des dérives dans des centres de santé peu scrupuleux. Cette disposition, comme l'a rappelé notre collègue adopté à l'Assemblée nationale au sein de l'article 4 bis de la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ne plus naturellement sa place dans la présente, proposition de loi. C'est pourquoi notre commission des affaires sociales a supprimé en commission et que cet amendement propose de la réintroduire au présent article de. Merci donc avis du rapporteur sur ces deux amendements. Monsieur le président, sur l'amendement porté par Madame, le héros et ses collègues cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi pour amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé consistante à plafonner le nombre d'assistants dentaires et ophtalmologiques au niveau des praticiens médicaux. Or la disposition concernant les assistants dentaires maintenu dans la proposition de loi voisine et celles relatives aux assistants ophtalmologique est défendue par l'amendement de Madame Imbert, par souci de clarté, je vous demande donc le retrait au profit de l'amendement de Madame Imbert à défaut l'avis sera défavorable. Concernant l'amendement de Madame Imbert, cet amendement plafonne dans les centres ayant une activité ophtalmologique le nombre d'assistants médicaux, au niveau du nombre d'ophtalmologues. C'est une disposition issue de la proposition de loi relative à la confiance dans les professionnels de santé qui vise à limiter les dérives dans les centres peu scrupuleux qui seraient tenté de substituer des assistants au médecin dans un souci de compression des coûts, la vie sera favorable. Madame la ministre. Pour les mêmes raisons évoquées que le rapporteur sur l'amendement. 11 rectifié de Madame Le héros nous émettons un avis demande de retrait sinon un avis défavorable au profit de l'amendement porté par Madame Imbert, l'amendement numéro 3, qui souhaite limiter le nombres d'assistant médical au nombre de médecins présents dans centre de santé, il en est une activité ophtalmologique votre proposition permet de lutter contres dérives observées dans un certain nombre de centres ou les assistants médicaux étaient présents en grand nombre et effectuer des tâches qui ne l'étaient pas forcément dévolue afin d'éviter les de salariés des médecins. Cette situation constitue un risque grave de compromission de la sécurité et de la qualité des soins délivrés sa disposition figurait d'ailleurs initialement dans la proposition de loi de madame Rist pour ces raisons, je suis favorable à votre amendement. Bien, donc un avis madame Le Houerou. Donc vous vous retirez l'amendement au profit de me de, souligne Tirs au profit de celui de Madame Imbert, donc. Nous partageons vos observations. Et donc je soumets l'amendement. 3 rectifier bis. On voit avec un double avis défavorable qui est pour. un double avis favorable. Pardon, mais je crois que tout le monde avait compris, excusez-moi, c'est la fatigue donc pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Je me vois l'article 2 qui est pour. Les contre qui s'abstient-il être adopté. Nous passons après l'article de un amendement numéro 9 Madame Cohen. Oui merci messieurs le président lors de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 un amendement avait été adopté visant à autoriser à titre expérimental, pour une donnée de cinq ans à déroger à l'article L. 5 du code de la santé publique au terme duquel les professionnels qu'exerce au sein des centres de santé sont salariés. Je me permets de rappeler que notre haute assemblée sur la proposition de mon groupe avait supprimé cette disposition cette expérimentation entre en contradiction avec un des principes qui fondent naissante de santé le salariat qui participe de l'efficacité de la pertinence de ce mode d'exercice regroupé et coordonner la possibilité pour les centres de santé d'avoir recours à des médecins gardant leur statut libéral avait déjà été examiné et rejeté en 2017 et en 2018 par les services du ministère de la Santé en particulier par la direction générale de l'offre de soins la DGOS. En effet, en concertation avec toutes les organisations des Centres de santé les gestionnaires et les professions de santé avait donc rejeté. Rien n'interdit et ça je le dis, je le spécifie à des praticiens libéraux d'exercer dans des champs de santé comme salariés. Ce cas d'activité mixte libéral et salariés et choisi par de nombreux partis sien et fréquemment rencontrés en de santé il satisfait toutes les parties depuis toujours. Il travaille en libéral et en centre de santé en tant que salarié. L'exercice libéral ensemble de santé témoignent d'une grande méconnaissance des caractéristiques fondamentales de ces centres, elle crée une confusion qui troublera certains promoteurs et professionnels de santé au moment de la construction des projets alors que de nombreux élus de toutes sensibilités, se tourne vers la création des centres de santé. Nous souhaitons donc profiter de cette PPL pour revenir sur cette mesure car nous considérons depuis le début qu'elle constitue un danger pour le mode d'organisation des centres et pour les valeurs qu'ils portent. Je vous remercie. Alors sur un avis défavorable chers collègues cet amendement abroge la disposition qui autorise la dérogation au principe du salariat dans les centres de santé. Introduite en 2019 à titre expérimental pour 5 ans dans les zones sous-denses. C'est un avis défavorable à la suppression d'une telle mesure d'application temporaire dont les effets n'ont pas été évalués. Madame la ministre. Oui, monsieur le président. Merci, comme vient de l'expliquer monsieur le rapporteur. Nous sommes ici dans le cadre d'une d'une d'une expérimentation qui n'a pas été terminé et laissons l'expérimentation aller jusqu'au bout et nous et vu le nous évaluerons cette. Cette évaluation qui doit durer pour 5 ans depuis 2020. C'est pour cette raison que nous sommes défavorables à votre amendement. Il y a donc un double avis défavorable Madame Cohen.

moi en général je me méfie toujours des des positionnements à géométrie variable et j'aimerais un peu plus de de cohérence surtout de la part du gouvernement, ça c'est ma première remarque.

fonctionne avec des professionnels qui exercent en tant que salarié à l'intérieur de ses cendres, de santé et qui exerce en tant que libéral à l'extérieur de ces centres de santé et ça ne pose aucun problème, au contraire, c'est la complémentarité de leur activité qui fait que, hé bien ils peuvent travailler dans les centres dans donc je ne vois pas là ce que vous a pas ramené de la de la confusion en permettant une espèce de perméabilité qui n'a pas de raison d'être. Je je je, vraiment. Nous maintenons notre amendement. Bien donc je l'amendement est maintenu avec un double avis défavorable qui est pour. Donc. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mets aux voix l'article 2 bis qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté l'article 3 a été supprimé, nous passons à l'article IV. L'amendement de Monsieur. Le numéro 16. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à éviter le nomadisme des fraudeurs et des structures commerciales déviantes

Mon cher collègue, cet amendement précise que le motif pris par le directeur général de l'ARS d'une décision de suspension ou de fermeture de centres pour refuser l'ouverture d'une nouvelle antenne ou un le Nouveau Centre doit s'entendre sur tout le territoire national. L'amendement semble satisfait par la rédaction de l'article et la création du répertoire national des mesures de suspension et de fermeture qui sera rendu accessible au service de l'État intéressé même s'il est vrai que la précision ne nuit pas, je vous la courbe. Je suis plutôt favorable à un retrait. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur vous souhaiter préciser le périmètre national de cet article qui permet au directeur général de l'Agence Régionale de Santé de refuser l'ouverture d'un centre de santé lorsque le gestionnaire a déjà vu un autre de ses centres. Il s'agit bien de l'objectif de cet article qui crée également un répertoire national permettant de recenser l'ensemble des mesures de suspension et de fermeture des centres de santé sur le territoire et ainsi apporter connaissance. Une connaissance nécessaires à l'application de cette mesure pour cette raison, je suis favorable à votre amendement. Bien, donc je vais soumettre l'amendement voit avec un avis favorable du gouvernement un avis de retrait de demande de retrait de la commission donc qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Donc il est adopté. Je mets aux voix maintenant l'article IV. Qui est pour l'article IV.

Vote sur l'article 8, un amendement monsieur Iacovelli. Oui, monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission l'amendement présent vise à renforcer la protection des patients et de se prémunir des pratiques déviantes existantes. Il vise en effet à rétablir la base légale permettant le déconventionnement d'urgence des centres de santé ayant commis des violations graves des engagements prévus ou ayant engendré un préjudice financier, il s'agit d'une modification nécessaire suite à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Monsieur le rapporteur. qui peut être lancé lorsqu'une violation particulièrement grave désengagement prévus par la convention ou ayant engendré un préjudice financier pour l'organisme de Sécurité sociale a été commise. Il est bien sûr utile de la rendre applicable à nouveau au centre de santé en rétablissant la rédaction initiale du code de la santé publique issus de la L. F SS pour 2022, la vie sera donc favorable. Madame la Ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur, à travers votre amendement ou souhaiter rétablir la base légale permettant l'application de déconventionnement d'urgence des centres de santé. La loi de financement pour 2022, en renforçant le dispositif de déconventionnement des professions de santé fraudeurs. A malencontreusement supprimé la base légale du déconventionnement en urgence des centres de santé introduite dans la la FSS précédente votre amendement rétablit cette possibilité qui permet de limiter le préjudice subi par l'assurance maladie en cas de faute grave. Le gouvernement partage votre objectif de sanctionner de manière adéquate les centres de santé d'Évian. Je suis donc favorable à votre amendement. Bien, donc un double avis favorable je soumets l'amendement voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté, je mets aux voix l'article 8 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté l'article 9 a été supprimé. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, y a-t-il des demandes d'explications de vote. Donc je le, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé qui est pour. Qui est contre. Il n'en a pas qui s'abstient. Il y a pas d'abstentions, le projet de loi est adopté à l'unanimité. Donc je vous propose, puisque les les mêmes vont participer au débat qui qui s'enchaînent de ne pas suspendre la séance et on va enchaîner directement. si vous êtes d'accord. Madame la présidente, vous souhaitez non c'est bon OK. Donc. Donc nous allons enchaîner l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi. Adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Et dans la discussion générale. La parole est donc à Madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Monsieur le président, madame de la présidente de la commission, madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs. Le début de l'année 2023 a été marquée dans le monde de la santé par d'importantes annonces. Le 6 janvier dernier, le président de la République a tenu à adresser ses voeux directement aux acteurs de la santé. Cela témoigne de l'importance accordée à ce que nous réussissions les changements profonds auquel aspirent les professionnels de santé et les Français. Avec le le Ministre de la Santé de la prévention François Braun. Nous avons également tenu à nous adresser fin janvier à toutes nos forces vives pour détailler la feuille de route et les jalons de cette refondation. Moins de 15 jours plus tard, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui traduit ses paroles fortes en actes concrets. Ce texte comporte de nombreuses dispositions importantes pour accélérer le décloisonnement de notre système de santé. Cette proposition de loi a été déposé par la rapporteure générale Stéphanie Rist est co-signé par l'ensemble du groupe Renaissance. Elle témoigne du besoin ressenti sur le terrain de favoriser les coopérations entre les professionnels de santé, en ville comme en établissement. Cela doit nous permettre sans dégrader la qualité des soins et encore moins en créant une médecine à 2 vitesses de libérer du temps médical et de faciliter l'accès à la santé. Et je veux le dire alors que nos médecins généralistes manifestent aujourd'hui il ne s'agit pas de nier le rôle essentiel du médecin généraliste c'est lui dans le cadre des coopérations dont je parlais, qui est au centre du parcours de soin, car il dispose d'une expertise essentiel. Nous devons Poursuivre la transformation de notre système de santé pour répondre à des besoins qui évoluent et une démographie médicale qui est celle que nous connaissons. En effet, la pandémie mondiale de Covid-19 a profondément bouleversé notre système de santé qui pour faire face à déployer des ressources et des moyens parfaitement inédit. Nous avons inventé des solutions expérimentées des modes d'organisation innovants et bâti des solidarités nouvelles. Je pense par exemple à l'extension des compétences vaccinales aux professionnels de proximité en 2021 qui a permis d'accompagner le déploiement d'une campagne de vaccination massive, qui fut une réussite collective. Un progrès que nous avons ensuite entériné dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. En élargissant l'accès à la prescription de vaccins au pharmacien maïeuticien et infirmiers. Car les contextes de crise on peut être le seul avantage d'être des vecteurs de transformation et des catalyseurs de changement portant eux les ferments d'une résilience de renouveler une fois les difficultés surmontées. Le budget pour 2023 de la Sécurité sociale prend d'ailleurs de nombreuses autres mesures opérationnelles et efficace pour l'accès aux soins, dont certaines sont d'origine parlementaire et transpartisane. Je pense à la simplification des aides à l'installation aux expérimentations relatives à l'établissement de certificat de décès par les infirmiers ou ou aux consultations avancées en zone sous-dense. Nous avons récemment lancé une expérimentation qui permet aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentale dans certaines conditions et dans un cadre sécurisé ce nouvel élargissement de compétences va être généralisé, fin 2023, renforçant ainsi l'accès à l'IVG pour toutes les femmes. Dans la continuité de la dynamique amorcée pour faire face aux défis actuels et futurs qui sont immenses, il nous appartient de nous inscrire dans ce mouvement qui fait bouger les lignes et de tracer le chemin d'un système de santé ou chaque professionnel trouve sa place. Ce système de santé que nous refont dont il doit être celui où le cadre une confiance et d'une collaboration renforcée entre tous les professionnels, permet de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et de lutter contre toutes les inégalités d'accès aux soins. la pandémie de Covid est désormais derrière nous, nous faisons face à d'autres défis majeurs auxquels il faut opposer des actions immédiates adossés à des changements structurels. Il faut nommer les choses. L'urgence à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est celle d'une crise de l'accès à la santé. En matière de santé publique, une bonne politique et celle qui fait se rencontrer le temps de la gestion des crises avec les nécessités de plus long terme. En ce qui concerne les médecins, nous avons corrigé une erreur historique en supprimant le numerus clausus. Il faudra toutefois attendre encore des années avant d'en voir les effets sur le terrain. Dans le cadre d'un grand pacte autour de la formation que nous construisons avec les régions. Nous avons déjà ajouter plus de 5000 places supplémentaires dans les instituts de formation en soins infirmiers et plus de 3000 en institut de formation d'aide-soignant. Par ailleurs, nous comptons déjà plus de 200 infirmiers et infirmières en pratique avancée et les 4000 assistants médicaux, nous en visons 10.000 d'ici 2024. Aujourd'hui, notre objectif et notre défi au delà de poursuivre le renforcement de nos effectifs c'est de mobiliser tous les leviers nous permettant de mieux partager les tâches et de gagner du temps médical pour nos soignants au service des patients. Les leviers que nous activons ici sont la rénovation des métiers du soin avec des compétences élargies pour chaque acteur de santé dans le rôle qui est le sien. La rénovation de l'organisation du parcours de soins autour du médecin traitant pour que chacun avec ses compétences soient le plus efficace possible au service du patient. Tout cela dans une logique partenariale entre les soignants dans une logique de confiance entre les pouvoirs publics et des professionnels et de coopération entre la ville et l'hôpital dans un esprit de dialogue et de responsabilité partagée. C'est là aussi un enjeu majeur d'attractivité et de fidélisation pour les jeunes en particulier alors que je souligner l'insuffisance de l'offre de soins par rapport aux besoins croissants de la population. Vous l'aurez compris, il s'agit de répondre à la double exigence de renforcer l'accès aux soins pour les Français et de donner de nouvelles responsabilités et perspectives d'évolution professionnelle aux soignants. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés grâce à cette proposition de loi qui nous permet d'avancer dans la voie du renforcement de la pratique avancée de l'accès Direct des partages de compétences et délégations d'actes qui doivent se déployer dans des organisations territoriales collective et coordonnée. Grâce à un débat parlementaire transpartisan de grande qualité, nous avons pu faire de ce texte un vecteur pour de nombreuses avancées qui n'était pas prévu dans le dispositif initial. Je pense par exemple à la possibilité pour les personnes souffrant de diabète, de pouvoir se faire prescrire directement par les pédicure pour de Gaulle podologue des orthèse plantaire à la possibilité pour le pharmacien de renouveler les traitements chroniques lorsque le médecin prescripteur n'est pas disponible pour une durée de maximal de 3 mois à la possibilité pour les infirmières formées à cet effet de prendre en charge le traitement des problèmes chroniques. À l'évolution du métier d'assistant dentaire en lien avec la demande exprimée par les chirurgiens dentistes pour libérer du temps médical. Ou encore à la reconnaissance des assistants de régulation médicale comme professionnel de santé qui contribue à améliorer l'attractivité d'une profession concentrant d'importants besoins de recrutement. Je salue ces élargissements et ces facilités d'accès et je suis profondément convaincu que le chemin que nous empruntons et le bon. Je veux aussi saluer Madame la rapporteure le travail effectué par les sénateurs en commission des affaires sociales. J'ai par ailleurs été sensible aux questions portant sur les évolutions du statut des infirmiers anesthésistes diplômés d'État Iyad. Les métiers des soins infirmiers sont aussi divers qu'indispensable et j'accorde la plus grande attention aux réformes qui les touchent. Des professions d'Iyad d'infirmiers de bloc opératoire i-mode d'infirmiers pure et culture sont aussi spécifique que celle d'infirmiers en pratique avancée qui est plus récente elle nécessite chacune une définition en propre d'un cadre d'exercice en pratique avancée. Un cadre qui est appelée à se stabiliser autour de concertation que nous mènerons et poursuivront en associant les parties prenantes intéressées. Le rapport IGAS IG ESR de Jean Debeaupuis et de Patrice Blaimont une que nous avons rendu public en janvier propose dans cette perspective de maintenir la notion de spécialité infirmière notion qui est ancienne et qui reste en France structurante dans l'identité dans l'identité de ces professionnels. La commission des affaires sociales du Sénat a choisi de ne pas retenir les dispositions distinguant IPA spécialisé et praticiens. Suite aux concertations que nous avons menée avec les représentants professionnels cette distinction semble en effet inadaptés au système français. Le gouvernement soutiendra donc ce choix. Les Ziad Bode QR toutes et tous sont une page à écrire dans ce que nous élaborons actuellement autour de la pratique avancée des parlementaires qui veulent être associés à ce travail qui sera suivie d'évolution principalement réglementaires sont bien entendu les bienvenus. Attentive à tous ces sujets, je le suis également tout particulièrement à certaines craintes qu'ont pu exprimer les médecins généralistes. Je veux encore m'adresser ici autant vous qu'à eux qui sont pour certains aujourd'hui dans la rue en grève. Je le redis, je le répète, l'objectif n'est en aucun cas de mettre de côté le médecin généraliste. Au contraire, c'est en renforçant la place centrale du généraliste traitant que nous voulons accroître le niveau de coopération entre les professions de santé autour du rôle pivot du médecin. Le président de la République l'a rappelé lors de ses voeux aux soignants. Nos médecins généralistes sont pour les Français le visage le plus familier de notre système de santé. La médecine de ville et la colonne vertébrale de notre système de santé, les généralistes, voient en moyenne un million de patients par jour. Ce chiffre est important et cela doit rester un motif de fierté pour la profession. Mais cela ne change rien au fait qu'aujourd'hui 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant c'est une c'est une situation qu'on ne peut accepter sans rien changer. C'est pour cela qu'il est indispensable de trouver les voies qui nous permettront de trouver, de trouver de toujours mieux concilier le principe de liberté qui structure la médecine libérale et qui ne saurait être remise en cause avec la nécessité d'un engagement territorial concernant en plus grand nombre de professionnels de santé. nous souhaitons qu'il y ait une part structurant de la rémunération qui repose sur ses objectifs de santé publique à l'échelle d'un territoire. Je crois profondément que le médecin traitant, assure un rôle central dans la réponse locale aux besoins de santé. Nous devons mieux reconnaître et mieux valoriser ce rôle quand un médecin s'engage pour ses patients et s'engage pour créer de la coopération à l'échelle de son territoire. Pour susciter et cet engagement, la solution n'est pas de créer de la contrainte, mais encore une fois d'accélérer les coopérations et l'exercice coordonné. C'est ainsi par une démarche collective pour la santé des Français qu'il nous faut encourager le plus grand nombre de médecins à s'engager au service de leurs patients et de leur territoire. Certains le font déjà et ils doivent pouvoir à ce titre-bénéficier d'une valorisation financière supérieure ce mécanisme d'engagement territorial que nous voulons inscrire dans la loi aura des traductions très concrètes. Il s'agit par exemple d'accepter de prendre en charge des patients qui ne trouvent pas de médecin traitant. D'assurer des soins non programmés, de limiter le reste à charge pour les patients ou bien encore de proposer des parcours de prise en charge pluri-professionnelles par l'exercice coordonné. Oui nous sommes toi mettre plus de moyens pour nos médecins généralistes mais pour qu'il soit efficace, il s'agit de les mettre au bon endroit. J'entends les craintes et je veux les rassurer mais je veux aussi profiter de cette tribune pour appelé chacun au sang-froid et déconstruire certaines affirmations que l'on peut entendre et qui relève de l'instrumentalisation politique. J'ai pu le détailler les mesures d'accès Direct ne sont en aucun cas généralisée. J'ai pu entendre que les serait une menace pour les médecins, encore une fois je m'inscris en faux. Cette montée en charge des infirmiers en pratique avancée ce déploiement d'assistants médicaux et bucco-dentaire cet accès plus facile aux kinésithérapeutes, orthophonistes, le tout dans le cadre d'un exercice coordonné pour le bien des patients. Ce sont autant de professionnels directement au service de ses patients que d'or gagner pour nos médecins, qui ont tout à y gagner. Mesdames, et messieurs les sénateurs pour réussir à convaincre sans contraindre et à transformer sans abîmer nous devons collectivement nous projeter dans une vision systémique de la réponse aux besoins de santé où chaque professionnel et chaque structure à sa juste place sera le plus efficace et le plus utile. Nous débattons aujourd'hui pour progresser dans cette voie et structuré ensemble les déterminants de l'exercice professionnel médical de demain. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement et la compétence des sénateurs dans ce travail collectif. Encore une fois et toujours au service de la santé de tous nos concitoyens, je vous remercie. Merci madame la ministre et je passe maintenant la parole à notre collègue Corinne Imbert rapporteure de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la Ministre, madame la présidente de la commission. Mes chers collègues. Lors du dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale. La commission des affaires sociales appelé de ses voeux une loi santé pour examiner les dispositions touchant aux compétences et aux conditions d'exercice des professionnels de santé. Les délais contraints attaché à l'examen d'un texte financier ne nous saouler ne ne semblait pas permettre le débat serein que ce type de mesures nécessite. Il faut croire Madame la Ministre que nous sommes mal compris. Le gouvernement a choisi de profiter d'un texte déjà hautement sensible discuté à l'Assemblée nationale pour insérer diverses dispositions sans étude d'impact et il faut le dire sans cohérence d'ensemble ni vision à long terme. Puis il a opté pour une inscription sans délai à l'ordre du jour du Sénat laissant moins de 2 semaines à la commission pour examiner le texte. Ne s'agit pas seulement d'un reproche fréquent et mérité sur le respect du travail parlementaire si j'insiste sur la méthode employée, c'est que cet examen précité a un effet délétère. Parmi les professions de santé et ruinent l'ambition affichée dans l'intitulé du texte. Loin de favoriser la confiance parmi les professionnels de santé. Le texte à opposer les professions entre elles ces dernières semaines. Très attendues des paramédicaux dont il valorise les compétences il a suscité. À l'inverse, l'incompréhension et l'inquiétude de nombreux médecins, jugeant que certaines de ces dispositions désorganise le parcours de soins présentaient un risque de dégradation de la qualité des prises en charge et in fine et de perte de chances pour les patients. Or l'examen intervient concomitamment aux négociations de la prochaine convention médicale et contribue largement à en détériorer le climat il lui était difficile de choisir un moment plus inopportun pour discuter de ce texte. Un mot en fin de la seconde ambition de la proposition de loi, l'amélioration de l'accès aux soins. Je crois, mes chers collègues, qu'il ne faut pas se bercer de chimères ce texte oppose à un problème structurel des réponses parcellaires et ne permettra pas de résoudre les graves difficultés auxquelles certains de vos territoires. Sont confrontés. La démographie des médecins ne va pas s'améliorer. Sitôt les professionnels de santé mettront plusieurs années avant de s'approprier de telles innovations et les patients pourront se sentir désorienté. Malgré ces vents contraires, la commission a examiné ce texte en retenant une approche équilibrée consistant à adopter des mesures les mieux à même de fluidifier le parcours du patient et de valoriser les compétences des professionnels de santé. Elle a au contraire amender le texte lorsque cela paraissait nécessaire pour garantir la sécurité des soins comme pour conserver le rôle central du médecin dans la coordination et de suivi des patients. Le 1er volet de ce texte, sans doute le plus conflictuel concerne l'accès Direct à 3 profession paramédical exerçant aujourd'hui sur prescription médicale préalable. Les infirmiers en pratique avancée, les masseurs kinésithérapeutes et les orthophonistes. L'article premier entend revaloriser la profession d'infirmier en pratique avancée en améliorant les conditions dans lesquelles celle-ci peut prendre en charge des patients. Pour cela il autorise SIPA à prescrire des prestations et produits de santé a prescription médicale obligatoire. Il permet surtout l'accès Direct aux infirmiers en pratique avancée dès lors que ceux-ci exercent à l'hôpital en établissement médico-social ou en ville, au sein d'une structure. Et il a sorti cette autorisation de conditions permettant d'assurer l'information du médecin traitant. Les infirmiers en pratique avancée bénéficient d'une formation de 2 ans supplémentaires et de compétences élargies dans l'un des 5 domaines d'intervention aujourd'hui reconnu. Ils apportent à l'hôpital comme en ambulatoire, un appui précieux aux équipes de soins autorisé en 2018, la pratique avancée d'connu jusque-là qu'un des développements limités. La France de côté l'été dernier qu'environ 1700 IPA et moins de 200, exerçait en libéral. Le nombre insuffisant de patients confiée par les médecins constitue l'un des obstacles au déploiement des infirmiers en pratique avancée des plus souvent mise en avant. Compte tenu de ses effectifs et, contrairement à l'ambition affichée les dispositions du texte ne résoudront donc rien à court terme des difficultés d'accès aux soins dans nos territoires, elles contribueront toutefois à renforcer l'attractivité et la reconnaissance de la pratique avancée. C'est pourquoi la commission les a adopté tout en veillant à ce que l'accès Direct s'exerce en étroite coordination avec les autres professionnels de santé en le réservant en ville aux structures les plus intégrés, qui partagent une passion telle commune. L'article premier il également restructuré la profession en créant 2 catégories d'infirmiers en pratique avancée spécialisé et praticiens, ces dispositions n'étant pas adapté au modèle français pratique avancée infirmières et les organisations d'infirmiers en pratique avancée elles-mêmes y étant opposés. La commission a choisi de les supprimer. Les articles 2 et 3, Vista permettre également aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes d'exercer sans prescription médicale préalable dans les mêmes conditions que pour les infirmiers en pratique avancée là encore la commission adopter ces dispositions susceptibles de simplifier le parcours de soins tout en veillant à mieux encadrer l'accès Direct pour le réserver aux structures les mieux intégrés et assurer la sécurité des soins. Un second volet de la proposition de loi vise à étendre les compétences des professionnels de santé. Ainsi l'article 1er bis autorisé infirmier à prendre en charge la prévention, le traitement de plaies y compris par la prescription d'examens complémentaires et de produits de santé défini. L'article 2 bis autorise les masseurs kinésithérapeutes à prescrire une acté une activité physique adaptée. La Commission à adapter à adopter ces dispositions, en précisant toutefois que la Haute Autorité de Santé devrait se prononcer sur leurs conditions de mise en oeuvre. L'article 4 entend confier de nouvelles compétences à des assistants dentaires dit de niveau de. Leur mission, qui aujourd'hui sont circonscrites à de la pure assistance du praticien serait étendu à une contribution active aux actes d'imagerie à visée diagnostic aux actes prophylactique aux actes orthodontiques et à des soins post-chirurgicaux. La commission a complété le dispositif en conditionnant l'exercice de ses nouvelles activités à la validation par l'assistante dentaire d'une formation spécifique. L'article 4 bis encadre le nombre d'assistants dentaires de niveau 2 en le limitant aux nombres de chirurgien dentiste, là encore, la commission a adopté l'article en précisant son dispositif afin de prévenir les risques de contournement de la règle. Ce ratio s'appliquera ainsi sur un même site d'exercice de l'art dentaire et au regard du nombre de chirurgiens dentistes effectivement présents. D'autres articles élargit ses compétences reconnues à certains professionnels de santé sans profondes modification. La commission a adopté les articles 4, qui est-ce qui élargit les compétences et pédicure podologue afin de fluidifier le parcours de soins des patients et d'éviter les retards de prise en charge du risque posologique pour des patients diabétiques. Elle a également adopté l'article IV qui est-ce qui élargit sous certaines conditions la compétence reconnue aux opticien lunetier d'adapter la prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact. La commission a en outre soutenu l'article 4 nièce qui permet aux professionnels de l'appareillage d'adapter de renouveler des prescriptions d'orthèse plantaire. En fin d'article 4, terre des siestes autorise à titre expérimental, les pharmaciens biologistes a pratiqué des prélèvements servi co-vaginaux pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous avons soutenu cet article en commission. Je regrette simplement que le gouvernement ne Périnne n'est-ce pas cette reconnaissance législative d'une compétence que les pharmaciens biologistes détiennent et qui permettrait de renforcer les efforts dans la prévention de ce cancer. Une 3ème partie de la proposition de loi concerne l'organisation du parcours de soin. L'article IV terre vise à permettre aux sages-femmes aux chirurgiens-dentistes aux infirmiers de concourir à la permanence de soins ambulatoires. Si ces dispositions sont souhaitables pour améliorer l'accès aux soins non programmés pendant les heures de fermeture des cabinets. La Commission a toutefois souhaité supprimer la notion de responsabilité collective imprécis juridiquement et qui inquiétait les professionnels impliqués. Elle a également supprimé l'article IV quater, qui visait à valoriser l'engagement territorial des médecins. La commission a jugé ces dispositions inutile dans la mesure où les partenaires conventionnels sont déjà en mesure de rémunérer l'implication du médecin dans l'amélioration de l'accès aux soins. Elles ont été faire et de plus avec les négociations en cours qui prévoit déjà la mise en place d'un tel contrat. En revanche et pour rendre du temps médical utile aux médecin. La commission a adopté un nouvel article 3 bis visant à lutter contres les rendez-vous médicaux non honorés cet article confie à la convention médicale le soin de déterminer une indemnisation du médecin à qui un patient fait faux bond sans raison légitime cette indemnisation serait mise à la charge du patient responsable de responsabiliser les assurés sociaux. Enfin 2 articles concernent le statut de certaines professions et leurs conditions d'exercice. L'article IV sex IS modifie les conditions de qualification permettant l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et pharmacies hospitalières afin de permettre aux étudiants du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, récemment créée de pouvoir exercer leur profession. Une fois diplômé. La commission a soutenu cet article, de même que l'article 4 des siestes qui vise à reconnaître les assistants de régulation médicale comme professionnel de santé. Ce nouveau statut. Devrait contribuer à améliorer l'attractivité d'une profession concentrant d'importants besoins de recrutement. Vous le voyez mes chers collègues, la commission s'est efforcé d'aborder le texte de manière pragmatique, elle a retenu les mesures qui apporte des améliorations attendues sur le terrain par les professionnels et mais a prévu a prévenu par un meilleur encadrement de certaines dispositions. Toute désorganisation du système de santé. La commission vous invite à adopter son texte issu de ces travaux. Merci madame la rapporteure et maintenant la parole dans la suite de la discussion générale est à madame Mélanie Vogel. Pour le groupe écologiste pour cinq minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues, nous n'avons bien identifié ici et je crois depuis bien longtemps notre système de santé est entré dans une phase qui a dépassé depuis un bon moment le stade de la crise. Un stade de réel effondrement que nous mais une trompe des décennies si tenté que nous ayons la meilleure volonté politique du monde et que nos décisions des investissements nécessaires à dépasser l'enchaînement en effet des décisions politiques à courte vue articulé autour d'une idéologie qui consiste à considérer que les services publics doivent coûter le moins cher possible à court terme que le privé le marché sont par nature plus efficace et qu'il faudrait marchandiser les soins à rentabiliser la santé a eu raison de la force de nos services publics et conditions de travail des personnels de santé se sont ainsi fortement dégradé accélérant d'autant plus cet effondrement tendent entre eux renonce et partent quand trop peu arrivent et ceux qui restent sont en proie à l'épuisement. Hé oh terrible sentiment d'impuissance face aux conséquences désastreuses pour leur vie et surtout pour cette des patients et des patientes que les politiques que nous avons menées jusqu'ici mettent en danger. Dans ce contexte revaloriser ces métiers est en effet l'une des batailles à mener, en permettant l'accès Direct aux IPA ma soeur de kinésithérapeutes et orthophonistes dans le cas de structures d'exercice coordonné le texte élargit leurs responsabilités et peut contribuer à améliorer, d'une certaine manière l'accès aux soins, à l'heure, nous ne savons où 6 millions de Français dont 600.000 avec une affection de longue durée n'ont pas de médecin traitant et de façon réaliste ne peuvent malheureusement matériellement pas en pas en avoir un à court ou moyen terme. Mon groupe salue évidemment la montée en responsabilité de ces professionnels qui participent à la reconnaissance de leur qualification. Mais nous sommes cependant surpris que ces propositions ne soit pas accompagnée de la perspective d'une importante revalorisation salariale. Si l'idée de remplacer les infirmières sous-payés par des infirmières sous-payés avec plus de responsabilité, je ne suis pas sûr que nous allions bien loin dans la résolution du problème de la même manière, nous savons qu'une des clés pour améliorer réellement l'accès aux soins réside dans les effectifs. Investir dans nos services publics pour former davantage de personnel de santé et surtout construire un système de santé basé sur les besoins de la population. Hé bien plus important que de pouvoir avoir accès à des séances de kiné en Direct cet impératif d'investissement public doit se retrouver dans les décisions à venir. Sans quoi le type de loi que nous examinons aujourd'hui ne fera office que de rustine sur un navire déjà à moitié englouti. Nous, regrettant par ailleurs l'adoption en commission d'un dispositif de sanctions laissée à la discrétion de la convention médicale sans cadre légal très précis pour les rendez-vous non honorés. Bien sûr il faut honorer ses rendez-vous et bien sûr, d'autant plus dans un contexte de pénurie de médecins réserver un créneau sans se présenter pose tout un tas de problèmes, un problème pour le médecin privé de la consultation et pour les patients privés d'accès aux soins qui n'auront pas pu prendre ce rendez-vous. Néanmoins, soit on a inscrit un dispositif réellement juste qui ne s'applique qu'aux cas réellement illégitime. Ce qui n'est même pas explicitement prévu dans le texte et pour qui la sanction financière ne serait pas une charge disproportionnée et alors là, nous aurons un coup sur une usine à gaz. Soit nous nous exposons à la mise en place d'une double peine pour beaucoup de malades doublé d'un mécanisme à peu près inapplicable. Nous avons déjà du mal à trouver des créneaux pour payer pour être soignés. Évitons peut-être de faire payer les gens pour ne pas l'être. D'autant que l'on sait, statistiquement que pour tout un tas de raisons, c'est parmi les publics les plus précaires que l'on trouve le plus de rendez-vous non honorés. Encore une fois, je suis tout à fait conscient du problème de son ampleur et qu'il faille y remédier. Mais je veux croire que d'autres dispositifs que la sanction peuvent être retrouvés ou le non-, remboursement de soins ultérieurs auquel personne n'a intérêt. Enfin je voudrais dire un dernier mot sur la philosophie générale du texte illustré de manière assez transparente par son titre, proposition de loi portant améliorant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Bon, nous savons très bien que les problèmes d'accès aux soins dans notre pays. Non pas beaucoup à voir avec la confiance dans les professionnels de santé ni celle que les pouvoirs publics leurs portes ni celle que les patients, leurs portes le problème majeur d'accès aux soins dans le pays. C'est le désinvestissement public dans notre système de santé. Cela doit rester notre cap réinvestir dans les services publics revaloriser les rémunérations construire un système de santé basé sur les besoins qui donne toute sa place à la prévention. D'ici là et sur le texte que nous examinons aujourd'hui et au vu de son équilibre général le groupe écologiste s'abstiendra sur le texte. Merci cher collègue. Et je passe la parole à Xavier Iacovelli pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Les chiffres sont là, 1,6 millions de Français renoncent chaque année à des soins médicaux. 11% des Français de plus de 17 ans n'ont pas accès à un médecin traitant et 600.000 d'entre eux ont se sont atteints d'affections de longue durée. Ces derniers ont besoin de suivi et de soins pour éviter d'éventuelles complications et une fine une hospitalisation. Face à cette situation, il y a aussi une autre réalité des professionnels de santé ont compétences variées qui peuvent collaborer utilement ou encore de nouveaux accès à des formations de plus en plus complète avec par exemple le cas des infirmières en pratique. Avancée. C'est compte tenu de ces éléments que le texte déposé par notre collègue députée Stéphanie Rist vice-à améliorer l'accès aux soins par la confiance dans les professionnels de santé. prises, ont déjà été prises pour renforcer l'accès à ce soin. Je pense notamment à l'investissement massif dans notre système de soins de avec les 19 milliards d'euros investis à travers le Ségur. La suppression du numerus clausus la revalorisation alors de 180 à 400 euros par mois. L'augmentation des places ouvertes aux infirmiers, l'assouplissement des règles. Concernant le cumul emploi-retraite ou encore le renforcement du déploiement des assistants médicaux. Plusieurs dispositifs votés ont également été déjà visé à renforcer la coopération entre professionnels de santé concernant la vaccination pour les pharmaciens ou d'autres professionnels de santé par exemple. la Ministre budget de la santé a augmenté de 50 milliards d'euros. Il nous faut donc désormais aller plus loin sur le sujet et je crois que les CNR territoriaux source de multi-propositions pourront utilement servir à une réflexion globale pour l'amélioration de notre système de de santé et l'amélioration de l'accès aux soins à moyen et à long terme. Le texte soumis à notre examen représente une étape supplémentaire qui vient s'ajouter à ces mesures. Si le médecin traitant demeure le maillon central de notre organisation de santé, les soins quant à eux peuvent être délégués dans le respect du parcours de soin à d'autres professionnels de santé compétents. Comme son titre l'indique, cette proposition de loi nous invite donc à faire confiance. Faire confiance aux compétences de nos professionnels de santé, faire confiance à leur expérience. Il ne s'agit pas ici de se substituer aux médecins. Mais ce texte nous invite aussi à réfléchir plus largement à la revalorisation la coopération et l'organisation plus globale des professionnels de santé. Lutter contre les déserts médicaux, améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Valoriser les compétences acquises tout en assurant une organisation cohérente des soins. Voilà les objectifs de ce texte. Il n'a certes pas la prétention de régler tous les maux d'un système malade mais il contribue grandement à cette démarche de refondation. La simplification du parcours de soin est un vrai sujet pour les millions de Français. Nous devons aménager l'accès Direct, c'est-à-dire la possibilité pour un patient de consulter en première intention un professionnel de santé, autre que son médecin généraliste et ce dans le cadre d'un exercice coordonné. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de Madame la rapporteure Imbert et l'ensemble des contributions afférentes sur ce texte pour parvenir à cet équilibre. Le texte prévoit en son article 4 terre une organisation de la permanence des soins organisée sur chaque territoire avec leurs spécificités grâce à une collaboration efficace entre les professionnels de santé présent sur le terrain. Il nous paraît opportun de pouvoir associer les communautés professionnelles territoriales de santé de la même manière que les hordes des professionnels de santé concernés. De même, l'introduction d'un principe de responsabilité collective, de participation à la permanence des soins nous semble également pertinent. C'est pourquoi nous proposons de le rétablir par amendement. Laisser aux partenaires conventionnels. La définition des modalités de l'engagement territorial des médecins est aussi d'importance pour qu'il puisse en saisir. Cela afin de définir les mesures envisageables pour une, pour une juste reconnaissance et la valorisation des professionnels qui s'engagent en faveur de la coopération mais aussi au profit d'un accès aux soins de proximité aux soins non programmés, ayant des pratiques tarifaires maîtriser au bénéfice de la population de leur territoire et au-delà de leurs propres patients-t-elle. Enfin, mes chers collègues. Une problématique que nous ne pouvons ignorer tant le retour de terrain sont nombreux, celle des rendez-vous non honorés. Nous en comptons plus de 26, 27 millions chaque année ces rendez-vous non honorés représente une perte de temps médical précieux, surtout au sein de territoires sous dotés. Nous Salon l'le dispositif proposé par la Commission mais il ne veut pas apparaît comporter certaines limites. C'est pourquoi nous avons souhaité proposer une réécriture prévoyant la possibilité du recouvrement d'une pénalité financière d'un euro symbolique en cas de plusieurs rendez-vous non honorés par un même patient. Enfin, mes chers collègues j'aimerais également avoir un mot concernant. Les métiers de la santé de saluer l'engagement et leur dévouement de le dévouement de ces femmes et de ces hommes au service des autres. Comme je disais, notre système de santé est à bout de souffle. Il existe des situations professionnelles extrêmement compliqué mais il existe aussi de beaux parcours de belles expériences dans ce secteur de soins qui fait la fierté de notre pays. Il ne tient qu'à nous de poursuivre la dynamique enclenchée depuis maintenant plusieurs années pour mettre en avant ses parcours agir face à cette crise de vocation et surtout continuer à les écouter et à co-construire ensemble. Le système de soins de demain. C'est pourquoi le groupe RDPI votera favorablement à ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente madame la rapporteure, mes chers collègues. Madame la Ministre je crois que ce texte là à ce moment-là est une faute. Car, votre gouvernement fait le choix en accélérant la procédure parlementaire au lieu d'attendre la fin des négociations conventionnelles pour saisir notre assemblée il fait le choix d'ignorer le respect qui est dû aux acteurs intermédiaires. Le président du Sénat avait d'ailleurs souhaité que ce texte ne nous soit soumis qu'à l'issue des négociations conventionnelles, votre gouvernement a refusé ces deux mois de report. Mais c'est devenu une habitude depuis qu'Emmanuel Macron et chef de l'État et aujourd'hui le monde de la santé qui a besoin d'écoute, de sens de la négociation et du compromis et un peu plus en rupture avec votre gouvernement, du fait de votre inaptitude à respecter la démocratie sociale. Il y a 2 semaines, madame la Ministre, dans ce même hémicycle, vous avez repoussé sans discuter, sans volonté dialogue le texte sur les soignants à l'hôpital, soutenu par toutes les catégories de soignants hospitaliers et très largement approuvé par le Sénat. Aujourd'hui vous cristalliser des oppositions entre les professions de santé là où il faut plus de coopération car il s'agit bien de permettre à notre système de soins, de répondre aux besoins de santé de notre population qui sont en grande qui qui est en grande Madame la Ministre, comment espérez-vous après avoir jeté toute cette huile sur le feu et en avoir mis si peu dans les rouages y reviendrez parvenir à un accord sur de nouvelles répartitions de mission entre les professionnels de santé. Car la difficulté elle débute quand vous commencez par poser un cadre par trop restrictif. Évidemment avec un Ondam hospitalier à 4% c'est un message négatif qui a été envoyé, alors que l'inflation est à six, nous l'avions dit haut et fort lors de la discussion du PLFSS et lors de cette même discussion nous avions pointé le fait que pour l'Ondam de ville. L'évolution à 2,9% étaient moitié inférieure à la hausse de l'inflation. Comment voulez-vous dans deux quel telle condition. Avoir du grain à moudre pour les discussions. Le résultat c'est que vous attribuez des centimes de revalorisation kiné. Et qu'ils ont dénoncé l'avenant numéro 7 de leur convention. Et aux médecins. Vous promettez des revalorisations également centimes alors que l'acte n'a pas été revalorisée depuis 2017 et que la convention courra pour 4 à 5 ans, donc une revalorisation qui portera sur plus de 10 années. Ils ont donc unanimement et tous syndicats confondus y compris les plus modérés claqué la porte des négociations. Je ne peux que constater que la recherche avec d'un accord avec les syndicats réformistes n'est pas toujours la ligne du gouvernement, c'est un euphémisme. Alors, votre projet est-il de demander aux soignants de maintenir leurs revenus en multipliant les actes. Eh bien c'est ce qu'a exprimé ce matin encore le directeur de la CNAM. En demandant aux médecins de voir plus de patients, alors qu'ils sont déjà surchargés. Il faudrait donc travailler plus pour gagner, pas plus. Est-ce que demain les infirmières de villes devront elles devront pardon maintenir leurs revenus en réduisant le temps des toilettes les kinés passé moins de temps avec leurs patients, les médecins se résoudre à des consultations toujours plus courtes ou le temps de la prévention disparaît. Nous ne pouvons pas répondre à la pénurie par la désorganisation des parcours de soins par la multiplication des actes. Dans ce contexte dégradé l'utilisation de la voie parlementaire pour imposer de nouveau partage de tâches et voué à l'échec. Alors non pas l'échec législatif un texte peut bien sûr être adopté mais un échec sur le terrain. Un échec dans l'application par des professionnels qu'on aura opposé au lieu de les rassembler. Alors que sur le fond. Oui bien sûr, de nouveau partage de tâches sont nécessaires, nous le soutenons et pas uniquement d'ailleurs pour répondre à la pénurie de médecins mais parce que notre système de santé ne reconnaît pas suffisamment et ne valorise pas assez les compétences des pro des différentes professions qui le composent. Je veux rappeler à cette tribune que depuis 5 ans. Mon groupe dépose des amendements pour mieux valoriser la profession infirmière texte après texte et que si cet hémicycle a souvent adopté nos propositions vos deux prédécesseurs s'sont systématiquement opposés. Au gouvernement, aux législateurs appartient à la responsabilité de fixer les principes et pour nous c'est partage de tâches doivent respecter la nécessité d'un haut niveau de compétence du professionnel en charge d'une mission et l'inscription dans un parcours de soins. Charge aux organisations professionnelles d'avancer par la négociation, aidés par un 4 tarifaire soutenant réformer l'organisation des soins de ville implique l'adhésion des professionnels concernés et je sais, je constate que dans chaque profession, médecins, kinés, infirmières, sages-femmes beaucoup, ils sont prêts. Laisser l'heure madame la ministre, un peu de temps car, quelles que soient les réelles importantes améliorations apportées au texte par la commission des affaires sociales, sur proposition de sa rapporteure dont je salue la qualité du travail mieux légiférer, c'est aussi savoir qu'on ne doit pas légiférer, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. hein. Chers collègues et je vais maintenant passer la parole à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, je salue le travail de notre rapporteure Corinne Imbert qui a tenté de repêcher une proposition de loi bien insatisfaisante. On a tendance à dire que très souvent les suites de films sont moins bonnes que la première version n'étions pas satisfait de la première PPL risque et je dois dire que cette 2ème saison n'est pas plus convaincante. Tout d'abord sur la forme cette PPL est en réalité une fois de plus un projet de loi déguisée du gouvernement. C'est pour cela que je m'adresserai direct vaguement à vous Madame la Ministre lors de cette intervention. D'autant que vous avez fait adopter plusieurs amendements sur des sujets majeurs et ce sans un, sans étude d'impact sans concertation. Nous avons donc à nouveau l'impression d'une loi fourre-tout de réorganisation de notre système de santé, mais sans vision d'ensemble, sans réelle ambition depuis 2017, ne compte plus le nombre de propositions de loi sur la santé censé régler un aspect du problème et six ans plus tard, la situation est toujours la même près d'un quart des Françaises et des Français vivent dans un désert médical beaucoup renoncent aux soins 13 départements non pas de gynécologue médical de nombreux patients non plus de suivi psychiatrique et je pourrais hélas poursuivent cette triste litanie votre pseudo réforme du numerus clausus ne produira aucun effet sur la pénurie des professionnels et sur le développement des déserts médicaux, les mesures du Ségur n'ont eu également aucun effet sur l'amélioration des conditions de travail des personnels et vos gestion de la pénurie aujourd'hui se transforme en discours pour soi-disant libérer du temps médical et mieux articuler les compétences des professionnels de santé. Pour notre part nous sommes favorables à une revalorisation des missions et des professions notamment paramédical une reconnaissance de leurs compétences mais cela ne peut être uniquement pour pallier le manque de médecins, vous devez être guidé par un haut niveau d'ambition pour notre système de santé, une vision globale et cohérente et surtout anticiper anticiper au lieu de réagir au coup par coup. Le PLFSS 2022 a proposé une expérimentation pour autoriser la primo-prescription pour les IPA et celui de 2023, une expérimentation pour l'accès Direct nous avions soutenu ces dispositions, mais quelques mois plus tard, alors même que cette expérimentation n'a pas eu lieu. Vous nous proposez la généralisation de ces dispositifs. Il ne s'agit pas ici de défiance de notre part à l'égard de ces professionnels mais de bien comprendre les raisons de cette accélération, madame la Ministre reconnaissait enfin que les politiques de restriction budgétaire n'ont fait qu'affaiblir notre système de santé publique et que nous sommes proches de la rupture, madame la Ministre travailler enfin à une loi sur la santé digne de ce nom en prenant en compte les revendications, les aspirations, les besoins des professionnels comme des patients, voilà l'urgence ce n'est pas du tout le chemin que vous empruntez sans même atteindre la fin des négociations conventionnelles, vous mettez à l'ordre du jour du Parlement cette PPL qui n'a fait qu'enfler au fur et à mesure des différentes lectures les conséquences sont immédiates, arrêt des négociations opposition des différentes professions médicales et paramédicales entre elles là où il faudrait plus que jamais coordination et complémentarité même les mesures qui pourraient améliorer les prises en charge des patients sont réduites dans leur portée ainsi que ce soit pour les IPA ou les orthophonistes l'accès Direct telle qu'il est envisagé et plus que restrictif puisqu'il serait uniquement autorisée dans les structures d'exercice coordonné. Il y a là une méconnaissance totale non seulement du territoire mais également des professions concernées ainsi avec cette rédaction, seule une toute petite minorité pour ne pas dire quasi aucune orthophoniste ne sera concerné, raison pour laquelle nous avions proposé plusieurs amendements pour cette profession, malheureusement, un seul a été jugée recevable. En résumé, avec cette PPL les Françaises et les Français auront toujours autant de difficultés à se faire soigner et ce ne sont pas les dispositions de l'article 4 terre sur la permanence des soins et l'élargissement de cette mission de service public à d'autres professions qui réglera le problème puisque vous ne revenait pas sur l'obligation de garde, le parcours de soins qui fait du médecin traitant le point d'entrée des patients ne peut être détricoté sans réflexion globale et cohérente pour trouver des solutions immédiates face aux 6 millions de Françaises et Français qui n'ont pas de maintien généraliste. Une nouvelle fois écouter nos propositions en investissant massivement dans notre système de sécurité sociale pour augmenter les capacités de formation des professionnels de santé et améliorer l'attractivité des carrières, tout en donnant aux universités, les moyens d'accueillir plus d'étudiants réorganiser notre système de santé en partant des besoins des usagers en maintenant les structures d'accès aux soins de proximité et en revoyant la gouvernance des hôpitaux pour une véritable démocratie sanitaire confier aux autres professionnels de santé, une mission en termes d'orientation du patient dans le système de santé en assurant une première prise en charge et en organisant avec les autres acteurs du territoire l'orientation vers un médecin traitant comme cela se fait dans les centres de santé en attendant Madame la Ministre, mes chers collègues, nous nous abstiendrons sur cette PPL qui est une fois de plus une occasion mens mentis et d'améliorer l'accès aux soins. Je vous remercie. Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à Élisabeth Doineau pour le groupe Union centriste pour huit minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues. 2 ans nous séparent de l'examen de la première loi risque au Sénat. Celle-ci était hospitalo-centrée et déjà elle avait suscité une avalanche de réactions, rappelez-vous. Aujourd'hui, la 2ème, proposition de loi de madame Stéphanie Rist concerne la médecine de ville. On ne peut pas dire aujourd'hui comme hier, que ces initiatives remporte l'adhésion des professionnels. C'est même tout le contraire. Les médecins sont en grève, ils sont dans la rue. Je donc par 2 observations. La première observation, c'est la question de la temporalité et mes collègues. L'ont déjà. Dit. Est-ce bien judicieux de choisir le temps des négociations conventionnelles pour réorganiser le système d'accès aux soins. Est-ce bien raisonnable de jeter de l'huile sur le feu et je crois que tu l'as dit. Bernard dans cette période privilégiée pour fixer avec la CNAM. Les tarifs les forfaits les bonifications liées au prix des actes et des consultations. Deuxième observation le choix du véhicule législatif. Pourquoi choisir l'initiative parlementaire en 2 temps qui désolidarisent l'hôpital et la médecine de ville alors que ces 2 sujets sont intimement liés. Pourquoi alors que le gouvernement soutient ces dispositions ne pas avoir construit un projet de loi cohérents et surtout enrichi d'une étude d'impact. C'était mes 2 observations. Je poursuis avec 2 obligations. La première, c'est d'assurer un accès à des soins de qualité à tous les Français. Nos concitoyens nos élus nous presse de trouver des solutions pour répondre à la faiblesse de la démographie médicale. Je comprends parfaitement l'exaspération des uns et des autres, mais doit-on y répondre sans l'adhésion des professionnels. Je ne le pense pas. Je pense au contraire qu'il faut absolument rétablir la confiance et la confiance comme c'est toujours dit ne se décrète pas, elle se construit. Or les médecins pour ne parler que de en ce jour de grève n'en peuvent plus. Le climat est devenu délétère au fil du temps. Mesures de régulation PPL de mesures de régulation PPL permanence de soins obligatoires pépé l'installation en zone sous-dense dixième année de médecine générale. On peut donc. Défendre l'objectif d'une offre de santé pour tous. Mais on doit aussi préserver nos médecins. Maltraités les soignants c'est maltraité les patients. Et je crois qu'il faut ramener la confiance et la sérénité. Les PPL qui traverse le temps législatif comme les ballons chinois traversent le ciel américain. Ils n'en peuvent plus. C'est insupportable et tout cela à de fortes conséquences pour la médecine générale. Je ne vous dis pas, combien de médecins. J'ai rencontré. Combien de futurs médecins j'ai rencontré. Combien de futurs étudiants en médecine m'ont exprimé leur désarroi et leur désaffection pour cette spécialité prenons-y garde. La 2ème obligation. Étant de reconnaître la montée en compétence d'autres professionnels de santé. J'ai toujours. Lors des Plfss tenté de proposer des amendements dans ce sens. Sans doute que le temps n'était pas venu. La première mars s'est d'ailleurs matérialisée à l'Automne dernier par les annonces du Clio. Je voudrais rappeler à mes collègues ce que, ce qu'est le Clio c'est le comité de liaison des institution ordinale et les différents ordres s'étaient mis d'accord. Pour agir sur la pluridisciplinarité sur la coordination des soins, la valorisation des compétences et l'amélioration de la lisibilité du système. Il me semblait que c'était une première marche qui était à saluer et que nous devions poursuivre justement et c'est sans doute l'opportunité de cette PPL que nous examinons aujourd'hui. Et il donc. À mon sens. Nécessaire de reconnaître que ces PPL a des raisons d'être voté pour justement ouvrir à de nouvelles professions des responsabilités. Mais comme je l'ai dit il faut se rappeler les observations et les obligations que nous avons parce que. Ces professionnels ont effectivement acquis en compétences, soit par des. Formation adaptée pour les infirmières en pratique avancée mais c'est aussi d'ailleurs le cas des infirmières. De bloc opératoire pour les infirmières. En en anesthésie. Pour les infirmières puéricultrices. Nous devons regarder combien elles ont acquis en compétences et c'est aussi le cas d'autres professionnels de santé de paramédicaux qui sont devenus. Dans des équipes pluridisciplinaires dans des équipes de soins primaires des éléments importants, donc nous devons tenir compte de cette montée en compétences. J'en viens aux dispositions prévues par la proposition de loi et je salue et je fais mienne l'approche équilibrée de Madame la rapporteure Corinne Imbert aussi je ne m'étendrai pas trop longuement sur le détail des articles dans un 1er temps, elle ouvre l'accès Direct aux infirmiers en pratique avancée aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes j'y suis favorable, la profession d'IPA n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il convient de faciliter son essor en étendant ses compétences et en en lui assurant un cadre sécurisant même ne nous leurrons pas, il y a pas énormément d'infirmières en pratique avancée en libéral, et donc on ne va pas du jour au lendemain. Atteindre des capacités en en accès aux soins supplémentaires. L'article 2 relatif aux kinésithérapeutes lors des différences examen du texte le nombre maximal de séance accessible sans diagnostic médical préalable a fluctué entre 10 puis 5 ici. Mais moi je m'interroge, est-ce vraiment au législateur de le définir. Est-ce vraiment à nous Par ailleurs, en concertation avec Madame Corinne Imbert. J'ai proposé un amendement visant à lutter contres les rendez-vous médicaux non honorés afin de regagner du temps médical. Moi je trouve inacceptable que certains prennent des rendez-vous et qu'il ne les honore pas au détriment de ceux qui en ont besoin et qu'ils n'en obtiennent pas son objet, et de confier à la convention médicale le soin de déterminer une indemnisation du médecin à qui impatient fait faux bond sans raison légitime. Je soutiendrai un amendement de la rapporteure pour étendre finalement ça à l'ensemble des professionnels de santé parce que évidemment on a pensé au médecin parce que c'était eux, surtout qu'ils nous ont dit que c'était un levier important qu'il fallait prendre en compte, mais je pense que dans d'autres professions médicales, il y a aussi des rendez-vous qui ne sont pas honorés. Donc cette indemnisation serait mise à la charge du patient responsable. Afin de responsabiliser les assurés sociaux. L'pam pourra par exemple déduire la somme des remboursements ultérieure verser aux patients. Mais même si ces amendements ne sont pas adoptés par le 11 ans il est nécessaire d'en parler aujourd'hui. Nous connaissons tous les difficultés rencontrées par les familles, pour accéder aussi un orthophoniste. Cependant, on sait qu'ils sont aussi en nombre insuffisant pour répondre à la demande mais essayons de faciliter justement leur accès en évitant de passer par le médecin traitant parfois lorsqu'ils sont vus par exemple par le médecin de la protection maternelle et infantile. Bon. Je je je reviens pas sur les autres articles parce que je suis totalement la vie de de la rapporteure. Mais pour conclure, je voudrais dire que cette proposition des de loi crée des tensions au sein et entre certaines professions de santé. Cela est regrettable. Alors que nous avons besoin de la pleine mobilisation de chacun dans cette lutte pour l'accès aux soins. Je me rapporte à une réflexion. De Jean-François Deniau, qui disait que faire dans la confusion et l'inquiétude. Dire ce que l'on croit. Or moi ce que je crois c'est qu'il y a le CNR, santé, nous n'avons pas encore les conclusions qu'il y a je dirais les 12 travaux du ministre de la Santé qui l'a annoncé. À la fin du mois de janvier j'en attends beaucoup et je pense qu'il faut se recentrer sur ces 2 éléments qui sont importants parce que sinon du même auteur, on dira dans le méli-mélo. J'ai toujours préféré le Mali et c'est dommage de ne pas choisir l'ensemble. Merci. Merci. Donc en l'absence en l'absence de monsieur Ravier je vais passer tout de suite la parole. À Madame Véronique Guillotin pour le groupe RDSE.

monsieur le Président la Ministre madame la présidente de commission madame la rapporteure, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une nouvelle proposition de loi dont l'objectif affiché est d'améliorer l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Souvenons-nous de la crise Covid. De l'extrême agilité des professionnels à s'organiser. À travailler ensemble comme jamais auparavant. Ils ont relevé des défis incroyables et nous avons tous salué cette nouvelle façon de faire. Nous avons tous dit que nous en tirerions les leçons et qu'il fallait laisser le terrain s'organiser. Mais l'examen de cette PPL prend une toute autre tournure. Elle intervient alors que les négociations conventionnelles ne sont pas terminées que les conclusions du Conseil national de la refondation ne sont pas rendus. Que l'expérimentation de l'accès Direct aux infirmiers en pratique avancée commence à peine et déjà se termine. La Concorde entre professionnels de santé s'est transformée en défiance. On voit les uns s'opposer aux autres et quelquefois de manière un peu fleuri. La colère et l'inquiétude sont grandes chez les médecins qui y voient un risque de désorganisation et de dégradation des soins les professions paramédicales, elle l'accueille avec satisfaction. Pour avoir beaucoup échangé avec les professionnels de santé ces derniers jours encore plus. Tous s'accordent à dire que la montée en compétence les partage de tâches sont une bonne chose d'ailleurs, je crois qu'ils sont nombreux à avoir entamé le virage de ces nouvelles pratiques. Alors quel est le point crispant. C'est principalement l'accès Direct et le sentiment de dévalorisation qui inquiète et fait monter la colère dans la profession médicale ce serait je pense une erreur de réduire cette colère à une simple réaction de corporatisme. Si je vois dans les monter en compétences des métiers un levier d'amélioration de la prise en charge des patients. Également un facteur d'attractivité des métiers je ne l'envisage que dans un cadre coordonné autour du médecin traitant qui est et qui doit rester le pivot de la prise en charge. C'est pourquoi, avant de légiférer à nouveau. J'aurais préféré que l'expérimentation de l'accès Direct aux IPA aille à son terme et nous permettent d'évaluer la mesure avant de l'étendre de manière définitive. Je tiens à saluer très sincèrement le travail pas facile de la commission et de sa rapporteure Corinne Imbert de manière pragmatique et équilibrée, elle renforce l'encadrement de l'accès Direct aux professions paramédicales afin d'Ali, accès aux soins et sécurité du patient. La suppression de la notion d'IPA praticienne et spécialisée va dans le bon sens ainsi que réserver l'accès Direct aux IPA aux structures de proximité que sont les équipes de soins primaires et les maisons de santé concernant l'accès Direct au kiné l'autorisées dans la limite de 5 séances comme la commission l'a proposé, me paraît acceptable À titre personnel moins favorable à la prescription de l'activité physique adaptée par les kinés qui demande un examen plus globale du patient. La création d'un assistant dentaire de niveau 2 est une bonne chose, tout comme la prise en charge par les infirmières déplaît allant de la prévention à la réalisation d'examens complémentaires sur les rendez-vous non honorés. Je partage l'ambition de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques. Que inacceptable qui pénalisent tout le monde. Il est urgent de responsabiliser les patients, afin de libérer des créneaux pour ceux qui en ont vraiment besoin mais je doute du caractère opérationnel de l'amendement adopté en commission qui me semble être sources de nombreux contentieux. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de rentrer plus dans les détails de cette PPL je m'exprimerai au, des cours de l'examen des amendements. Si la crise de notre système de soins nécessitent des réformes profondes et durables et je sais que c'est pas simple. Si le statu quo n'est pas possible, nous en sommes convaincus, notre groupe demeure vigilant quant à une potentielle désorganisation du parcours de soins, voire à une dégradation de ce dernier. Les médecins les professions paramédicales doivent travailler ensemble, de manière coordonnée, le médecin doit rester au puis le pivot de cette équipe. Gardons-nous de l'inflation de PPL qui n'apporte pas de réponse structurelle. L'urgence est de former des médecins de rendent l'exercice des professions de santé attractive de donner envie aux jeunes de s'installer, de répondre à une crise identitaire que traverse la médecine générale et pour cela il faut restaurer la confiance. Je formule le voeu qu'en ce jour de Saint-Valentin, nous parvenions à réunir tout le monde médicaux et paramédicaux autour d'un projet commun de refondation profonde de notre système de santé et nous devons le faire avec les professionnels et pas contre les professionnels, je vous remercie. Merci cher collègue. Et je vais maintenant passer la parole à la présidente Catherine Deroche. Les républicains. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues. Comme la rappeur les Corinne Imbert dans son rapport la question de la répartition des compétences entre les différentes professions de santé étaient déjà posée par le rapport du professeur Yvon Berland qui invité à redéfinir les missions des médecins avec le souci qu'il soit utilisé de manière optimale à leur juste niveau de formation. C'était il y a 20 ans en 2014 dans un rapport co-signé par Catherine Génisson notre collègue Alain Milon. Invité à ce nouveau partage des tâches. Alors que la formation des médecins s'allonger et que se renforçaient dans le même temps, celle des paramédicaux. Il y a donc bien une voie exploré dans laquelle notre pays s'engager plus tardivement et moins fortement que d'autres du fait de son histoire et probablement de l'expérience des officiers de santé passer à la postérité sous les traits. Peu flatté de Charles Bovary et du pied bot du malheureux Hippolyte. Pourtant, cette évolution est d'autant plus nécessaire que le temps médical se fait plus rare et que nous souhaitons parallèlement développer la coopération des professionnels de santé autour du patient. Je crois pouvoir dire que cet objectif plutôt consensuel. Et nous le voyons quotidiennement sur le terrain dans les les les ASP ou Les MSP qui sont sur notre territoire, mais ce qui l'est beaucoup moins c'est la façon très concrète dans cette coopération doit s'opérer. Les infirmiers de pratique avancée créé par la loi 2016 n'ont connu qu'un développement limité entravée par des textes réglementaires restrictif. Les expérimentations adopté dans différents projets de loi du financement de la Sécurité sociale n'ont pas été jugé suffisamment prioritaire pour se voir dotée d'un décret d'application. Plus récemment, l'annonce d'un accord intervenu dans le cadre d'un comité de liaison inter-ordres le Clio a rapidement fait place à un niveau de défiance très élevé entre les professions et à l'égard du gouvernement. Pour compliquer encore le dossier son calendrier est parallèle à celui des négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et les cinq Dukan médecin, ce dernier ayant quitté la table de négociation, le 20 janvier dernier. Voici le contexte dans lequel nous sommes appelés à légiférer. Un contexte devenue tendue dans lequel chaque partenaire prête à l'autre les intentions, les plus sombres. Tout en partageant l'objectif poursuivi. Je ne crois pas que la méthode soit adapté. Lorsqu'il s'agit notamment de pérenniser une expérimentation prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 dont l'encre est à peine sèche, mais aussi pour ajuster parfois de façon très pointilliste les compétences de telle ou telle professionnel cette matière réglementaire et l'intervention du législateur produit scène matière des résultats plus concluant. S à la loi de rentrer dans un tel niveau de détails, sans doute pas. Faut-il utiliser le débat parlementaire. Dans le cas de négociation conventionnelle. Je ne crois pas non plus. C'est pourquoi notre commission a supprimé les dispositions relatives à l'engagement territorial de médecins trop flou pour produire elles-mêmes des effets normatif sans s'est par ailleurs être traité par la voie conventionnelle et souvenons-nous de l'article 35, voter au PLFSS est de nature agiter eu inutilement un chiffon rouge dont il serait plus judicieux de se passer. Rappelons par ailleurs que notre système de santé abîmé par une crise structurelle et des professionnels confrontés à une perte de sens. Avec la rapporteure Corinne Imbert. Nous aurions préféré un report de ce texte, le temps qu'un nécessaire apaisement soit obtenu. Cela n'a pas été possible. nous invitons donc le Sénat à garder le cap d'un nécessaire partage de tâches à retrouver les conditions d'une nécessaire sérénité entre les professionnels et à sécuriser les questions et de responsabilité et de formation et c'est toujours l'intérêt du patient qui doit nous guider. Dans l'intérêt du patient. Nous invitons le gouvernement changer de méthode à utiliser prioritairement le levier conventionnelle puis à réinscrire ce texte dans un chantier plus large qui comprendrait notamment une refonte de l'ingénierie de formation des paramédicaux. Néanmoins, tout en exprimant un grand nombre de réserves, nous avons je pense trouver un équilibre fragile qu'il conviendra de préserver et je remercie notre rapporteur Corinne Imbert sur cet exercice d'équilibriste délicat mais néanmoins que je vous demande de voter parce qu'il nous semble important de préserver cet équilibre et je vous remercie de votre attention. Merci et je vais passer maintenant la parole à notre collègue Daniel Chassain pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente madame rapporteur. Améliorer l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, un titre qui sert un objectif ambitieux que nous partageons sans doute tous. Oui, l'accès aux soins date être renforcées dans notre pays dans lequel beaucoup de territoires sont considérés comme désert médical et dans lesquels 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Oui, il faut redonner du temps médical au médecin. Oui, il faut renforcer l'attractivité des métiers de santé et former davantage d'infirmières et DPA si nous partageons ce constat est l'objectif. Affiché de cette PPL les moyens pour y parvenir ne font en revanche pas l'unanimité et cette PPL a largement divisé au sein des professionnels de santé. Je remercie. Corinne Imbert rapporteure d'abord essayer d'améliorer. Ce projet. Le texte. Propose un élargissement des compétences de certaines professions de santé et l'accès Direct à trois d'entre elles, certains articles remettent en question l'organisation du parcours de soin du patient et nous devons être prudents, afin que réorganisation ne rime pas avec des organisations. L'article a notamment vise à autoriser l'accès Direct aux infirmières de pratique avancée les IPA. Devrait être aujourd'hui un un peu un appui précieux aux équipes de soins en assurant un suivi des patients chroniques qui leur sont confiées par le médecin. Permettant d'augmenter le temps médical de ce de ce dernier. Nous ne souhaitons pas remettre en cause les compétences ni la légitimité la légitimité des IPA. Elles sont une chance. Comme vous l'avez dit, Madame le ministre à condition qu'elle soit utilisée par délégation des médecins. Les IPA sont formés à la. Prise en soins des pathologies chroniques stabilisées, elle ne peut remplacer celle de médecins qui a bénéficié de 10 années d'études en sémiologie Physiologie Pathologie et d'une expérience de plusieurs années en internat dans les services hospitaliers, un médecin doit garder la compétence du diagnostic. Nous pensons que les médecins, et ils perdent médecin hyper doivent travailler ensemble en synergie et par délégation et ce afin de sécuriser tant la prise en charge du patient. Que l'activité de l'IPA elles-mêmes. Les travaux portant d'ailleurs sur les IPA dans d'autres pays montre. Des preuves d'efficacité uniquement lorsqu'il existe une collaboration réelle entre médecins traitants et infirmiers sur l'article de concernant les si nous pensons que les médecins donc. Conserver la prescription, nous avions déposé un amendement pour autoriser les kinés avec avis du médecin à renouveler des séances lorsque il y a des. Lorsqu'il l'exerce en Ephad. L'accès aux directes aux orthophonistes mérite d'être soutenu, compte tenu du type de prise en charge très ciblée de ces professionnels. Que sont amenés à faire les nouvelles compétences octroyées aux assistants médicaux dits de niveau 2. 2. Orthoprothésiste et aux aux opticiens semble représenter elle des solutions pratiques. C'est vrai. Dans l'article 1er relatives à la prise en charge par les infirmer, de la préservation et le traitement des plaies chroniques, il serait important de préciser que le renouvellement pourra se faire par l'IDE avec l'avis du médecin en effet Simply chronique ne guérit pas, cela peut signifier une mauvaise prise en charge par la non-détection ne trouble la Terre éthique ou d'une mauvaise contention effectué par une sur une insuffisance veineuse et dans ce cas, l'intervention du médecin est nécessaire concernant les pédicures podologues dans l'article 4. Elle bénéficie d'une consultation tous les trois mois par prescription pour les patients diabétiques effectivement que l'homme propose le texte, pourquoi pas l'autoriser un accès direct Si un patient diabétique, a besoin d'une consultation plus fréquentes qu'une fois par trimestre. Cela peut traduire en risque d'artérite et Anne assistions nécessité de consulter un médecin. La possibilité étendue de renouvellement d'une prescription par le pharmacien et je regrette coconne mais amendements élargissant ses compétences n'a été accepté et bien sûr je soutiens l'extension aux vaccinations des pharmaciens aux infirmières la place du médecin traitant doit rester central, tout simplement car c'est le professionnel qui détient aujourd'hui de par sa formation les meilleures compétences pour assurer la coordination du parcours de soin. Du patient, l'ensemble des amendements que j'ai proposé ou que je soutiendrai vont dans le sens pour les patients et pour sécuriser les para-médicaux Madame les milices. Nous devons je pense écouter davantage les médecins et les professionnels. Merci Merci la parole est maintenant à notre collègue Émilienne Myrhol pour le groupe socialiste pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la rapporteure Madame la Ministre madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une nouvelle proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans notre pays. Ce texte déposé par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale a été très largement amendé par le gouvernement puisque pas moins de 9 articles ont été rajoutés à la proposition de loi initial. Peut-être serait-il temps pour le gouvernement de nous proposer enfin le projet de grande loi santé que nous appelons de nos voeux dans cette assemblée et plusieurs de mes collègues l'ont évoqué. En préambule. De notre examen au niveau du sénat je tiens à remercier Madame la rapporteure Corinne Imbert pour son travail et son écoute des professionnels de santé. La commission a ainsi supprimer ou modifier des dispositions qui nous apparaissait comme favorisant la destruction du parcours de soin. Mesures telles que la création des infirmiers de pratique avancée praticienne dont on ne sait ce que recouvrait. Nous sommes également favorables à la suppression des CPTS parmi les structures autorisant l'accès Direct parce que ce n'est pas leur rôle ou à la réduction du nombre de séance un accès Direct chez un kinésithérapeute. Parmi les dispositions du texte. Nous soutenons la. La création de la provision d'assistant à Messine bucco-dentaire, cela a été évoqué tout à l'heure sur dans l'autre texte de la même façon. Nous saluons la reconnaissance de la captivité de professionnels de santé aux assistants de régulation médicale qui sont j'allais dire les au 1er maillon de la chaîne de secours. Néanmoins je tiens à rappeler l'attachement de notre groupe, du groupe sert pour le respect du groupe du parcours de soin et l'exercice coordonné de la médecine et son refus d'une médecine dégradé et à 2 vitesses si je regrette que la médecine coordonnées qui est, nous le savons bien l'avenir de l'exercice de la médecine et une partie de la réponse à la problématique de l'accès aux soins ne soit pas la question centrale de ce texte il traite toutes les professions de santé en silos article après article IPA qui naît orthophonistes podologues opticien orthoprothésiste et etc. Au lieu de repenser l'exercice collectif collaboratif de la médecine. Pourtant, seule une organisation centrée sur un partage des tâches et je dis bien un partage des tâches entre le médecin traitant et les autres professionnels de santé donc les infirmières de pratique avancée au travers de projets. Du Mans établi par l'ensemble de l'équipe traitante permettra de dégager du temps médical et ainsi favoriser l'accès aux soins pour l'ensemble de la population. Il s'agit d'ailleurs d'un souhait, ça a été rappelé de l'Ordre des médecins qui propose de le rendre obligatoire dès 2027 projets que nous avions repris à l'article 2 de notre proposition de loi visant à rétablir l'équité territoriale face aux déserts médicaux en décembre. Cette proposition de loi consacrent donc l'accès Direct des patients et la primo-prescription à différentes professions de santé et à ce titre, nous saluons la possibilité de l'accès Direct au kiné ou aux orthophonistes formés au diagnostic. De plus si nous soutenons le développement du rôle des IPA. Celui-ci n'a effectivement de sens que dans le cas d'un exercice coordonné telle que nous commencions d'équipes de soins primaires, une maison de santé pluri-professionnel ou un centre de santé afin de développer la présence des IPA et multiplié les IPA sur notre territoire, il est indispensable de renforcer non seulement leur formation mais surtout de mettre en place des aides financières pour les soutenir face au cou et au sacrifice que représente cette formation de deux ans. Enfin, juste un petit point particulier sur l'article 3 bis. L'idée développée dans le texte selon le la laquelle il suffirait de sanctionner les patients. Qui ne se présente pas le rendez vous pour gagner du temps médical nous apparaît comme simpliste et inefficace. Aussi, malgré quelques mesures qui vont dans le bon sens. Le groupe socialiste s'abstiendra il ne votera pas en faveur de ce texte a en effet face au moyen et au manque surtout de moyens accordés à la santé de façon générale au non respect du processus de négociation des conventions médicales. Cela a été évoqué par plusieurs de nos collègues et surtout l'absence de vision d'ensemble de cohérence et je dirais d'ambition, de l'accès à la santé en France. Donc, notre groupe socialiste s'abstiendra. Merci cher collègue. Et je vais maintenant passer la parole à Florence Lassaad. Groupe les républicains. Pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Face à la désertification médicale insuffisance d'offre de soins. Cette proposition de loi cherche à renouveler notre façon d'aborder la prise en charge médicale. L'esprit de ce texte et de favoriser l'accès aux soins pour nos concitoyens. Nous ne pouvons que partager cet objectif tout en nous interrogeant sur les modalités et les choix qui sont mis en oeuvre par le gouvernement et sa majorité. Il y a bien urgence car, comme l'on dit, mes prédécesseurs, 6 millions de Français sont aujourd'hui dépourvues de masse en traitant et parmi eux, 600.000 patients atteints d'affections de longue durée, alors que leur maladie chronique exige prévention dépistage et soins. Cette absence de médecins traitants engendre des complications des hospitalisations. Ce qui est très grave. Cette proposition de loi cherche à pallier ces difficultés en ouvrant l'accès Direct et en élargissant les compétences de plusieurs professionnels de santé. L'objectif est de permettre de fluidifier le parcours de soin du patient et de libérer du temps médical. Ce texte donne la possibilité aux patients de consulter en première intention un professionnel de santé sans devoir passer par un médecin 3 professions principalement concernés par cet accès Direct. Les infirmiers en pratique avancée, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes. Il propose ensuite d'étendre le Champ des compétences des IPA à la prescription de produits de santé et de prestations et de prestations soumises en principe à des prescriptions médicales obligatoires n'eut-il pas été préférable d'attendre la fin de cette expérimentation pour envisager cette extension. Ce texte ne précise d'ailleurs pas les conditions d'exercice et les protocoles de prise en charge. Comment concrètement se fait cette ouverture. Il ne s'agit pas de contester les compétences et IPA. Mais je voudrais partager mes inquiétudes en ma qualité de médecin qui existé de longues années en milieu hospitalier et en libéral. Je m'interroge pour savoir jusqu'où les IPA et les masseurs kinésithérapeutes pourront aller avant de pratiquer la médecine. Et par conséquent, comment pouvons-nous déterminer leur responsabilité en cas d'erreur médicale qui endossera la responsabilité d'un acte qui aura été mal effectués. Est ce que les médecins devront endosser les responsabilités des actes réalisés en 1er recours par les IPA. Vous évoquez une responsabilité collective. Mais comment cela se traduira-t-il juridiquement. Ce n'est pas clair du tout. Il convient d'encadrer formellement ce dispositif et j'aurais aimé que nous puissions être éclairé sur cet aspect avant de voter le texte. Je poursuis les IPA pourront donc intervenir en premier sur des pathologies courantes et bénigne mais pour affirmer que c'est bénin. Il faut poser un diagnostic et donc intervenir comme un médecin la dignité apparente peut aussi parfois cacher une pathologie grave. Madame la Ministre. Il faut également entendre les médecins sur ces évolutions du système de santé. En premier le jeu mais en 1er lieu je m'étonne que l'examen de ce texte coïncide avec les négociations sur la revalorisation du tarif de la consultation. Cette revalorisation est d'autant plus nécessaire que l'inflation est importante. Or la seule. La seule revalorisation tarifaire proposé et de 1 euros 50 de l'acte de base. Cela ne rattrape même pas l'inflation liée au blocage des honoraires depuis 2016. C'est inacceptable de surcroît aucune valorisation financière n'est prévue dans le texte car il est impossible de créer une charge pour les finances publiques dans une proposition de loi. Ainsi la revalorisation des actes restent encore dans les. Sans Sans exclure la nécessité de mieux considérer les propos les professions paramédicales, je considère que le médecin doit rester au coeur du notre système de santé. Je vous rappelle que 10 à 15 années sont nécessaires pour former un médecin à faire de lui permettent de poser des diagnostics, d'éliminer des diagnostics différentiels et de donner la bonne indication au bon moment. Les infirmiers font les soins pour lesquels ils ont été formés. C'est très différent et les formations sont différentes, nous sommes complémentaires. Mais pas substituables les soins peuvent être partagés avec d'autres professionnels de santé, à condition de travailler en coordination avec les médecins. Enfin, cette proposition de loi mais bel et bien en oeuvre une santé à 2 vitesses, il aura ceux de nos concitoyens qui auront un médecin. Et ceux qui auront accès à des non-médecins pour établir un diagnostic et prescrire un traitement. C'est le choix du gouvernement et de sa majorité. À l'initiative de la rapporteure dont je salue le travail Corinne Imbert. Le texte, nous allons examiner, a fait l'objet de nombreuses modifications. Ces dernières sont les bienvenues, notamment pour conserver le rôle central du médecin dans la coordination et le suivi des patients. Je vous remercie de votre attention. Merci et puis pour clore ces interventions des groupes, je passe la parole à Patricia de ma. Du groupe les républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme toutes les Françaises et les Français. Je partage l'exigence d'un accès aux soins pour tous soumis à une scène régulation surtout lorsqu'on sait que 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant. Que chaque médecin partant à la retraite laisse orphelin une moyenne de 1550 patients et qu'au regard de leur pyramide des âges et des effets tardifs attendu de la suppression du numerus clausus. Tout laisse à penser que la situation ne peut que s'aggraver. Ce constat d'urgence alarmant nous pose un cas de conscience et pour y répondre, l'obligation inévitables d'une évolution de notre système de santé. Le gouvernement a annoncé vouloir développer la profession des infirmiers en pratique avancée IPA pour lutter contre les déserts médicaux et soigner le système de santé. Son objectif était de 5000 IPA en 2022, ils sont quelque 1700 en 2023. C'est bien peu. Dans la mesure où les IPA trouveront cependant leur place, ils pourraient être rapidement plus nombreux à remplir un rôle important dans la régulation d'un secteur au bord de l'asphyxie, mais aussi dans la résorption de situation de soins dégradé par manque de médecins. Il pourrait être de plus un levier non négligeable de reconnaissance et d'attractivité pour les soignants. Ceci étant, le statut des IPA mérite d'être mieux encadrées et surtout mieux compris lorsqu'il s'agit d'accès Direct ou de primo-prescription comme le prévoit la proposition de loi, le risque. Je félicite à ce propos notre collègue rapporteur Corinne Imbert pour la qualité de son travail et le rééquilibrage du texte en discussion. Élu de la ruralité au prise directe des problématiques de désertification médicale. Je me suis essentiellement attachée aux implications concrètes que ce texte aura au quotidien. Mon principal sinon unique baromètre. Les patients trouveront-ils demain davantage d'IPA dans les déserts médicaux, particulièrement dans les territoires ruraux. Ce n'est pas certain, il faudrait qu'ils soient suffisamment nombreux et incité à s'installer dans un périmètre géographique sans médecin généraliste. Il conviendrait aussi que l'accès, la prise en charge durant les formations d'IPA soient les mêmes pour tous les infirmiers, ce qui n'est pas le cas il y a effectivement une rupture d'équité inacceptable qui frappe les infirmiers libéraux et qui est défavorable aux territoires sous tension où ils exercent souvent. J'invite donc le gouvernement a encouragé l'émergence de nouvelles passerelles et à favoriser censée exister mais dont l'application varie d'un département à l'autre. Autre point d'interrogation périphériques cependant en lien avec le sujet. Celui des assistants médicaux censés décharger les médecins des tâches administratives. J'aimerais comprendre Monsieur le Ministre pourquoi au regard des besoins exprimés par la profession. Il semblerait que nous soyons encore très loin du compte. Et puis dans la lutte contre les déserts médicaux. Je voudrais revenir sur l'appel à des médecins étrangers comme une autre solution insuffisamment exploité ce qui est regrettable, vous en conviendrez. Enfin j'ai le souvenir d'avoir voté dans le Plfss un article prévoyant en dernière année de médecine générale. Un stage en priorité dans les zones sous-denses. Qu'en est-il à présent. Notre système de santé est malade, nous le savons. Il nous faut agir avec lucidité, mais aussi avec courage, je plaide pour notre système de santé collective dont les besoins évoluent au fur et à mesure que notre population vieillit pour davantage de fluidité, de flexibilité, d'efficacité et de reconnaissance. Je plaide pour un système de santé évolutif au final utile à tous les Français. Je vous remercie. nous allons attaquer avec un amendement avant l'article 1er. Amendement présenté par Monsieur Chassaing. 74 rectifié. Merci monsieur le président, monsieur le ministre. Madame la présidente, madame le rapporteur, mes chers collègues. Donc cet amendement vise à préciser à l'article L. 41 du code de la santé publique définissant les missions du médecin généraliste de premier recours qu'il est le seul responsable du parcours de soins de ses patients, ainsi que de l'adressage vers un second recours. Le médecin généraliste et les ponts, la clé de voûte du parcours des soins coordonné bien au-delà de son rôle de coordinateur. Le médecin généraliste traitant et le responsable est le garant de la qualité et de et de la sécurité des soins prescrits aux patients. Cet amendement, nous paraît utile pour réaffirmer le rôle et les missions. Du médecin généraliste. Qui doit rester l'acteur et le responsable des soins coordonnés, merci. Merci monsieur le président, monsieur Ministre, mes chers collègues. Cet amendement me semble largement satisfait en droit, en effet, la loi, le code de la santé publique reconnaît déjà au médecin généraliste, l'émission d'orienter les patients dans le système de soins, de s'assurer la coordination des soins et de contribuer au suivi des maladies chroniques, notamment en coordination avec les autres professionnels de santé qui prennent en charge des patients donc d'autres professionnels de santé peuvent utilement intervenir dans le parcours de soins. En fait nous avons supprimé en commission la demande de rapport sur la pertinence de supprimer l'adressage préalable du médecin traitant précisément pour réaffirmer son rôle dans le parcours de soins, donc c'est un avis défavorable de la commission. Monsieur le Ministre. Je vous prie de l'excuser mon mon retard mais j'ai été pris à l'Assemblée par les écu âgé et et n'ait pu venir malheureusement pour la pour la discussion générale mais je suis vraiment ravi que nous nous retrouvions pour discuter des points. Précis de ce ce projet de loi qui est. Qui est important qui a été enrichi déjà par vos débats en commission qui j'espère va être encore enrichie dans dans les heures qui viennent. Monsieur le sénateur Chassaing vous proposez effectivement que le médecin généraliste soit le seul responsable du, du parcours de soin. Je vous rejoins lorsque vous dites que le médecin généraliste est la clé de voûte du système de santé bien entendu, je partage cette analyse. Mais la rédaction comme cela vient d'être dit actuel du code de santé publique précise déjà que le médecin généraliste et d'organisateur du parcours de soins de ses patients. Je vous donne l'Arctique ces deux elle 41 30 tirer hein qui précise que le médecin généraliste oriente ses patients selon leurs besoins dans le système de soins et s'assure de la coordination des soins nécessaires à ses patients. La souplesse qui est permise aujourd'hui doit être d'être être préservés pour 2 raisons, la première c'est continuer à rendre possible l'accès Direct à certaines spécialités, je pense en particulier à la gynécologie et. À la l'ophtalmologie ou le médecin traitant pour le coup généraliste n'est pas responsable de cet accès Direct la rédaction que vous proposez viendrait également à rendre le médecin responsable de tout événement. Au cours de du parcours de soin. Ce qui est quelque chose qui ne semble pas non plus raisonnable et un, un peu excessif. Donc de fait le votre demande étant déjà satisfaite. Je vous demande de retirer cet amendement sinon j'y serais défavorable.

Vous le retirer. Ou bien. Donc nous allons débuter le. La discussion de l'article premier j'ai quatre aux demandes de prise de parole. La première. Notre collègue à nouveau allô. Oui, merci monsieur le président, mes chers collègues dans les territoires médicalement sous-dotées la présence médicale de proximité constitue un enjeu vital dans bien des départements et notamment le mien, celui de l'Ardèche se faire soigner est devenue difficile tant les professionnels de santé s'font rares tiens je tiens à saluer le dispositif de l'article 1er prévue par les auteurs du texte qui consiste à revaloriser la profession d'infirmier en pratique avancée tout en remerciant Madame la rapporteure pour son travail de précision. Le mode de vie et l'éloignement géographique rendent de plus en plus difficiles et l'accès aux soins, tandis que le vieillissement de la population exige au contraire davantage de prise en charge. Nous observons de plus une explosion des pathologies chroniques, parmi lesquels le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, respiratoire. Si elles sont liées à notre mode de vie et notamment à notre sédentarité elles peuvent néanmoins être soignées à condition de mener un suivi régulier des patients. Dans ce contexte, il est donc judicieux d'intégrer la formation d'infirmier en pratique avancée dans le souci d'amélioration constante des professions paramédicales visant la qualité des soins et particulièrement ceux du quotidien. Au-delà de l'objectif de les bières et du temps médical l'IPA en exercice coordonné répond aux besoins de santé de la population par son implication et ses activités d'orientation d'éducation, de prévention ou de dépistage. N'oublions pas que ces professionnels sont des infirmiers expérimentés qui détiennent un diplôme d'état reconnu au grade universitaire de master Ainsi ses soignants selon moi toute leur place dans le parcours de soin du patient et un rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités médicales et territoriale. Alors certes, il convient d'avancer prudemment sur cette question, mais à condition que la rédaction du décret qui définira les contours de cette avancée ne savent pas les espoirs que fait naître cet article 1er je vous remercie. Merci cher collègue. Et je vais passer maintenant la parole à Madame Raymonde Poncet mon jeu. Merci monsieur le président. suite à l'adoption d'un amendement de Madame la rapporteure en commission l'article 1er permet l'accession à la pratique avancée des auxiliaires médicaux disposant d'un diplôme équivalent si l'objet de l'amendement précise que les infirmiers anesthésistes diplômés d'État les Ziyad sont concernés par cette accession à la pratique avancée. Le dispositif actuellement intégrés dans l'article 1er prévoit que la liste des diplômes équivalents sera fixé par arrêté du ministère chargé de la santé. Or une reconnaissance statutaire. Garantie est inscrite dans la loi est attendu depuis trop longtemps par la profession Iyad. Les Iyad bénéficie depuis. 1973 d'un diplôme bac plus 5, qui impose 2 années de pratique préalable à l'entrée en formation. Et qui a de grade master de depuis 2014. En août 2022, l'IGAS et j'. SR ont publié un rapport conjoint dans lequel elles appellent à reconnaître en pratique avancée d'exercice des Ziad. Ils ne veulent plus attendre. Monsieur le Ministre, un arrêté défini par le ministère qui les inclura de façon incertaine d'autant plus que ministre après ministre leur inclusion dans la pratique avancée l'promise sans être réalisés et ceci depuis Olivier Véran. une nouvelle fois renvoyé à une nouvelle promesse comment donc, dans ces conditions se fiait à un futur arrêté par conséquent nous Orion qui soit reconnu en pratique avancée dans le code de la santé publique. C'était l'objet de l'amendement que nous avons déposé et qui a été déclarée irrecevable alors même que cela ne modifie en rien la formation requise, comme la rémunération. Qui a fait justifiée au regard des évolutions porté par les articles 2 et 3 qui reconnaissent la caractéristique principale de la pratique avancée soit l'absence d'obligation de prescription médicale pour exercer à de professions qui ont aujourd'hui en terme d'autonomie, de pratiques et de formation les caractéristiques historiques des Ziad. madame la Ministre, précédemment nous a invités au travail sur les évolutions réglementaires faut gros. Oui, il est temps Monsieur le Ministre, de les reprendre et de les conclure justement avec les Merci. La parole à notre collègue. A pour sous-. Je souhaiterais donc intervenir à l'occasion de l'examen de cet article 1er sur la situation particulière des infirmiers et infirmières anesthésistes diplômés des d'État ce que l'on appelle les IADE. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir en commission des affaires sociales et dans cet hémicycle pour relayer leur lutte pour la reconnaissance de leurs compétences à l'occasion de l'examen de cette PPL une occasion nous est donnée de faire évoluer le statut des Iade en auxiliaires médicaux de pratique avancée. Pour rappel, en février 2021 nous débattions déjà favorablement de ce dossier pour finalement voir les IADE confronté à un blocage gouvernemental depuis janvier 2022, ils attendent que les engagements de ce même gouvernement sont se se concrétise. La seule réponse qui a été donné jusqu'en octobre dernier, était l'absence de vecteur législatif, nous y sommes tout est réuni pour leur attribuer enfin un statut à la hauteur de leur valeur au sein de notre système de soins là le faut de la la faute de l'article 40 à bloquer tout amendement visant à leur revalorisation. Il n'y a que le gouvernement qui puisse faire cette démarche et nous vous y invente Viton, Monsieur le Ministre, en attendant cet article donne l'occasion de rappeler la nécessité d'intégrer cette spécialité aux dispositifs auxiliaires médicaux en pratique avancée de fait les IADE remplissent les critères de la pratique avancée depuis des années mais sont exclus de la reconnaissance de cette pratique. À l'heure où le gouvernement souhaite faire reconnaître toutes les spécialités infirmières en pratique avancée il y a un risque réel de disparition des Iade, que faut-il penser de l'absence des Iade dans cette proposition de loi alors que la députée Rist leur a affirmé avoir rédigé cette PPL pour reconnaître leur métier en pratique avancée, que faut-il penser de tous les amendements déposés tous tombés à la faveur de l'article 40, les IADE nous regarde aujourd'hui et veulent des réponses. Merci. Merci. Et la parole est maintenant à notre collègue Philippe mouiller. avec un certain nombre de sénateurs et je pense notamment à collègue ma collègue Frédérique Puissat et mon collègue Derec point une usine si présent nous souhaitons profiter de cette proposition de loi pour attribuer un statut spécifique aux infirmiers anesthésistes diplômés d'État, au sein des auxiliaires médicaux en pratique avancée mais l'article 40 de la Constitution en a décidé autrement malgré des recherches de notre rapporteur pour trouver des solutions. En effet, la profession IADE, pionnière de l'exercice en autonomie supervisée a d'ores et déjà le niveau de qualification requis. Le manque de valorisation compromet dangereusement cette profession qui souffrent depuis de nombreuses années, du dissensus entre son activité réelle et son exclusion d'un statut juridique à l'auteur de ce compétence. Monsieur le Ministre, cette reconnaissance statutaire et recommandé des de plus d'un an par l'IGAS et avait été garanti par votre prédécesseur monsieur Véran s'engageant devant les instances médicales représentatives des professions de l'anesthésie à l'obtention d'un statut en pratique avancée pour tous les IADE différencier de celui disait PA au maintien des décrets des décrets réglementaires régissant la profession dit adieu et au maintien de d'formation actuelle. Le principe était de consacrer législatives ment aux IADE un statut unique et distinct de celui de la profession DPA. Au sein du Titre préliminaire du livre 3 partis du CSP par l'ajout d'un article L. 43 01 3. Nous souhaitions leur permet d'être reconnue comme une profession réglementée exerçant officiellement en pratique avancée avec des modalités spécifiques dans leur quatre domaines de compétence, ce qui est le cas depuis des années les médecins. Anesthésistes-réanimateurs soutiennent cette démarche de reconnaissance statutaire au sein de la pratique avancée dans le respect des décrets de sécurité anesthésique face à ce blocage, Monsieur le Ministre, nous souhaitons connaître hé bien votre position et quelles mesures souhaitez mettre en place. Merci. Merci Merci la parole à notre collègue Émilienne Pumerole. Merci monsieur le président. L'exercice de la médecine évolue en 2017 il n'y avait que très peu de MSP, et elle représente aujourd'hui plus de 20 pour % de l'exercice libéral. L'exercice coordonné un équipe de soins primaires est une nécessité à la fois pour faciliter le travail des soignants, mais surtout pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Il faut donc une équipe avec un projet de santé co-construit qui crée un véritable parcours de soins autour du patient dans ce projet co-élaborer et évaluer les IPA spécialisés ont toute leur place. La formation à la réponse à la prise en charge complexe leur permettra de répondent parfaitement à la démarche de soins primaires, il faudrait donc former plusieurs milliers d'IPA au suivi des pathologies chroniques, mais aussi en pédiatrie en cancérologie en psychiatrie en pédopsychiatrie etc par contre l'accès Direct aux IPA et la possibilité de primo-prescription en dehors de ces structures de soins coordonnés est une fausse bonne idée puisque donner une responsabilité à 10 IPA non formés au diagnostic est un risque pour les patients et on irait vers une médecine à 2 vitesses, les patients qui peuvent consulter un médecin généraliste et les autres qui, faute de médecins généralistes en particulier dans les zones sous-dotées serait vu par des IPA. Pour notre part nous sommes favorables à un parcours de soins coordonnés avec un partage et non une délégation même partage des tâches et le maintien un haut niveau de compétence donc une formation adéquate, je voudrais rebondir sur ce que viennent de dire mes collègues sur les IADE pour. En étant entièrement d'accord avec eux et, pour évoquer également le problème des iPods, c'est que les iPods ont aussi une formation de 2 ans supplémentaires. Aujourd'hui un décret est paru comme quoi on peut avoir, on peut faire en étant infirmier faire fonction de 10 Bode avec 28 jours de formation y a deux craignent le même décret, est-ce que vous allez les rassurer, Monsieur le ministre. Va très bien. Bien merci. Donc nous allons maintenant passer à l'examen des amendements. Monsieur le Ministre pour les diamants, allez-y. Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs je vous remercie d'avoir mis sur sur la table si je peux m'exprimer ainsi le le sujet des Iade. C'est effectivement un sujet que nous devons traiter. Mais je suis désolé de vous le dire, il ne pourra pas être traité ici pour plusieurs raisons. La première c'est que de par leur formation. Les IADE ne rentre pas dans le cadre des IPA les IPA ont d'abord une formation tronc commun et ensuite une formation de spécialités qui leur permet d'ailleurs au cours de leur carrière, de pouvoir changer de spécialité PA donc il faudrait, dans l'absolu rajouter une année aux IADE, ce qui serait totalement absurde. Notre raison c'est que vous avez parlé des Iade. Vous savez avez parlé des iPods. Il y a également des infirmières puéricultrices. Et toutes ceux-ci font partie du statut en tout cas c'est le le rapport vous avez évoqué de rapport IGAS IGF ESR du statut d'infirmières spécialisées qui est un statut différent. Ce que je me suis engagé à faire et et je continue à vous le dire, c'est de travailler sur ce statut d'infirmières spécialisées pour. Les reconnaître en pratique avancée toutes les trois et pas simplement les IADE de travail cela avec les sociétés savantes, j'en ai discuté avec la société française d'anesthésie-réanimation encore la semaine dernière en ce qui concerne les Ziad. Nous allons travailler avec les professionnels, médecins, infirmiers de chaque groupe pour aboutir, nous aurons des textes législatifs en fin d'année, bien entendu pour aboutir sur un statut particulier qui reconnaîtra un exercice de pratique avancée mais sans pour autant les enfermer dans le statut d'IPA en tout cas je suis particulièrement sensible à à ce sujet et nous allons avancer. Ça a été effectivement promis aux Par mon prédécesseur et je vais avancer sur cette ligne, mais surtout n'oublions pas les iPod et les plus pierres dans ce sujet, je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. L'Arctique le 1er étend le Champ des compétences des infirmiers en pratique avancée aux prescriptions de produits de santé et à la prise en charge directe des patients dans le cadre d'un exercice coordonné cette PPL présentée comme une réponse aux déserts médicaux ne répond pas aux attentes et besoins en matière de soins, le médecin doit rester celui qui pose le diagnostic est défini la stratégie thérapeutique. Il est formé pour cela, 9 ans d'études prochainement 10 ans comment une IPA ou un IPA formés aux soins et n'y voyez aucune défiance pourrait avoir la même connaissance et la même compétence en 5 ans seulement. Le dispositif pratique avancée est une perte de temps et éventuellement une perte de chance pour le patient. C'est une médecine à 2 vitesses, ceux qui auront accès à un médecin et les autres. Mes chers collègues, quand vous avez besoin pour vous-même ou pour vos proches d'une prise en charge médicale à qui vous adressez-vous à un médecin bien sûr, je souhaite que tous les Français puissent avoir le même accès ce dont les médecins ont besoin c'est de plus de temps médical moins de tracasseries administratives, traiter le problème des rendez-vous non honorés. Et je ne parle pas du signal envoyé aux patients, aux jeunes médecins aux étudiants en médecine cette PPL éteint l'heure c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Cet amendement vise donc à supprimer cet article, je vous remercie.

Je pense que sans surprise. Dominique que le l'avis de la commission est un avis défavorable en effet certes article 1er a été largement revu par notre commission pour mieux encadrer l'accès Direct et la primo-prescription permis et j'espère qu'il permettra, dans sa rédaction actuelle texte telle qu'issue des travaux de la commission qu'il permettra d'améliorer à la fois l'attractivité de la pratique avancée mais aussi et c'est important de sécuriser les conditions de prise en charge. Voilà donc ce sera un avis défavorable de la commission. Je ne vous en veux pas ma chère collègue je connais vos vos préoccupations. La qualité des soins ne doit pas être. Mise à mal et je vous rappelle que la façon dont nous l'avons encadré. C'est avec un décret en Conseil d'État préavis de l'Académie nationale de médecine. Avis de la Haute autorité de santé l'avis des représentants des professions concernées. Voilà en termes de garanties. Ce que nous avons apporté avec la Commission et donc c'est un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le ministre. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs, madame la sénatrice de Seine. Bon, bien évidemment, vous comprendrez que je suis également défavorable à votre amendement mais je voudrais juste développer un tout petit peu. Les IPA sont des infirmières qui ont trois ans de formation qui ont 4 ans d'exercice professionnel Pulse, 2 ans de formation complémentaire on arrive donc à neuf ans de formation pour pour ces infirmières, ce qui est loin d'être négligeable. Pour autant bien entendu elle ne remplace pas et ne remplaceront jamais un médecin et le médecin généraliste. Je pense qu'il est important dans cette place des IPA dans notre système de santé que nous voulons reconstruire, c'est bien de comprendre que les hypers ne sont pas là pour remplacer le médecin les IPA sont là pour donner une solution complémentaire dans l'organisation de notre système de soins la colonne vertébrale que représente le médecin traitant un exercice coordonné la commission a travaillé en ce sens et à renforcer ce principe de l'exercice coordonné. Mais pour autant, la question qui continue à se poser, c'est l'IPA peut-elle doit-elle être un point d'entrée lorsqu'on ne peut pas trouver de médecin traitant. On ne peut pas trouver de médecins généralistes. Eh bien certainement. Je pense qu'il est plus intéressant qu'elle soit le point d'entrée pour diriger vers un médecin traitant. Et c'est bien dans ce sens-là qu'on, qu'on soit son entrée plutôt que le patient ne trouvent pas de médecin traitant et se retrouvent dans les services d'urgence où vous connaissez particulièrement les problèmes donc pour l'ensemble de ces raisons je suis défavorable les IPA ont une place dans notre système de santé. Ce n'est pas la seule solution. Par contre c'est pas une emplâtre sur une jambe de bois. Je suis désolé, il y a d'autres solutions, et c'est par la combinaison de l'ensemble de ces solutions. Vous parlez du temps administratif hé bien la semaine dernière j'ai annoncé 15 mesures pour diminuer la paperasserie. Si je peux m'exprimer ainsi des médecins. Ça va dans ce sens. C'est avec toutes ces solutions mises côte à côte, qu'on arrivera à prendre en charge les 6 millions de nos concitoyens qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant.

Merci monsieur le président. Je dois dire que les propos de Chantal de scène on pouvait souscrire très largement. Ça aurait emporté la conséquence éventuellement de notre part de dire que l'article n'était pas recevable. S'il n'avait pas été modifié par la commission parce que l'article un tel qu'qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale avec cette distinction entre les IPA spécialisés et les IPA et les IPA praticiens aux praticienne. Je ne sais plus quel genre auraient été. Utilisé. Mais. Prêter à interprétation de par le flou de cette notion d'IPA praticien qui n'est nulle part dans le code et qu'qui n'était pas définie dans la proposition de loi, proposition est pas proposé le projet de loi, Monsieur le Ministre, comme vous l'avez dit, mais c'est un lapsus qui comme tous les lapsus c'est très révélateur. Hé bien. Ce cette cette rédaction. Vous donner entièrement raison cher collègue. C'est-à-dire qu'on en, on mettait les 2 pieds dans un système dont les deux vitesses était institutionnalisée et il y aurait eu des territoires où les en avait le droit de voir un médecin et les autres auraient eu le droit de ne voir qu'un infirmier et ça n'est pas péjoratif en première intention mais voilà, la commission a quand même clarifier les choses à poser des bornes et un cadre qui est beaucoup plus restrictif. Et l'objet de mon intervention, c'est non seulement de dire que, qu'on ne on votera contre cette ah la la suppression puisqu'on approuvera l'article 1er telle que rédigée mais n'en appeler aussi à la responsabilité du gouvernement puisque c'est lui qui êtes. Qui est Qui est à la manoeuvre sur ce projet. Cette proposition de loi et qu'il. Que dans la suite de ce texte on n'aboutisse pas à ce que Madame de scène. Décrit donc c'est en rejetant son amendement et en votant pour l'article hein c'est un peu un vote de confiance aussi, mais nous tenons à le préciser de façon très claire. Monsieur Jomier, donc nous allons passer au vote sur cet amendement qui est favorable à l'amendement.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il est rejeté. Donc maintenant nous allons.

Merci monsieur le président. Alors si vous voulez, notre système de santé est en difficulté notre pays manque de médecins. Bon ça va pas s'améliorer et il faut évidemment trouver des solutions pour améliorer à court terme, l'accès aux soins des Français. Nous ne pensons pas que l'accès Direct. Aux infirmiers aux IPA soit une solution. Certes la création de cette profession. Est plutôt tout à fait bien et nous le souhaitons, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques l'SIPA peuvent assurer le suivi des patients qui leur sont confiées par un médecin pour certaines pathologies permettant d'augmenter le temps médical de ce dernier toutefois remplacé en première intention un médecin par. Un infirmier ne saurait être la solution au manque de médecins, donc souvent. Ça souffrent souffrent certains Français. Quand bien même les IP a bénéficié d'une formation approfondie sanctionnée par un master, elle ne peut pas remplacer celle de médecins qui doit garder la compétence du diagnostic nous pensons que médecin IPA doivent travailler ensemble en synergie, par délégation, seul un médecin est apte à faire un diagnostic après 10 années d'études. hein donc. 4 année d'internat, une collaboration étroite et indispensable. Cependant, c'est le médecin qui est en fonction des rendez vous doit décider quel patient il va être confiée à l'IDA en consultation et oui en visite. Et en cas d'anomalie des constantes retrouvées par l'IPA le médecin qui sera présent à proximité pourra intervenir et presse créer éventuellement des examens complémentaires. Une modification de de traitement ont un accès Direct à l'IPA. une une absence de médecin, le médecin le patient devra revenir en consultation, ce qui risque d'entraîner une perte de temps. Une confusion les travaux portant sur la pratique d'une infirmière Manser monte des preuves d'efficacité uniquement lorsqu'il existe une collaboration réelle entre médecins traitants et infirmiers. Merci cher collègue.

Madame le rapporteur, madame la présidente de la Commission. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les médicaments à prescription médicale obligatoire sont classés en 3 catégories liste un disque de stupéfiants en fonction des risques pour la santé qu'il présente et de la nécessité d'une surveillance médicale du patient. Tout au long de son traitement. Certains de ces médicaments présentent des conditions particulières de prescription et de délivrance dans la mesure où les infirmiers de pratique avancée pourraient désormais prescrire ces produits de santé a prescription médicale obligatoire et que ces prescriptions auraient un impact pour différents professionnels, il convient de consulter les ordres des professions de santé compétent avant de déterminer la liste des médicaments et dispositifs médicaux concernés. Merci. Ensuite l'amendement 53 Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, comme je l'ai rappelé lors de mon intervention en général nous avons soutenu l'expérimentation de la primo-prescription par les IPA lors du PLFSS 2022 je l'ai dit également nous sommes favorables à la valorisation des professions paramédicales, à l'octroi de davantage de compétences. nous aimerions que vous nous expliquiez, d'une part. Pourquoi une expérimentation votée en décembre 2021 n'a toujours pas débuté. Et d'autre part qu'est ce qui justifie une généralisation sans évaluation de fait dès aujourd'hui. Il y a de nombreuses propositions, adoptées par le Parlement, qui sont d'abord des demandes d'expérimentation. Quel est le sens de mesures de généralisation sans passer par des expérimentations qui sont votées dans les hémicycles. Il y a quand même là un certain paradoxe, Monsieur le Ministre, vous êtes venu, vous dites que vous tenez à être parmi nous. Au niveau de cette haute assemblée ben dites-nous pourquoi vous faites PACA des votes que nous émettons quand il s'agit d'expérimentation au mieux on a perdu un an et demi et la généralisation aurait pu débuter dès 2022 au pire on risque de regretter cette généralisation trop hâtive. Nous avons bien noté que l'évolution du nombre d'IPA en France était insatisfaisante car trop lente. De ce fait l'article 1er, De ce fait l'article 1er, ah pour vous vocation y remédier en renforçant leur mission mais n'est-ce pas aussi votre crainte de finalement voir comme nous le pensons des effets quasi nul du numerus apertus sur l'accès aux soins qui vous fait aujourd'hui accélérer le calendrier. La primo-prescription médicale n'est pas un acte anodin et il nous semble essentiel d'avoir bien tous les arguments pour justifier une introduction directe dans le droit commun. C'est le sens de notre amendement et j'espère, Monsieur le Ministre, ce que vous nous apporterez des réponses. Bien ensuite l'amendement 77 rectifié Monsieur Chassaing. l'amendement supprime la possibilité pour les IPA de prescrire des produits de santé, ainsi que des prestations soumises à prestation médicale obligatoire il est licite de lister une série d'actes et de. Il est très Il est en effet du ressort du médecin généraliste d'apporter un diagnostic complet de juger du caractère bénin et non de symptômes après examen clinique. Alors si vous voulez le lorsque moi je préconisé. Une infirmière de pratique avancée. Qui fonctionnerait en collaboration avec le médecin avec un partage par exemple des consultations des visites mais. Toujours le médecin à proximité si long, si par exemple

le travail doit se faire mais moi je suis pour l'IPA à fond mais la le travail doit se faire entre l'IPA et le médecin et le médecin doit déléguer à l'IPA et travailler en synergie, mais ça c'est très bien parce que ça va apporter du temps aux médecins du temps médical. Merci l'amendement 89. Madame Imbert. Si si. Rédactionnel, monsieur le président. Amendement rédactionnel le 7 rectifié. Madame Delmont Koropoulis. Monsieur le Président Madame Monsieur le Ministre, Mesdames, messieurs les rapporteurs. Mes chers collègues. Dans la même veine des diagnostics de de certains de mes collègues et je rapporte l'amendement de Madame Delmont Koropoulis. L'objectif des IPA effectivement été dédié aux prises en charge protocole Izé en ville et notamment en soins primaires et ne saurait donc s'exonérer du diagnostic il n'apparaît donc pas concevable au regard des exigences de qualité et de sécurité de soins que des patients qui n'ont pas bénéficié de ce diagnostic médical soit pris en charge directement par un IPA en dehors d'un médecin dans toute équipe de soins ambulatoires ou hospitalières. Il y a un médecin qui assure la coordination de la prise en charge du patient et un protocole organisationnel. On ne saurait substituer à cette organisation. Une démarche d'accès Direct aux IPA. Bien Madame Guillotin nous suivons. Oui donc le le l'objet et est le même que le précédent. L'idée effectivement de, de dire que l'IPA Les Halles infirmières de pratique avancée nécessite effectivement une montée en compétences et je crois qu'elle doit travailler dans un dans un espace coordonnée. Moi je suis très attaché, en fait à ce que le médecin traitant, reste au coeur de cette de cette coordination et que le si accès Direct il doit le, il y a, il doit y avoir, c'est toujours en lien avec le médecin traitant et ne pas laisser en fait une désorganisation de la médecine. En tout cas s'installer. C'est pour ça que j'ai posée cet amendement.

l'exercice de l'IPA et toujours coordonné par un médecin et protocoles Izé les termes sans adressage du médecin crée une confusion. Donc c'est défendu. Défendu. Bien. Donc madame la rapporteure notre avis sur cette série d'amendements. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc ces amendements pour la plupart pour objectif de revenir sur les compétences attribuées aux infirmiers en en pratique avancée par l'article 1er, l'amendement. Numéro 78 de Monsieur Chassaing supprime l'accès Direct et la primo-prescription. Le 77 de Monsieur Chassaing supprime la primo-prescription. Le 53 de Madame Cohen supprime la primo-prescription est rétabli en la matière, l'expérimentation votée en 2021. Les amendements identiques cette de Madame Delmont, Koropoulis c'est 36 de Madame Guillotin limite l'accès Direct à un exercice protocole Izé avec le médecin. Et les amendements identiques huit de Madame Delmont Koropoulis ses 37 Madame Guillotin supprime la mention d'actes sans adressage préalables. L'accès Direct et la primo-prescription correspondent à des attentes importantes des infirmiers en pratique avancée doivent améliorer les conditions de prise en charge des patients, ils ne seront possibles. Que dans le cadre d'un exercice coordonné avec le médecin. La commission d'ailleurs renforcer les conditions en réservant l'accès Direct en ville aux structures les plus intégrés partageant une passion telle commune. En outre, le décret sur les infirmiers en pratique avancée prévoit déjà qui n'exerce que dans le cadre d'un protocole d'organisation conclu avec le médecin. Cette condition est donc déjà satisfait en droit. C'est pourquoi la Commission à Nîmes a émis un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements en fin d'amendement numéro 42 de madame Berthe et prévoit que les ordres professionnels doivent être saisis préalablement à toute adoption d'un décret relatif aux compétences d'un auxiliaire médical en pratique avancée. La loi prévoit déjà la consultation de l'Académie de médecine et des professionnels concernés. Nous l'avons en commission enrichi pour prévoir également la saisine de la Haute autorité de santé la commission sur cet amendement numéro 42 émis un avis favorable cette implication permettra d'inclure les ordres dans les réflexions relatives au partage des tâches à la suite notamment des travaux importants menées ces derniers mois par le comité de liaison inter-ordres le Clio. merci madame la rapporteure et monsieur le ministre. Très brillamment déployés par par la rapporteure mais simplement apporter quelques éléments de concept et en tout cas de de précision déjà je remercie le le sénateur, je mets pour sa confiance et je suis sûr que j'en serai digne parce que l'idée que nous avons sur la reconstruction de notre système de santé pour mieux répondre aux besoins de santé de la population, nous le partageons. Nous voulons tous ensemble, améliorer notre système de santé. Je vous le redis, ça ne se fera pas par une seule mesure mais par un ensemble de mesures qui vont se compléter. Je reviendrai sur le point de l'exercice coordonné. Je crois que c'est, c'est le mot essentiel dans toutes ces discussions, l'exercice coordonné veut bien dire coordonnée par un médecin traitant, par un médecin généraliste traitant voir quand même dans le cadre du décret des IPA par un médecin spécialiste dans le cadre de protocole défini avec les PA pour la suite de la suivre les pathologies chroniques. Je pense en particulier un diabète par exemple donc déjà nous avons un un cadre qui nous permet d'avancer cet exercice coordonné précise sécurise cet accès aux IPA en lien, en coordination avec le médecin traitant du patient. Pour cette raison sur l'ensemble des amendements qui ont été cités et qui remettent finalement en cause cet accès Direct à l'IPA j'aurais un avis défavorable en ce qui concerne les amendements 89 37 et 8 qui sont des amendements essentiellement rédactionnel un avis favorable du gouvernement. Bien. Donc nous allons procéder au vote de ces amendements je suis saisi je je préviens ou une demande de scrutin public sur le 78 sur le 53 et sur le 77 rectifié. Donc comme nous allons commencer par le 78. Donc il y a une demande de scrutin public sur le 78. Alors. Pardon. Il faut souligner pour explication. Monsieur Jo. C'est Global une une explication de vote global sur les amendements. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci Monsieur Président donc sur l'amendement 78 que pardon, nous nous ne voterons pas. Nous suivrons la position de la commission mais sur cette question du manque de médecins quand même un mot. Parce que la pénurie de médecins. On voit bien une motivation majeure à tout ce dispositif. J'ai rappelé tout à l'heure Monsieur le Ministre, que vos deux prédécesseurs avaient refusé dans cet hémicycle. Tous les amendements qui visaient à la valorisation de la profession infirmière des amendements qui ont été votées par le Sénat. Plusieurs années de suite et là d'un coup on voit que il s'agit même plus de créer un infirmier référant d'avoir des petites avancées mais un espèce de seau quand même majeur. On va dire

Mais malgré tout il faut répondre à la pénurie de médecins, et moi je tiens à souligner que la transformation du numerus clausus en numerus apertus c'est une simple opération de communication pardon. Mais 15% de médecins formés en plus alors que. Tous les indicateurs nous disent que les jeunes ne veulent plus choisir la médecine générale du fait de l'avalanche de dispositions négatives envers cette profession et que le taux d'abandon maintenant est à 2 chiffres dans les études. Ce simple fait va annihiler. Complètement l'augmentation du nombre de médecins formés. Alors on nous a d'abord dit la pénurie le creux sera 2026, puis ce sera de 2030. Maintenant nous parle de 2032 à 2035. Monsieur le Ministre, si on augmente pas fortement le nombre de médecins formés effectivement on donne raison à ceux qui disent qu'on est en train, au nom de la pénurie de changer d'île hébergement de système et donc de dégrader l'accès aux soins dans notre pays. merci merci Monsieur le Président, je voulais juste intervenir parce que c'est vrai que l'amendement de notre collègue chassant m'a interpellé depuis plusieurs jours et je, je me suis posé la question pendant. Ces jours ci ces derniers jours pour le cosigné ne pas cosigné, j'ai bien écouté la discussion générale et ce qui m'a surpris quand même dans cette discussion générale c'est que une majorité de sénateurs qui se sont exprimés. Globalement, le fond, la forme n'était pas là, mais finalement on allait voter parce que, ben oui. Beaucoup de patients n'ont pas de médecin général liste aujourd'hui mais on ne sait pas si c'est une bonne solution mais on décide de le voter lorsque j'entends aussi notre collègue à l'instant parler de l'attractivité de la médecine générale. Oui c'est un vrai problème aujourd'hui toutes les mesures qui nous sont proposées au travers de divers. PPL nous. Finalement réduisent l'attractivité de la médecine générale, lorsqu'on décide de peut-être de se dire on va imposer une installation dans les dans les On va finalement. Changé le, le parcours de soins. Donc moi je. Je je je souligne le travail de la rapporteure vraiment le qui a tenté d'améliorer le texte mais je vais voter l'amendement de notre collègue chassant parce que le protocole qui est proposé pour moi c'est pas une garantie de simplification j'ai pas l'impression qu'on simplifie les choses, j'ai l'impression qu'on complexifie les choses je me connais pas. Quand je dis ça. La formation complémentaire qui des

1er telle qu'il est sorti de la commission des affaires sociales vous convient. Or ça n'est pas du tout celui qui est sorti de l'Assemblée nationale qui vous convenait aussi et moi je vous pose une question simple qui allait finalement du Sénat ou l'Assemblée nationale au niveau de la CMP, le texte qui aura votre soutien.

d'abord, on parle beaucoup mais en fin de compte il y a très peu d'IPA donc voilà c'est on parle un petit peu pour rien et puis on a l'impression qu'on est en train de dresser de profession, l'une en face de l'autre, à savoir peut être que les médecins. Donnerait l'impression de défendent leur précarité et qu'en face on refuserait, donnez des attributions infirmiers alors ce serait tellement grave de faire ça en ce moment alors qu'on a besoin de tous nos professionnels de santé et Monsieur chassa insiste sur le fait que le seul moyen de s'en sortir c'est en jouant sur la collaboration entre tous les professionnels de santé, c'est pour ça que je voterai son amendement. Oui, je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit ce Jomier. Je suis complètement d'accord avec lui, mais pour avoir davantage de médecins. Il faudrait aussi par exemple laisser redoubler les élèves qui ratent leur premières années qui sont motivés pour faire médecine. Parce que Au lieu de les décourager leur dire de toute façon vous avez raté la première année. Donc vous êtes un bon à rien. La 2ème chose. C'est dire qu'effectivement vous prenez comme exemple, toujours pour vanter je dirai la possibilité de résoudre le problème de la désertification médicale avec les IPA en prenant toujours l'exemple des maladies chroniques. Or l'accès Direct ne sera pas si j'en crois ce que je peux, j'ai pu lire ou comprendre que ce soit uniquement pour les maladies chroniques, on comprend bien que les maladies chroniques seront d'abord diagnostiqué par un médecin et qu'il y aura un suivi et là on comprend la coordination. Dans les autres cas, je ne le vois pas et je pense que c'est pas une avancée, c'est véritablement une médecine à 2 vitesses, voire à 3 vitesses parce qu'il y a aussi les déconventionner. Bien, je n'ai plus de demandes d'explications de vote, donc nous allons voter. Les amendements un par un. Donc on va commencer par l'amendement 78 je suis saisi d'une demande de scrutin public. Il y a un double avis défavorable. il y a un double avis défavorable sur l'amendement 78. Donc demande de scrutin. Public. Et donc nous allons procéder au scrutin public dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement. C'est vraiment

Le scrutin est clos. Votants 343 exprimés, 312 pour 37 contre 275. L'amendement n'est pas adopté. Ensuite, sur l'amendement 42 de Madame Berthet donc un double avis favorable. De la commission et du gouvernement. Donc il est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Sur le 53 de Madame Cohen. Je suis saisi d'une demande de scrutin public. Avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. Votants 343 exprimés, 312 pour 86 contre 226. Amendement n'est pas adopté. Ensuite le 77 rectifié Monsieur Chassaing demande de scrutin public. Donc avec un double avis défavorable. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions prévues par l'article 56 de règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. Votants 343 exprimés, 327 pour 36 contre 291. Il n'est pas adopté ensuite l'amendement 89 amendements rédactionnels. Madame Imbert. Avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté le 7 rectifié présenté par Monsieur saumon avec un double avis défavorable. Alors les 2 sont identiques, le 7 et le 36 rectifié le 1er présenté par Monsieur saumon le deuxième par Madame Guillotin avec un double avis défavorable. Qui est pour.

Si je ne me trompe pas, là il y avait un avis défavorable de la commission mais favorable du gouvernement, du gouvernement. C'est bien ça. Donc il est pour ces amendements. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Donc nous, ah. Il y a un dernier amendement sur cet article. Un amendement présenté par Madame Berthet le 41 rectifié. Merci monsieur le président. Madame le rapporteur, Monsieur le Ministre. L'article 1er de la présente, proposition de loi instaure la possibilité d'une primo-prescription par les infirmiers de pratique avancée. Or le renouvellement et l'adaptation des prescriptions médicales par les IPA dans le cadre d'un protocole de soins défini avec le médecin pose déjà aujourd'hui, difficultés d'application concrète pour les pharmaciens chargée de dispenser ses ordonnances. En effet, selon l'article R 42 35 48 du code de la santé publique. Le pharmacien doit assurer l'acte de dispensation dans son intégralité et réalisé notamment une analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, quel que soit le prescripteur. Les bonnes pratiques de dispensation prévoit d'ailleurs que le pharmacien doit vérifier la validité de l'ordonnance d'identité du patient la régularité formelle de l'ordonnance et L'article R 43 01 tiré quatre du code de la santé publique prévoit que le protocole établi entre l'IPA. Et le médecin est porté à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins. Or le pharmacien d'officine s'n'exerce pas au sein d'une structure d'exercice coordonné n'est pas reconnue comme faisant partie de l'équipe de soins telle que définie au elle en se disent tiré 12 du code de la santé publique. Il ne dispose donc pas des informations nécessaires à la dispensation sécurisée des médicaments prescrits par les IPA alors même qu'ils peuvent renouvelé ou adapté des traitements qui présente des conditions particulières de prescription. pour exercer sa mission en toute sécurité réalisé l'acte de dispensation dont il a la responsabilité. Le pharmacien doit pouvoir vérifier le cadre dans lequel l'IPA peut renouveler et adapter la prescription initiale ainsi qu'être informé de la procédure établie par le médecin qui précise les modalités de ce renouvellement Ehud d'adaptation ainsi le présent amendement prévoit que dans le cadre d'un exercice en pratique avancée, le pharmacien délivrant les médicaments médicaments prescrits et réputé, membre de l'équipe de soins en conséquence le protocole lui sera communiqué et il pourra assurer l'acte de dispensation dans son intégralité dans un cadre sécurisé. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les conditions dans lesquelles un infirmier en pratique avancée pourra prescrire et le maintien notamment des protocoles d'organisation actuelle devront être déterminées par décret en Conseil d'État prix avis. De la Haute autorité de santé de l'académie a. De médecine. Sur l'opportunité d'inclure dans ce cadre, le pharmacien dans l'équipe de soins. La commission a souhaité solliciter l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Monsieur le Ministre. Oui monsieur le le président, madame la rapporteure mesdames et messieurs les les sénateurs. Donc votre amendement propose que le pharmacien délivrant les médicaments prescrits par un IPS soit réputée, membre de l'équipe de soins dans le cadre d'un exercice de la pratique avancée donc. Je voudrais juste préciser quelques éléments réglementaires actuel. Ah bon, pardon excusez. Préciser quelques règlements le règlement actuel. En tout cas, le cadre législatif. Tout d'abord le patient est libre de choisir la pharmacie de son choix et c'est quelque chose d'absolument essentiel dans notre organisation le le concept de pharmaciens traitant n'existe pas en tant que telle peut donc aller chercher avec une ordonnance, ces médicaments dans toutes les pharmacies et le pharmacien déjà actuellement peut délivrer des médicaments qui sont prescrits par un professionnel, y compris en pratique avancée dès lors que la prescription est conforme à la réglementation. Dès lors, je pense que rajouter cet échelon va complexifier le parcours de soins l'alourdir. Ce qui est quand même l'effet adverse de ce que l'on cherche dans ce cette PPL cette région ce serait défavorable à votre amendement.

Dans le parcours de soins il ne n'aura pas tous ces éléments et cela pose déjà problème actuellement. Par rapport aux presque fin au renouvellement d'ordonnance aux adaptations de posologie, que peuvent faire les IPA. je pense qu'il y a vraiment nécessité à ce que le pharmacien soient bien inclus dans le parcours de soins. Dès lors, puisqu'il y a justement et c'est important, comme vous l'avez souligné, puisqu'il y a liberté de choix de son pharmacien dès lors que le pharmacien est confronté à une ordonnance prescrite par un IPA mais n'est pas dans le parcours de soins, il faut bien qu'il ait l'ensemble des éléments. Merci Madame Berthet. Donc quel est l'avis de la commission.

Merci monsieur présent pour notre part, nous allons nous abstenir parce que Madame Berthet. Elle pose au fond la question de la responsabilité et que la réponse qui est donnée n'est pas satisfaisante. et c'est d'ailleurs hein. Une question qui plane sur l'ensemble de ce texte, c'est que quand on exerce une mission de soins, un acte de soin, on en est responsable individuellement et donc madame Berthe et réclame un peu une garantie d'une meilleure connaissance du dossier du parcours pour pouvoir exercer sa responsabilité dans des meilleures conditions et il y a une fragilité dans tout ce texte c'est que à chaque fois ben ce principe de responsabilité, on ne sait pas trop comment il va s'exercer, précisément, ça a été dit tout à l'heure, pardon, j'ai oublié par qui. Excusez-moi mais. Entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle en tout cas c'est clair. Le professionnel du du de santé a une responsabilité individuelle et à partir du moment où il accepte le transfert d'une mission, il va devoir ex-verser cette responsabilité individuelle l'infirmier qui voit un enfant qui a mal au ventre. Si 10 gastro-entérite et qu'en fait c'est une colite ischémique et qu'il la rate et ben il en assumera les conséquences à titre individuel, et ça on ne l'explicite pas beaucoup je trouve dans le texte qui est proposé parce que c'est une proposition de loi, on n'a pas l'avis du Conseil d'État sur cette question qui est pourtant essentiel et qui fragilise le dispositif. Voilà donc on va s'abstenir, mais nous on entend tout à fait la légitimité l'importance de la question que pose notre collègue. Monsieur le ministre. monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je, je me permets juste de rappeler sur cette question de responsabilité. Vous avez raison, c'est un sujet qui est, qui est essentiel. Tout professionnel de santé responsable de ses actes et je me permets de rappeler l'article L 43 01 tirer 1 du code de la santé publique qui spécifique sur les exilés médicaux en pratique avancée le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'ils réalisent. Donc en tant que telle. Ils sont responsables les IPA au même titre que les autres professionnels de leçon. bien je vais donc soumettre l'amendement. On voit avec un double avis défavorable. Qui est pour cet amendement.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Donc maintenant on va passer au vote de l'article 1 et je suis saisi d'une demande de scrutin public. Par le groupe Les Républicains. La ville, la commission et.

qui aura l'Avantage et le soutien du gouvernement puisqu'il est différent de l'article 1 de l'Assemblée nationale. monsieur millions juste pour vous. C'est que, au cours des débats parlementaires le texte a été améliorée et que bien sûr je, je m'en remets à la commission mixte paritaire sur le choix qui sera fait.

Merci monsieur le président pour une explication de vote également sur cet. Article. Parce que j'entendais les arguments d'orateur précédent alors j'ai pas toutes les qualifications que certains peuvent avoir mais je revendique au moins une pratique avancée de mon territoire qui me permettent d'apporter un point de vue et je dois dire, j'ai entendu c'est la mise en place d'une médecine à 2 vitesses à 3 vitesses, mes chers collègues, la réalité c'est que aujourd'hui hélas dans beaucoup de territoires, et d'ailleurs nous posons pas la ruralité à la ville et c'est. Ce que nous pouvons trouver parce que certains de nos concitoyens. N'arrive pas à trouver un médecin traitant. Et donc nous avons avec cet article. un outil supplémentaire dans une palette d'instruments, le ministre-là parfaitement bien dit c'est pas une mesure unique qui va permettre de résoudre le problème de l'accès aux soins. Je crois que nous avons déjà depuis quelques années pris. Ce chantier à bras le corps avec enfin le numerus apertus. Avec également récemment le. Le ministre a rappelé les 15 mesures prises pour simplifier aussi l'avis du médecin pour dégager du temps médical et donc j'aimerais dire enfin enfin nous y arrivons parce que j'ai souvenir, il y a une quinzaine d'années des débats que nous avions sa loi HPST et à l'époque hein combien il était difficile d'avancer sur des mesures. Supplémentaires pour favoriser cet exercice coordonné. Alors certes il y a eu des embryons de de dispositifs mis en place à l'époque, mais aujourd'hui je crois que c'est un moment important que le vote de cet article. Et c'est pourquoi pour ma part je le voterai dès demain. Alors nous, Monsieur le Président merci. Nous allons vous nous prononcer tout de suite. Personnellement. Ce vote est important et. L'échange qui vient d'avoir lieu entre Alain Milon. Et le ministre aussi important, il faut remercier le ministre, de nous répondre dans dans l'hémicycle à chaque fois ça n'a pas toujours été le cas, on a des souvenirs. Eh bien il est important parce que ce cadre-là font vraiment notre vote et quand je veux parler de confiance tout à l'heure, c'est que le texte reste malgré tout instable et imprécis et nous avons. Fermement et fortement critiqué la méthode du gouvernement d'avoir imposé la délibération de ce texte dès maintenant alors que des négociations conventionnelles sont en cours. La CMP n'est pas obligatoirement convoquée très rapidement du temps peut être donné maintenant dans la suite de la procédure parlementaire. Pour réfléchir et pour trouver la meilleure solution. Alors la réponse du ministre qui dit qu'il s'en remet parlementaire est logique S'agissant d'une CMP, on n'aurait pas attendu une autre réponse de la part d'un ministre, mais encore une fois. Nous sommes. Quand même dans des dispositions qui sont de reconnaître aux infirmiers à certaines conditions. Une juste valorisation de leur profession. Mais cette juste condition c'est d'entendre les inquiétudes à la fois sur le système à 2 vitesses et sur la place du médecin parce que ceux qui disent que le médecin est formé et ce sera plus 9 ans pour les médecins généralistes, ce sera 10 ans, je je le rappelle au regard de la complexité de leur métier ne peuvent pas entendre, en même temps qu'on ouvre la porte dans n'importe quelle condition à des exercices de fonction de diagnostic et de traitement et donc c'est cet article que nous approuvons. Monsieur le Ministre, avec le cadre qui a été posée et moi j'en appelle encore une fois la responsabilité de l'exécutif qui a la main sur ce texte pour que ce cadrage là soit au mieux respectés dans fendu dans la suite de la procédure, je vous remercie. merci, Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Alors chers collègues. Pour voter ce texte dès demain. Sincèrement, faut quand même prendre son élan. Moi je vais le voter mais c'est un petit oui à un grand mais. Oui parce que il y a le travail de la commission et de Corinne Imbert mais parce que on voit bien que beaucoup de questions se posent et qu'on a un vrai doute Monsieur le Ministre et que vous lever ces doutes partiellement sur la question de la médecine à 2 vitesses sur la question du devenir de la médecine générale de son attractivité. Quand on a des étudiants en médecine dans notre famille, on voit bien le terrible doute. Qui les empare sur notre capacité au-delà des éléments de langage et de la communication comme ça a été dit

S'il advenait que la CMP fasse évoluer différents articles et il y aura une responsabilité très forte d'ailleurs de nos collègues ici qui vont siéger en en CMP hein voilà c'est c'est c'est c'est je veux à nouveau dire que le travail de de la commission est déterminant mais que sur un certain nombre de sujets nos doutes sont grands. Je vous remercie. en fait les mêmes raisons que ceux qui vont voter pour et les mêmes raisons que ceux qui s'abstiennent. C'est-à-dire que en fait on sent bien le malaise de cet article hein les doutes qui s'inscrivent notamment sur la pratique avancée non pas la montée de compétences. Je pense que personne n'a envie ici en tout cas d'opposer les médecins ou soignants ou paramédicaux, c'est pas le sujet. favorables à cette montée en en compétence l'accès Direct de dans ce texte en fait pose beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétude et ça a été dit excellemment tout à l'heure, on vient de nous faire voter une dixième année supplémentaire pour dire qu'un médecin devait avoir 10 ans parce que le diagnostic est compliqué et c'est compliqué de faire un diagnostic

Doucement mais on l'entend quand même mais les IPA vont pouvoir être là là où il y a pas de médecins et ben non les IPA ne sont pas faites un accès Direct pour être là quand il n'y a pas de médecin alors elles doivent être là parce que ça peut améliorer l'accès aux soins, j'en suis perdent pas l'accès aux soins. Ça peut améliorer la prise en charge des maladies chroniques. J'en suis persuadé. C'est pour ça qu'on ne mettra pas un vote contre mais en tout cas en tout cas je pense qu'il y a une grande responsabilité voilà derrière ce texte et notre groupe s'abstiendra. Oui le groupe communiste républicain citoyen écologiste et pour l'accès Direct aux IPA et pour la primo-. Prescription là on l'a souligné, on l'a défendu lors de l'examen des différents Budgets de la sécurité sociale mais en fait on est très partagé parce que effectivement et je l'ai dit, mais Monsieur le Ministre, vous n'étiez pas pas présent et je ne vous en tient pas grief mais je je je je l'ai dit lors de de de mon intervention générale c'est que on est quand même dans un paysage qui est extrêmement inquiétant par rapport à la santé et au lieu de prendre la responsabilité de nous proposer une loi sur la santé. Une loi globale une loi avec ambitieuse. Hé bien vous soutenez en fait une PPL qui. N'est pas satisfaisante du tout parce que nous avons vu que c'est une loi fourre-tout. Donc vous ne réglez pas vraiment les problèmes, vous réagissez au lieu d'agir au lieu d'anticiper et c'est source d'inquiétude pour nous, parlementaires et donc on est partagé entre le vote favorable pour effectivement reconnaître la montée en compétence des personnels infirmiers des personnels médicaux, paramédicaux et on est aussi ben talonné par par par ce doute donc finalement. On vous répète une nouvelle fois qu'on aimerait bien avoir une réponse à notre question pourquoi pas d'expérimentation avant comme ça avait été voté ici même pourquoi vous vous précipitez dites-nous les raisons réelles et malgré tout ça, on va quand même voté favorablement pour donner un coup de pouce à aux infirmières et on vous appelle aussi, puisque vous leur demandez plus de responsabilités. Hé ben. Faites un effort au niveau salarial aussi pour revaloriser leur salaire. Je pense que ça contribuera plus d'attractivité. donc cet article. Le premier, même si à certains nombres de de voix donc de questions sont posées sur la table et je trouve que d'une façon générale ce. On a de nouveau dans ce sujet dans le traitement de de de ces enjeux là un vrai problème de méthode. On l'a évoqué lors de la discussion générale, on voit bien qu'aujourd'hui on vote ce texte dans une période qui est extrêmement compliqué alors que qu'créant notamment une rupture de négociations avec les médecins dans un calendrier qui n'est pas approprié. Et à travers ce texte là qui n'est globalement pas abouti pas suffisamment Putty beaucoup de questions restent sur la table, on arrive à opposer de tous les acteurs. On nous pousse les médecins avec le professeur de santé même parfois au sein même des ce problème de santé, on a des oppositions et lorsque vous vous avez l'occasion de rencontrer les acteurs de ces BTS sur le territoire. Celle qui fonctionne, on se rend compte que même au sein de ces BTS ça crée de la tension sur les territoires, alors que les choses ne sont pas clairement abouti et on arrive également à opposer le rural et l'urbain sur les grandes désertification de grands enjeux désertification médicale, alors qu'on devrait plutôt créer une dynamique globale pour essayer de trouver des solutions, donc un vrai problème de méthode et que à travers ce texte qui a été en partie corriger améliorer avec un équilibre trouvé par notre rapporteur, hé bien nous on a le sentiment quand même d'un chemin qui n'est pas aboutie. Donc c'est clair qu'à travers ces éléments-là. Vous évoquiez tout à l'heure le résultat de la commission mixte paritaire. Nous, nous serons d'une extrême vigilance et que les marges de négociation sont extrêmement limitées. Parce que vous avez bien qu'aujourd'hui on bascule entre on hésite clairement entre le fait de vous suit sur ces débats-là, le fait d'avoir donné de renvoyer la copie sur un globe Nous avons besoin aujourd'hui, une véritable stratégie d'organisation de la santé en France avec l'ensemble des acteurs, une vraie dynamique et de pas prendre les sujets morceau par morceaux, en opposant les uns et les autres. Merci monsieur le président, monsieur le ministre. Madame la rapporteure mes, mes chers collègues. Effectivement nous exerçons de métiers différents. Les infirmières sont formés aux soins. Nous nous sommes formés au diagnostic et surtout au diagnostic différentiel. C'est ça le coeur coeur de notre métier, c'est de ne pas se tromper dans le diagnostic, donc je salue bien évidemment le travail de de de Corinne Imbert la rapporteure. Mais je voudrais aussi qu'on réfléchisse à comment rendre notre médecine générale on sait que 25% des médecins ne n'exerceront pas la médecine, il faut la rendre attaque attractive. Est-ce que c'est en la bradant ainsi. Il nous faut 10 ans pour apprendre la vie et la mort. C'est 10 ans d'études, 10 ans pendant qu'on est jeune, 10 ans de sacrifice pour tout cela et ça s'apprend. Avec l'expérience, donc je voudrais aussi que nous soyons très prudents avec l'exercice illégal de la médecine et quelle sera la responsabilité de chacun. Quand ce ne sera pas coordonnée comme comme il le faudrait donc. Corinne a fait un énorme travail, mais moi sur ce cet article-là, je m'abstiendrai. Bien. Il y a plus d'explications de vote, nous allons passer au vote et je rappelle que. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions prévues par l'article 56 de règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. Votants 343 exprimés, 308. Pour, 287 contre 21. Donc l'article 1er est adopté. nous engageons la discussion sur le premier bis avec 2 amendements en discussion commune le premier lot 75 rectifié Monsieur Donc le. Le. Présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les infirmières diplômées d'État de prescrire des examens et produits de santé. j'ai cité dans mon intervention si vous voulez. Effectivement. Les les infirmières dans la loi, ont le droit de prescrire des produits pour des plaies chroniques. Mais si vous voulez dans les plaies chroniques, il peut y avoir au bout de quelques au bout d'un ou deux mois quand ça guérit pas ben c'est souvent une artérite où c'est souvent aussi une insuffisance veineuse grave qui est mal. Si vous voulez où il y a une grande tension qui a été mal fait et et donc je pense que c'est quand même pas mal d'avoir l'avis du médecin, merci. Merci madame la rapporteure. Excusez-moi, vous avez en discussion commune. Donc on a les 2 amendements celui-là et le le suivant le 69 rectifié. C'est vous aussi. Donc allez-y. Il est défendu. Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les dispositions de cet article vise à permettre aux infirmiers exerçant structures d'exercice coordonné et ayant suivi une formation complémentaire de prendre en charge de manière plus autonome. Les plaies. La surveillance des play-figure déjà pour partie dans le rôle propre de l'infirmier supprimer la possibilité de prescrire des examens complémentaires ou la soumettre à un avis systématique du médecin traitant d'viderait de leur sens, ces dispositions. La commission a cherché. À mieux les intégrer en prévoyant la consultation de la Haute autorité de santé sur la liste des produits examen dans la prescription est autorisé à la con en conséquence émis un avis défavorable sur ces deux amendements. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs dans le le cadre des. Aménagements de l'article par la commission. Même avis. Et puis en plus. Donc un double avis défavorable je les soumet aux voix donc l'amendement 75 rectifié qui est pour. Qui est contre.

Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Passons à l'article de avec un amendement le de rectifier madame de Doucen. Merci monsieur le président. Pour les mêmes raisons que la suppression de l'article 1, je demande la suppression, je propose la suppression de cet article de je vais pas reprendre. Les arguments mais surtout ne brade ont pas à la médecine. Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. La commission a a déjà cherché à mieux encadrer l'accès Direct en le réservant aux structures les plus intégrée et en limitant le nom maximal de séance en l'absence de diagnostic préalable à 5 séances. Dans ces conditions l'accès Direct et souhaitables pour faciliter l'accès au vaccin certes kinésithérapeute et libérer du temps médical la Commission émis un avis défavorable à cet amendement. Oui, monsieur le président. Même avis que la commission en remerciant le travail de la commission, en particulier pour avoir ramené de 10 à 5. Le nombre d'actes réalisés avant un avis médical. Donc un double avis défavorable, je le soumets aux voix qui est pour.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs au même titre que pour les orthophonie cet amendement vise à supprimer le conditionnement de la prise en charge de la consultation d'accès Direct du kinésithérapeute par le régime obligatoire d'assurance maladie au versement du bilan initial et du compte-rendu de soins au dossier médical partagé du patient si tenté qu'il en existe hein. Cette mesure risque d'entraver les les remboursements perçus par les patients eux-mêmes et donc nous sommes pour la je je je c'est le bon. J'ai dû me tromper pardon. C'était pas le bon. Christine militaire. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure effectivement, il n'est pas concevable au regard des exigences de qualité, de sécurité, continuité des soins que les patients qui n'ont pas bénéficié d'un diagnostic médical soit pris en charge par un masseur kinésithérapeute, en dehors de l'intervention du médecin dans toute équipe de soins ambulatoires et hospitalières comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un médecin qui assure la coordination de la prise en charge du patient et un protocole organisationnel. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la commission comme je l'ai rappelé tout à l'heure à déjà encadrer l'accès Direct en le limitant structures d'exercice coordonné les plus intégrée et en prévoyant que le nombre de séance de 20 ce qui n'été kinésithérapie sans diagnostic médical préalable ne peut excéder 5 séances. Dans ces conditions l'accès Direct au masseur kinésithérapeute. Est possible, souhaitable et fluidifier ira le parcours de soins. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le Ministre même avis Monsieur Prix. Même avis donc un double avis défavorable je soumets l'amendement voit qui est pour.

Alors l'objet pardon de cet amendement est mal rédigé donc je je je l'explique l'Arctique le qui autorise les ma soeur kinésithérapeute à procéder à des séances. En accès direct prévoit donc dans son la dernière phrase de l'alinéa que si le masseur kinésithérapeute ne transmet pas un compte-rendu au médecin traitant les axes sont mis à sa charge et donc nous souhaitons supprimer cette dernière phrase. D'abord parce qu'elle est imprécise de la locution mis à sa charge laisse un flou dans l'application, ça risquerait même d'entraver les remboursements perçus par les patients eux-mêmes et ce serait injuste. Par ailleurs, ce serait inéquitable car les fondements sur lesquels elle a été supprimée, à juste titre par la Commission pour les orthophonistes sont exactement les mêmes pour les masseurs qui n'hésitera peut donc outre l'imprécision précédemment évoqué la convention des ma soeur qui est une idée kinésithérapeute prévoit elle aussi d'ores et déjà. information du médecin prescripteur. Enfin, il ne semble pas opportun d'assortir l'obligation de coordination d'une sanction financière. Dans le contexte de tensions global avec les professions de santé. Nous demandons donc que cette sanction soit supprimée, je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cette sanction en ne on voit en effet un mauvais signal aux professionnels de santé ne paraît pas nécessaire. Nous l'avons déjà supprimé comme vous l'avez rappelé en commission pour les orthophonistes en conséquence et pour être équitable vis-à-vis des bien sûr kinésithérapeute. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement. commission de la Commission, monsieur le ministre. Oui, Monsieur le député, monsieur le président, pardon, excusez-moi. Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Jomier. Il est important, ça a été discuté à plusieurs reprises de s'assurer vraiment de cet exercice coordonné d'assurer du transfert des informations concernant le DMP ou plutôt devrais-je dire maintenant mon espace santé. Il faut quand même garder présent à l'esprit que 98% de nos concitoyens, donc certainement tous vous dans cette salle ont donné leur accord pour avoir l'ouverture de mon espace santé dans lequel il y a le dossier médical et dans lequel il y a. Les éléments du dossier médical de ce fameux DMP. Donc pour cela, le gouvernement reste favorable à ce que les informations circulent le plus possible dans le cas de cet exercice coordonné et donc insiste sur la mise en place de ces comptes rendus. Dans le dossier dans le cadre de cet exercice coordonné. J'aurais donc un avis défavorable. Donc un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Donc je soumets aux voix l'article.

oui parce que effectivement. Ça va dans le bon sens. Ça va permettre aussi de libérer du temps médical. Pour. Les médecins mais, mais. C'est vrai que la Commission dans son travail. A restreint le Champ de l'article. Puisque un certain nombre de professionnels qui ne sont pas dans. Les maisons de santé par exemple. Ne pourront pas. Avoir bénéficié de cet accès Direct et en milieu rural. Il est vrai que nous avons beaucoup de professionnels qui en fait vont chez les patients se déplace ne sont pas partie prenante d'une maison de santé en elle-même d'un centre de soins et donc ces personnes ben très concrètement sont exclus du bénéfice. De la mesure. Donc c'est un, un peu un peu dommage parce que je crois que. ça aurait permis sur le terrain d'apporter une vraie réponse là aussi de dégager du du du temps médical on s'est parfois il faut courir après l'ordonnance de renouvellement de soins liés la gériatrie ou est-ce qu'il y a besoin vraiment d'aller voir le médecin pour la lombalgie du lundi matin. Toutes raisons qui font que voilà cet article peut être dans la navette pourra là aussi. Je dirais les débats pourront se poursuivre parce que je pense que on se prive de de certains apports de professionnels qui du coup ne sont plus pris en compte dans la rédaction voilà donc oui mais c'était le sens de mon expression de votre monsieur le président. Merci Monsieur Lemoine. Madame Imbert. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mon cher collègue, c'était pour assurer notre collègue effectivement on a enlevé les, les communautés professionnelles territoriales de santé. Dans cet article, comme nous l'avons fait. Pour l'article 1er mais il n'y a pas que les, les maisons de santé pluri-professionnelles. Il y a aussi les équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés. Il y en a pas partout mais c'est facile à mettre en place parce qu'il suffit de 3 professionnels pour faire une équipe de soins primaires. Un médecin qui n'ait une infirmière et vous faites une équipe de soins primaires, donc je pense on peut encourager les professionnels à travailler comme ça au plus près du terrain souvent partageant une passion telle commune et c'est comme ça que la confiance s'installe peut qu'on peut travailler en confiance et de façon coordonnée. Voilà je voulais vous rassurer aussi sur ce point là. Bien merci. Donc nous allons passer au vote sur l'article 2. Qui est pour. Qui et contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Nous passerons l'article 2 bis. Avec trois amendements identiques de suppression. Le 1er défendue par Monsieur saumon.

car la pas suppose une vision globale de l'état de santé et pas seulement fonctionnelle, qui va bien au-delà des compétences donc de se le kinésithérapeute mais également une mesure du risque médical du patient que seul le médecin peut évaluer. Il n'en est bien sûr pas de même pour le renouvellement de la prescription initiale par le médecin le, le masseur-kinésithérapeute. Et son adaptation déjà prévue par les textes qui ne présente donc pas ces mêmes difficultés. Il est proposé donc de supprimer cet article. Oui, merci Monsieur le Président, nous avons déposé nos si elle n'a un article de suppression parce que les bienfaits de l'activité physique adaptée sont prouvé aujourd'hui de nombreuses recherches ont démontré. Que l'activité physique et sportive, on traite des bénéfices tant au niveau physique et physiologique que psychologique et social et permet de réduire la consommation de certains médicaments à Didier. Exemple, en cas 0. Outre la réduction de la fatigue lors des traitements, l'activité physique adaptée permet une réduction de risque de récidive, jusqu'à 24% dans le cas de cancer du sein et pourtant son développement est encore confidentiel. L'instauration de la prescription par le kinésithérapeute pour les personnes en affection de longue durée de cette à pas est une avancée de la reconnaissance de l'efficacité dans le cadre du parcours de soin néanmoins en l'espèce le texte stipule que l'activité prescrite par le kiné ne peut pas faire l'objet d'un remboursement dit des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale. Or l'absence de prise en charge financière représente un véritable frein au développement et à l'accès à cette à pas de plus, cette disposition introduit une différenciation entre la pas prescrite par des médecins qui peut être dans certains cas rembourser et là pas prescrite par les kinés qui ne peut faire l'objet de remboursement par la Sécurité sociale et cette différenciation est difficilement compréhensible et justifiable. Enfin, le texte semble permettre au au kiné de prescrire des séances d'appart qu'ils réaliseront eux- mêmes cette disposition contrevient aux principes déontologiques selon lequel on ne peut être à la fois et prescripteurs et effecteur de soins de santé aussi le groupe sert qui défend l'élargissement de l'accès pas. son inscription dans le droit commun. Doit demande la suppression de cet article. Concernant les kinés uniquement. mon. C'est le même article de suppression considérant effectivement qu'une primo-prescription d'une activité physique adaptée reste un acte plus globale en fait qu'une simple rééducation remise en mouvement et qu'il faut avoir une une appréciation fonctionnelle globale de la personne, donc il est plus adapté à la prescription médicale. Donc c'est pour cela que nous demandons la suppression de cet article. Madame Imbert. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dont trois amendements identiques de suppression. De de cet article alors. Ben on en revient à des problèmes de méthode. Monsieur le Ministre, c'est les c'est. Facilité pas le travail puisque la loi sur le sport de 2022 a déjà permis ou ma soeur kinésithérapeute d'adapter. Les prescriptions médicales de l'activité physique adaptée alors évidemment cet article qui s'inscrit dans la continuité en leur permettant d'en prescrire. La Commission a à mieux encadrer ses compétences en prévoyant qu'un décret fixera les conditions de prescription d'activité physique adaptée après avis de la Haute autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Ce décret pourra prévoir les conditions dans lesquelles une prescription par le masseur-kinésithérapeute est possible et celle à l'inverse, dans laquelle une évaluation par un médecin de l'état de santé du patient est indispensable. Il permettra la HAS. La Haute Autorité de Santé de se prononcer sur les bonnes pratiques en matière de prescription d'activité physique adaptée selon la situation médicale de chaque patient parce que bien évidemment. Toute la difficulté de ce texte. Nous ne souhaitons pas sacrifier. La la santé des patients et leur faire prendre de risques. Donc la la commission. Avait émis une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable sur ces amendements à titre personnel. Sagesse. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la rapporteure. Je pense que vous connaissez tous mon investissement dans le cadre de la prévention et dans le cadre du sport santé, bien sûr pour la prévention primaire, c'est-à-dire avant la maladie. Pour la prévention secondaire et tertiaire c'est-à-dire lorsque. Les patients sont malades pour éviter une aggravation éviter les récidives éviter des des complications. Dans ce cadre-là et cela a bien été rapportées. Nous avons dans la loi de de 2000, la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes. D'adapter la prescription d'activité physique adaptée en fonction de leur évaluation et ils sont tout à fait formé pour cela. Dans le guide d'utilisation de l'activité physique adaptée, qui a été validée par la Haute autorité de santé il est précisé que cette activité physique adaptée cette prescription doit être précédée d'un examen médical examen médical qui prend en compte bien sûr des antécédents du patient, son mode de vie mais surtout l'ensemble de la complétude. De son de son exercice. 2ème point également en fin d'année dernière comme je, mais il était engagé. J'ai mis en place une mission sport santé qui est dirigée par le Docteur de l'ordre et qui s'est entouré de sportif de haut niveau et de l'ensemble des spécialistes français du, du sport santé, cette mission me rendra ses premières conclusions au au mois de mars. En ce qui concerne l'état actuel de la prescription du sport santé, je rappelle que. Les lois précédentes avaient permis entre autres la création des maisons Sport-santé, nous allons dépasser 500 et pour bien apprécier quel est l'état de la situation et fera ensuite des propositions d'évolution. Sur la prescription de l'activité physique adaptée et du sport, santé et ce deuxième partie arrivera au mois de juin. Me semble donc prématuré d'avancer, de part l'attente des conclusions de cette mission d'expertise. Et puis par rapport à la raison de la nécessité d'avoir un examen médical préalable à la primo-prescription d'activité physique adaptée. Je le gouvernement est favorable à ces amendements de suppression.

le 1er c'est que l'article 2 bis telle qu'il est rédigé spécifiques. En cas de prescription par le masseur kinésithérapeute. Il n'y a pas de prise en charge par la Sécurité sociale. Qu'est-ce qu'un Français peut comprendre quand des actes qui sont jugés. Utiles pour la santé selon qui sont prescrits par telle ou telle professionnels sont ne sont pas prises en charge. Concrètement, le Français qui va avoir un médecin qui lui prescrit de la pas certes le le le le périmètre de prise en charge est restreint mais il aura droit à une prise en charge et s'il va voir un kiné parce que la loi l'autorise à avoir un kiné autorise le kiné à faire la prescription, ce sera pas pris en charge. À la crainte de la double vitesse là on ajoute une 3ème, une 4ème vitesse et ailleurs selon les territoires. Vous aurez le droit de la pas prise en charge ou non prise en charge. Donc il faut régler cette question là et la deuxième et que Prescrire est une chose est effectué. Ma collègue la la rappeler une autre, je le dis parce que on forme des étudiants dans la filière Staps. Ils peuvent faire une licence en activité physique adaptée, c'est-à-dire qu'on les spécialistes et ils sont formés pour faire de l'activité physique adaptée. Est-ce que les kinés vont adresser quand ils prescrivent vers ces jeunes professionnels conforme à l'activité physique adaptée ou est-ce qu'ils vont les garder pour effectuer eux-mêmes les actes. Moi j'aimerais bien qu'on nous le dise. Mais vous savez dans le système de santé, celui qui a les compétences les plus restreinte, il regarde toujours celui qui est au-dessus parce qu'il en veut un morceau mais regarde pas celui qui a des compétences encore plus restreinte que lui pour les lui transférer et ça c'est valable pour les médecins, pour les infirmières. Question des toilettes et là pour l'activité physique adaptée, donc, il faut préciser, il me semble. Ces points la prendre ce temps là et donc moi j'appelle clairement à supprimer cet article dans cet attentat. Bien, donc nous allons passer au vote, sur ces trois amendements de suppression avec un avis favorable du gouvernement et un avis. Défavorable de la commission mais avec une rapporteur qui. Donné un avis de sagesse. Donc. Nous allons voter qui est pour ces amendements de suppression. Qui est contre. Qui s'abstient. Donc ils sont adoptés. Donc il n'y a plus d'2 bis.

Oui c'était un amendement de repli concernant toujours l'activité physique adaptée, je vais pas revenir. Sur les bienfaits de de l'activité physique adaptée juste rappeler par exemple que. Cette possibilité donnée déjà depuis quelques mois hein puisqu'il y a une expérimentation en cours qui n'est pas encore évalué, mais j'ai pris attache. De spécialistes sur mon territoire. Et il a une formation qui est une l'exercice qui est actuellement en fait sur Linux, c'était de l'Oncopole de Toulouse et ou avec une association de la Camif, ils oeuvrent de concert pour mettre en place une activité physique adaptée pour les patients de l'Oncopole de Toulouse et après 6 mois d'accompagnement des patients l'hôpital on note que près des 3 quarts des patients ont diminué leur fatigue 2 tiers ont augmenté leur force de préhension et 9 à 100 sur 10 ont d'améliorer leur résistance et la souplesse de leurs membres inférieurs. 6% d'améliorer leur endurance aussi donc convaincu des des bénéfices de cette activité physique adaptée pour les patients et contraint par les règles de recevabilité financière nous avions déjà déposé au cours du PLFSS 2023 un amendement en ce sens. Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur l'élargissement possible donc de l'activité physique adaptée et sur son, j'allais dire son remboursement pour qu'il soit effectivement. Efficace. Peut être en en commission nous avait été suggéré de de le travailler au niveau du groupe de cancer mais je crois qu'effectivement c'est quelque chose dois travailler puisque on a la preuve vraiment avec l'INSERM aussi de l'efficacité de cette qui avait physique adaptée et donc des billets, le fait qu'elle pourrait amener donc du nécessaire remboursement. Merci madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je partage avec vous l'approche. C'est le constat fait de de l'apport favorable de l'activité physique adaptée pour les patients et notamment les patientes. Atteint de 2 cancers. C'est une demande de rapport, donc vous connaissez l'avis défavorable de la commission mais comme vous l'avez rappelé, comme je l'ai dit ce matin en commission, je pense que c'est un sujet qui pourrait être étudiée par le groupe cancer du Sénat si la la présidente le souhaite donc voilà ce sera peut être un sujet à à remettre en débat au niveau du groupe quand mais c'est un avis défavorable sur cette demande d'Europe. Monsieur le Ministre, prévoit déjà la remise d'un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie, des séances d'activité physique adaptée prescrite en application de l'article L. 11 72 Tiret 1 du code de la santé publique. Par ailleurs, je vous ai signalé l'existence de cette mission de Londres qui mettra de rapports ces rapports seront bien sûr à la disposition des parlementaires. C'est pour cela que considérant votre amendement satisfait. Je vous demande de le retirer. Madame Pumerole. Oui bien sûr, Monsieur le Ministre, je vais le retirer mais l'expérimentation. Je crois que droit doit durer 3 ans. Ce qui nous amène quand même après les JO et j'avais cru comprendre que le la perspective des JO permettez peut-être d'accélérer le mouvement et de dire qu'on aurait rapports plutôt pour pouvoir avancer sur ce sujet qui est. Je crois important. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. L'article 3 est consacré à l'accès Direct aux orthophonistes sans prescription médicale. Je vous rappelle, mes chers collègues, que les orthophonistes depuis 2013 ont une formation qui a été portée à 5 ans et qui donne accès au grade de master. Alors effectivement, favoriser l'accès Direct peut permettre une meilleure prise en charge des patients, alors qu'on connaît les difficultés pour obtenir des rendez vous chez les orthophonistes. Et d'ailleurs Monsieur le Ministre, je me permets de réitérer ma ma demande quand allez-vous enfin augmenter le quota des orthophonistes. Mais la rédaction actuelle limitant l'accès Direct aux structures d'exercice coordonné n'est pas satisfaisante et montre une méconnaissance de cette profession une infime proportion pour ne pas dire dire aucune orthophonistes n'exercent dans ce type de structure, on peut le regretter mais c'est un fait. Quand nous avons reçu en audition madame la rapporteure là la présidente nous a signalé qu'il y avait 25.000 orthophonistes dont 21.000 seulement exercer en libéral. Donc à Paris par exemple sur 750 orthophoniste si seulement exercent en maison de santé pluri-professionnelles. Donc on voit bien là que. Il ne faut, faudrait pas conditionner l'accès Direct à l'exercice coordonné parce qu'en fait cette disposition ne bénéficiera pratiquement à aucune de ces professionnels et elle risque par ailleurs d'induire des accès différenciés entre les patients selon leur lieu de vie. C'est pourquoi, monsieur le Ministre et mes chers collègues je je vous j'attire votre attention et je me permets donc cette intervention sur article parce qu'effectivement nous avions proposé un amendement mais malheureusement il a été retoqué. Bien merci madame Cohen. Donc nous passons l'examen des amendements l'amendement 22 de Monsieur Merci monsieur le président. Donc c'est un amendement effectivement qui relatif à l'accès aux orthophonistes. Madame Cohen parle très bien du département de Paris c'est une voisine et effectivement dans mon département, il n'y a quasiment pas d'orthophonistes qui exercent. Dans les structures type type MSP, et donc on voit que le cadrage qui est fait là pour les orthophonistes. Et trop restrictif. D'autant que c'est une profession qui est formé au diagnostic et qui est formé au traitement à la prise en charge ce qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est pas le cas. Des infirmières par exemple dont on parle donc cet accès aux orthophonistes il fonctionne depuis longtemps, il est. Formellement, il nécessite un transit par le médecin traitant mais tout le monde sait comment ça se passe le patient dit à son médecin, j'ai besoin d'une ordonnance que demande l'orthophoniste, le médecin l'a fait et leur Denis l'orthophoniste fait la prise en charge et l'orthophoniste a l'habitude de retourner vers le médecin traitant et d'envoyer le bilan ça fonctionne bien, donc j'ai été surpris que la commission je partage la suppression de la mention CPTS. Pour les autres, notamment pour l'article hein on l'a voté. Mais pour les l'orthophonie, je ne comprends pas très bien et donc je propose par cet amendement de revenir pour le coup, à la rédaction de l'Assemblée nationale, vous voyez on est on est très ouvert au au Sénat. Donc c'est de rétablir la mention la CPTS comme étant une des conditions de l'accès à l'orthophoniste. Voilà l'objet de cet amendement. Merci madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La commission effectivement après, c'est au contraire supprimer l'appartenance à une communauté professionnelle territoriale de de santé parmi les conditions suffisant à à autoriser l'accès Direct aux IPA masseurs-kinésithérapeutes. Comme aux orthophonistes. les les les les communautés professionnelles territoriales de santé de constitue pas une structure d'offre de soins. Je pense que vous partagez cet avis et ne garantissent pas un niveau de coordination suffisant entre les professionnels qui bien souvent ne ne partage pas une passion telle commune. J'avoue que j'ai hésité. Quand tu, quand j'ai j'ai supprimé la CPTS au niveau des des orthophonistes. Et j'ai aussi voulu le traiter de façon équitable. Tout en sachant que les enjeux d'accès Direct n'étaient pas les mêmes. Pour les infirmières en pratique avancée pour les masseurs kinésithérapeutes et pour les autres, les orthophonistes. Mais je l'ai traité de façon équitable parce que. Si j'avais voulu être cohérent jusqu'au bout, il aurait fallu qu'il y ait aucune coordination imposé. Pour l'accès Direct aux orthophonistes et là je me faisais rattrapé par l'article 40. Voilà c'est pour ça que j'ai supprimé aussi pour les orthophonistes. La notion de ces BTS donc c'est un avis défavorable à cet amendement. Santé. Monsieur le ministre. monsieur le président, Mesdames, et messieurs pour pour répondre sur les les orthophonistes. Le nombre d'orthophonistes elle est leur formation. Alors en terme de, de chiffres mais on parlera surtout en termes d'évolution, nous avions au au 31 décembre 2021. 24.208 orthophoniste dont l'immense majorité 20.657 exerçait en libéral ou en exercice mixte très peu en centre de santé 71 et un peu plus de 1000 en maison de santé, ce qui montre que les orthophonistes ont essentiellement un exercice isolé et pas encore dans des équipes, des Il faut noter quand même qu'entre 2012 et 2022 il y a une augmentation de 25% des effectifs d'orthophonistes donc un effort quand même important et que le quota en formation est passé de 800 à presque 1000 sur cette même période. Bien sûr, nous continuons à travailler sur l'adaptation des effectifs aux besoins. Je l'ai dit sur l'ensemble des professionnels de santé, ça concerne bien sûr des autres optimiste, les autres les orthophonistes pardon et et nous continuerons à à favoriser l'augmentation de ces professionnels, tant le le besoin est important au niveau de la population française. En ce qui concerne la notion de 2 CPTS alors vous savez comme moi que les CPTS sont de maturité différentes sur tout l'ensemble du territoire. Je me suis engagé également à ce qu'il y en ait, partout sur le territoire national pour la fin de l'année et je compte je compte suivent bien entendu cet engagement. Pour autant, j'ai eu la même. Hésitation. Que la rapporteur de la commission et et pour ce fait, je m'en. Je me range à la sagesse des sénateurs par rapport à cet amendement. un, je ré-insiste sur le fait que quand on dit par exemple qu'il a peu d'orthophonistes qui travaillent. Dans des, dans des structures. Que ce soit des centres de santé des maisons de santé que elles exercent de manière plutôt individuel majoritairement monsieur le mini j'attire votre attention sur le fait qu'on ne reconnaît pas leur statut, c'est-à-dire que on manque cruellement d'orthophonistes dans les hôpitaux, dans les CMP et pourquoi on manque cruellement d'orthophonistes alors que la l'orthophonie, c'est une l'orthophoniste. C'est une professionnelle qui intervient pour remédier en fait aux problèmes de langage, le langage dans tous ses états. Et c'est aussi au niveau neurologique par exemple et quand tu nous y sommes allés avec mon groupe, faire le tour de France des hôpitaux. Quand nous sommes allés visiter des services de neurologie. Quand j'ai demandé s'il y avait un manque de personnel en disant oh la la il manque des kinés et et quand je disais mais les orthophonistes parce que les orthophonistes si elles interviennent pas immédiatement face à une aphasie. Il y a une perte de chance. Qui pour le pour pour les patients et les patientes et on me disait on, bah on se débrouille. Donc Monsieur le Ministre, je vois que vous avez une attention particulière pour les pour les orthophonistes. Alors il faut que vous alliez jusqu'au bout, il faut que vous puissiez reconnaître leurs compétences et qu'elles aient un autre statut au niveau salarial dans les hôpitaux, dans les CMP et vous allez voir les orthophonistes vont aller travailler dans, dans ces centres et 2ème remarque c'est que même si elle travaille de manière isolée, elle travaille toujours. Comme l'a dit mon collègue, mon collègue Jo Jomier en lien vraiment de proximité avec avec les médecins à qui elles envoient leur bilan à la fin y compris leur compte rendu de enfin de de rééducation. Donc il y a pas de souci particulier avec les orthophonistes et c'est dommage qu'elle soit traitée à la, à la même enseigne. Parce qu'elles ont vraiment une, une compétence qui leur permet d'avoir un accès un accès Direct. Je suis Jomier. Merci. Monsieur le président. Alors effectivement moi moi j'ai eu la même réflexion que la rapporteure mais l'article 40 évidemment. À freiner de de la même façon et la même réflexion que que le ministre visiblement Corinne Imbert a soulevé une notion qui est importante, dit je veux être équitable. Être équitable cette juste ce n'est pas un principe d'égalité ou alors on va faire l'égalitarisme, mais les professions des caractéristiques différentes et ont des niveaux d'intervention qui sont différents et tout le monde reconnaît en tout cas lors des travaux en commission, tout le monde reconnaît que les orthophonistes sont une profession. Voilà qui est formé. Encore une fois à, à des prises en charge à des diagnostics. Comme par ailleurs les sages-femmes posent aussi ont des caractéristiques particulières. Donc les conditions d'accès, on est obligé. De les différencier. Si on ne les différencie pas alors là, on a entre dans un nivellement qui qui qui n'est pas souhaitable. Donc pourquoi cet amendement. Ben oui c'est un peu une cote mal taillée. On est d'accord, on est d'accord il ne respecte pas complètement le principe qu'on aimerait défendre mais le respecte mieux que la rédaction actuelle en tout cas et dans beaucoup de départements et le ministre a a a rappelé les conditions d'exercice des orthophonistes la rédaction actuelle amènerez en fait a très peu Donc c'est la raison pour laquelle cet amendement si je reconnais tout à fait qui n'a pas la pureté qu'on voudrait porter sur cette question-là permet au moins d'améliorer. Considérablement la situation. Ou une ce président que ce ministre. Je je souscris totalement aux réflexions et aux argumentaires notre collègue Jomier. Ce, ce métier d'orthophoniste est un métier. Singulier un métier important dans les réseaux de soins, notamment en direction. Des plus jeunes de nos concitoyens et vu la présence de ces professionnels. Libéral pour une grande partie puisque ce sont essentiellement des Dom. Présente au plus près de réseau d'écoles, notamment les plus rurales. Je crois qu'il est important qu'il puisse y avoir un accès Direct dans les conditions qui ont été évoqué effectivement avec les réserves de forme juridique ont été évoquée également par madame la rapporteure et et je pense qu'il est important que le texte puisse intégrer l'amendement proposé par. Le sénateur Jomier afin qu'il puisse y avoir un débat ultérieur et peut-être en commission mixte paritaire pour trouver une solution intelligente qui permettent effectivement de consolider cette profession très utile pour les réseaux de soins, notamment des plus jeunes de nos concitoyens. Donc nous allons passer au vote sur cet amendement. Donc il est favorable à l'amendement.

s'abstient. Il est adopté, il. Nous reste deux amendements. Identiques sur cet article 3, le 1er. Le 55 Madame Cohen.

dossier médical partagé qui est ouvert. la loi de 2019 offrent la possibilité aux patients en effet de refuser l'ouverture de de son espace numérique de santé toutefois la disposition ne peut se lire que comme visant les cas dans lesquels le DMP le Dossier médical partagé est ouvert ne pourrait pas être reproché un orthophoniste, me semble-t-il de ne pas avoir alimenté un DMP qui n'existe pas dans ces conditions, la commission a considéré que ces amendements étaient satisfaits sera donc une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable.

Donc ils sont retirés. Donc je vais demander. Votre vote sur l'article 3. Qui est pour l'article 3. Qui est contre. Qui s'abstient.

Si on continue. Ça ne va pas durer un quart d'heure hein. Donc je pense que c'est plus raisonnable de suspendre, je suis désolé mais. Donc on va suspendre la séance elle sera prise à 21h 30 pour la suite de l'examen du texte. La séance est suspendue.